La séance est reprise et la parole est au président rénale je suis saisi d'une de pardon, monsieur le président, excusez-moi. madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, donc c'est une information pour la mission suivante, donc c'est après la mission qui nous occupe, cet après-midi, nous aurons donc à examiner la mission Agriculture sur laquelle plus de 80 amendements sont déposés, compte tenu de leur gage la quasi-totalité de ces amendements sont en discussion commune, on a eu ce débat tout à l'heure avec l'amendement de Monsieur Sautarel en en effet, l'adoption de certains amendements sinon tomber les amendements suivants sans que les auteurs et même pu les présenter cependant suite aux échanges que nous avons eus en commission des finances, ce matin, des échanges qui étaient très simple, on a eu dans le la l'émission passé là hier par exemple, des espèces de tunnel avec en discussion commune des fois 40 30 40 amendements en discussion commune, ce qui fait qu'à la sortie, c'est arrivé sur santé par exemple,

et en même temps c'est notre manière de fonctionner puisqu'on est obligatoirement en discussion commune donc, afin de clarifier le plus possible de nos nos débats, je propose un lien évidemment avec la séance d'appeler par priorité, certaines de ces amendements pour les regrouper autour de 2 grandes thématiques que nous avons identifié de manière à avoir des débats organisés ben ça empêchera pas qu'on vote le vote se fera sur l'ensemble, hein, bon, donc on mettra un thème autour de la restauration collective et un thème autour des moyens de l'Office national des forêts, ceux-ci faisant de paquets extrêmement important dans l'ensemble, ainsi les rapporteurs et le ministre-pourront donner leur avis sur ces 2 ensembles d'amendements, j'allais dire de manière séparée que que les que les interventions se fassent de manière construite et que ce ne soit pas un peu un peu, passant d'un amendement à un autre, et donc d'une thématique à une autre, je vous indique enfin que plus nous terminerons tôt la mission RCT ça je ne peux pas m'empêcher évidemment cet après- midi, plus vite nous pourrons enchaîner sur la mission Agriculture dans le nombre d'amendements est particulièrement élevé cette année, c'est-à-dire qu'on a 2 missions avec beaucoup d'amendements et donc ça oblige à tenir compte dès maintenant, de ce fait et et donc comme d'habitude la m'excusant de le faire, hein, vous appelez à la sobriété dans la présentation de vos amendements pour laisser le temps de parole non pas ou rapporteur qui vont aller vite, mais à la ministre, pour qu'elle donne la réponse du gouvernement : voilà, je voulais vous dire en cet instant. monsieur le président, quel est l'avis du gouvernement sur cette demande de priorité, madame la ministre. Le gouvernement est d'accord avec monsieur le rapporteur. Hé bien, la priorité est ordonnée, alors nous reprenons la discussion de la mission Relations avec les collectivités territoriales dans la discussion, nous sommes parvenus à l'article 45 et nous avons une demande de parole de monsieur Laménie. Merci madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, messieurs les rapporteurs, chers collègues, alors cet article 45 concerne la répartition de la DGF s'était largement abordé aussi par tous les collègues en rappelant que la DGF fait partie des différents transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales, ces transferts financiers s'élèvent à hauteur de 107 6 milliards d'euros dans le PLF 2023, soit plus 1 virgule 7 milliards d'euros par rapport à l'année 2000 22 et s'inscrit aussi par référence à l'article 12 que nous avons étudiés en première partie, la DGF représente en 2022 26 8 milliards d'euros, dont 18,3 milliards d'euros pour le bloc communal et intercommunal et 8,3 milliards d'euros pour les départements, avec une hausse de 320 320 millions d'euros sur les composantes de péréquation de la DGF, dont 200 millions au titre de la dotation de solidarité rurale à noter également donc, cette réforme de la dotation de solidarité rurale, la réforme des dotations attribuées également aux communes d'outre-mer, augmentation de leur niveau, les modalités de calcul de l'effort fiscal et du potentiel financier qui sont aussi importantes, injustement des critères d'éligibilité d'éligibilité de la dotation politique de la ville, qui vise à soutenir les communes confrontées à des charges particulièrement lourde au regard de la politique de la ville, mécanisme de le de garantie également pour le fond, le fonds de péréquation

nous passons à l'examen de l'amendement 605 rectifier Monsieur Savary. Oui bonjour je présente l'amendement de Monsieur Mounier et que je soutiens bien volontiers, puisque le département de la Marne est concernée par un certain nombre de structures qui héberge des militaires, madame la ministre, de ce cet amendement propose de bien clarifier la loi par rapport à la prise en compte de la population malienne terre dans les casernes ou dans les centres de formation, qu'elle soit bien rattaché à la population au calcul de la population DGF de la commune, comme il est implicitement dit à travers les modifications au lieu entre 1999 et 2019 donc, cet amendement précise bien que les ces militaires rentre dans le cadre du calcul de la population DGF de la commune dans laquelle il réside.

simplement nous aimerions savoir si cette recommandation était techniquement envisageable et nous avons besoin de l'avis du gouvernement. Avis du gouvernement. Merci madame la présidente. Monsieur le sénateur Philippe mouiller sur l'amendement 605 vous proposer d'inclure dans la population des communes indicateurs prison. Vous proposez d'inclure dans la population des communes indicateurs pris en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement de l'ensemble des collectivités, les militaires vivant dans les casernes ou dans des camps et bases militaires, vous avez raison, les militaires qui vivent et travaillent dans les communes doivent être pris en compte dans le décompte de la population, utilisé pour la répartition de la DGF, c'est en fait déjà le cas, les militaires vivant caserne étant inclus dans la population des communes des communautés entre prises en compte dans le recensement de l'Insee, utilisé pour le calcul. Et la répartition de la DGF donc votre amendement est déjà satisfait, je vous demande de bien vouloir le retirer, autrement nous y serions défavorable. Merci, Madame la Ministre Monsieur Savary. Compte tenu des engagements le madame la mini-je retire bien volontiers l'amendement. Je vous remercie l'amendement 605 rectifier retirer 3 amendements identiques, le 231 pour commencer Madame Micouleau. Merci madame la présidente, cet amendement vise à intégrer la majoration de la taxe d'habitation, résidences secondaires dans le potentiel financier non pas en tant que produit mais en tant que potentiel merci.

merci madame la présidente, très rapidement, la, la taxe d'habitation sur la résidence secondaire est une des rares taxe sur laquelle les collectivités peuvent encore agir et percevoir des ressources parfois conséquente, le seul problème, comme cela a été indiqué précédemment, c'est que son régime et des incitatifs pour les communes, puisque une majoration de CHRS accroît le potentiel fiscal de la commune et a donc des conséquences sur les autres dotations, c'est la raison de cet amendement porté par mes collègues et moi-même. Merci, cher collègue, monsieur le rapporteur, avis de la Commission à Monsieur le Président, pardon. pardon. Rapporteur dans ce cas je suis rapporteur donc écoutez d'abord on, on voit que ces amendements sont largement cosigné donc on verra, mais je me lancer quand même dans une réponse avec plutôt une demande de retrait. Sur ces sur cela, donc il s'agit effectivement d'ajuster le mode de calcul du potentiel financier pour ce qui concerne la prise en compte de la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, alors il faut faut bien voir que, effectivement, la la fille 2022, mais c'est pas le seul cas d'ailleurs à intégrer cette recette au potentiel fiscal, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des éléments de potentiel et les éléments finalement de produits ce n'est pas le seul cas dans ce qui se fait aujourd'hui en terme de. De de fiscalité locale et et de comparaison de potentiel et sur différents l'évolution proposée ne semble pas opportune, bon, d'abord parce que, comme toujours, si elle est favorable à certains, elle va être défavorable à d'autres, ça c'est un 1er 1er sujet d'ailleurs, je suis pas toujours certain, quand je vois les noms de nos collègues que tout le monde soit bien dans le cas qui leur bénéficie pourrait y avoir des surprises, c'est-à-dire que si on si on voyait le résultat et si on faisait les les analyses, peut-être que certains des signataires

faire basculer, c'est-à-dire que la perte que d'un côté des certainement pas compensée par le gain de l'autre, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans les mêmes dans les mêmes échelle cantonne Nestor la RS bon le gain de THS est largement supérieur par rapport à l'impact que sur l'ensemble des collectivités que l'on peut avoir sur sa propre activité sur la une baisse de dotation ailleurs donc je pense que c'est pas dans les mêmes échelle et puis enfin c'est une, c'est un système qui est issue d'une délibération précise du comité des finances locales et donc moi j'appellerai plutôt au retrait en demandant plutôt puisque au CFL il y a des représentants de tous les territoires que ce sujet soit porté en CFL pour une éventuelle, d'éventuels chiffrage et une vision claire du sujet, je pense qu'on ne peut pas le faire, de mon point de vue, au détour d'un amendement, c'est un sujet qui peut être posée mais je pense qu'il faut d'abord le poser au CFL est plutôt ensuite revenir statuer éventuellement merci. Merci, monsieur le rapporteur, madame la ministre, avis du gouvernement. Merci madame la présidente. Monsieur le madame la sénatrice Micouleau donc simplement ne pas développé les mêmes arguments qui viennent d'être développées par monsieur le président président et rapporteur vous dire que l'avis du gouvernement, c'est une demande de retrait pour les raisons évoquées et sinon un avis défavorable du gouvernement. Merci madame la ministre, alors au vu des arguments madame Micouleau, vous, monsieur, je retire, vous retirez donc le 231 est retiré madame Joseph. Retiré pour le 319 et le 630 Monsieur Marie. Vous le retirer, je vous remercie et donc le 630 et retiré 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 230 rectifié madame Micouleau. Merci madame la présidente, cet amendement vise à ne pas flécher les 110 millions d'euros de DGF supplémentaires sur la seule DSR mais sur l'ensemble des composantes de la DGF. Y'madame Joseph pour le 317. Même argument donc défendu. Merci le 364 madame Monge. Merci madame la présidente, alors cet amendement propose effectivement de flécher l'abondement de 110 millions d'euros de la dotation globale de fonctionnement, non pas sur la seule dotation de solidarité rurale mais de manière équilibrée et équitable entre cette dernière et la dotation de solidarité urbaine, si nous nous félicitons de la décision du gouvernement d'abonder là de la DGF afin de permettre la hausse tant de la dotation de solidarité urbaine que de la dotation de solidarité, solidarité rurale à hauteur de 90 millions d'euros chacune le parti pris consistant à augmenter la seule dotation de solidarité rurale de 110 millions d'euros supplémentaires ne se justifie pas, en effet, cela entraînerait entérinerait un découplage inédit entre l'évolution de la DSU et celle de la DS et ce, alors même que précédemment, le législateur s'était employé ces dernières années à une augmentation identique des 2 dotations de péréquation, en effet, il n'y a guère d'éléments permettant de justifier un besoin de solidarité moindres envers les communes de banlieue principales bénéficiaire de la dotation de solidarité urbaine que de l'autre, dotation cet amendement qui fait consensus au sein de l'association des maires Ville et Banlieue de France a été suggérée par la métropole de Lyon et diverses communes autour.

pour laquelle il y a une augmentation de 200 millions prévu à l'alinéa 8 de l'article 45 lors de la de l'examen à l'Assemblée nationale, le gouvernement a prévu en fait que 60 % en moins de la hausse de la DSR sera affecté affecté à la fraction de péréquation, ce que je salue cet amendement, en fait, il est totalement différent des précédents vise à compléter cette répartition en fixant un minimum de 20 % pour la fraction cibles qui gère le rappelle et est amené à permettent de soutenir les communes rurales les plus fragiles, moins de 10000 communes sont considérés dans le cadre de cette fraction cibles et l'intérêt de la démarche est effectivement d'éviter, Madame la Ministre, que même si on on verse 60 pour la péréquation, hé bien cueillez peut être 35 % pour les bourgs centres et que ces 10000 communes en grande situation de difficultés ne se retrouvent qu'avec 5 % de 7 DSR voilà donc un amendement de répartition de répartition Merci madame Loisier et là, monsieur le rapporteur, vous pouvez nous donner l'avis de la commission sur ces amendements. Oui, effectivement, je pense que ce dernier amendement devait être avec, pour les raisons qu'a évoqué précédemment le le président mais bon en ce qui concerne les deux premiers amendements et d'ailleurs,

il est pas opportun de revenir sur cette mesure qui est très attendue par le monde rural et il convient quand même de rappeler que pour l'instant, la DSR cumulativement d'écart 1 milliard 9, alors que la DSU est 2 milliards 6 alors, c'est pourquoi je demanderai le retrait de ces amendements en ce qui concerne l'augmentation pour l'amendement 364 de la dotation de solidarité urbaine, ça ferait passer quand même non d'enveloppe de 90 millions à 200 ce qui est frais quand même un rythme de progression particulier pour la DSR, qui est déjà bien augmenté et, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure la la la DSU n'est quand même pas en mal de d'augmentation puisqu'elle est quand même toujours devant la la DSR même si on devait les comparer, donc ce sera également une demande de retrait. Quant à l'amendement 490 de Madame Loisier bon, cet amendement prévoit d'augmenter de 200 millions la DSR dont 60 francs 60 pour 100 fléché sur l'infraction péréquation par dérogation au droit commun, alors je voudrais simplement lui dire que, effectivement, on peut comprendre la la demande, mais de toute façon si on adoptait votre amendement ça enlèverait un un peu toute latitude au CFL qui a qui, normalement, on fait ce choix et en plus, en tout état de cause, il l'a toujours fait dans ce sens, on ne voit pas pourquoi il le le ferait pas, et dans la pratique, je voudrais vous dire qu'il est satisfait puisque on arrivera à cet effet, je regarde à cet égard. Les gens qui siégeait au CFL qui ont l'habitude de ce genre de pratique, c'est pourquoi je vous demandera retrait parce qu'il est, il est tout à fait satisfait d'avance. Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. Merci madame la présidente, donc une réponse pour les amendements 230 317 et 364 sur lequel la position du gouvernement sera un retrait sinon défavorable, en fait, pour rappel, l'article 45 du PLF prévoit que la hausse de la DGF en 2023 est réparti à hauteur de 200 millions d'euros sur la dotation de solidarité rurale, la DSR et de 90 millions d'euros sur la dotation de solidarité urbaine et de 30 millions d'euros sur la dotation d'intercommunalité cette répartition est calibrée de telle sorte que le maximum de communes voient leur DGF augmenter ou rester stable en 2023 je vous disais 95 % des communes. Je ne pense pas me tromper en faisant l'hypothèse qu'une très grande majorité de sénateurs ici présent souscrit à cet objectif, l'augmentation plus forte de la DSR que nous proposons, par rapport à la DSU permet également d'amorcer un rééquilibrage entre ces 2 dotations je rappelle en effet que la DSU est à la fois plus conséquentes et plus concentré que la DSR en 2022, elle représente 2 milliards 6 réparties sur 851 communes éligibles, contre 1 milliard 8 répartis sur 33000 communes pour la TSR et qui bénéficieront donc presque toutes de l'augmentation or Léo se passer de la DSI de la DSU ont déjà permis d'améliorer sensiblement la situation financière des communes bénéficiaires dont l'écart en terme d'épargne brute avec les communes de plus de 10000 habitants ne bénéficiant pas d'ADS U s'est resserré entre 2017 et 2020, malgré cette relative concentration des mesures nouvelles sur la DSR son enveloppe globale restera inférieur de près de 700 millions d'euros à celle de la Donc, nous vous demandons de bien vouloir retirer ces amendements, sinon le gouvernement prendra une position défavorable pour ce qui est de l'amendement 490 qui est portée par la sénatrice Anne-Catherine Loisier. Je voudrais juste m'appuyer sur la position du rapporteur simplement insister sur le fait que votre mesure aurait pour effet de réduire encore le pouvoir de la loi que le pouvoir de la loi confère au comité des finances locales de répartir la hausse de la DSR entre ces 3 fraction, seuls 20 % de la hausse prévue en 2023 pourraient être ainsi répartis par le comité des finances locales, donc notre avis est aussi retrait sinon défavorable merci.

donc je vais mettre aux voix le 364 qui est pour. Ah pardon, monsieur Delcros, explications de vote. Merci oui sur ces amendements, alors j'ai bien entendu que la métropole de Lyon proposez qu'on diminue quand diminue la part DSR finalement dans l'augmentation de la DGF à hauteur de 320000 millions d'euros, mais très franchement, les chiffres ont été rappelés et par le rapporteur et par Madame la Ministre, aujourd'hui, l'enveloppe consacrée à la DSR, qui, concernant la dit 33000 communes est largement inférieure à celle de la DSU donc vouloir avoir une augmentation symétrique ne correspond pas à la réalité des choses, donc je pense que il serait

de 2 Anne-Catherine Loisier je trouve qu'il a du sens parce qu'il vient parachever en quelque sorte, ce qui a été déjà fait sur la répartition des 200 millions puisque le 60 % pour pour l'appart péréquation a été acté et là il s'agit de cibler 20 % pour l'appart cibles. Si cher collègue Monsieur Bilek. Oui merci madame la présidente, il y a un an, dans cet hémicycle jeu proposé alors que le gouvernement a proposé 90 millions d'euros pour la DHR 90 millions d'euros pour la DHU, un amendement augmentant de 20 millions la dotation de été rural pour commencer au rattrapage, madame la ministre, vous avez ajouté un 0 à ma proposition de l'année dernière, dont je vous en remercie, mais je crois que c'était nécessaire d'un au rééquilibrage, vous l'avez dit, parce que un pauvre des Deschamps, hé bien il vont bien ne pas avoir des villes. Je vous remercie, monsieur Marie. Merci madame la présidente, nous ne soutiendrons pas cet amendement 364 à la fois pour les raisons qui ont été évoquées par le rapporteur spécial et et la ministre, considérant que les montants initiaux sont clairement différents et que ça pénaliserait la DSR or nous avons ici connaissance des difficultés qui peuvent être rencontrées par les communes, notamment au regard de ce que nous avons évoqués précédemment, l'augmentation de l'inflation et donc de leur charge, par ailleurs, cela pose toute une série de questions que nous évoquerons plus tard sur la somptueux Lisa la sanctuarisation d'une partie de la DSR effectivement en direction des communes rurales, alors qu'aujourd'hui, dans les commissions d'attribution, on constate un éparpillement de 7 DSR y compris au bénéfice de PCI qui n'en ont pas nécessairement besoin et donc je crois que il faudra revenir sur ces critères pour les resserrer au bénéfice des communes rurales. Si la parole est à monsieur le Président Longeau. le conflit qu'il pouvait avoir ou les divergences qu'il pouvait y avoir entre le monde urbain et le monde rural, je crois que si nous votions ces ces amendements, ben nous reviendrions à une guerre entre le monde rural et le monde urbain et je pense que le monde rural a aussi besoin effectivement qu'on abonde 7 DSR et donc je je pense qu'il ne faut pas voter ces amendements, il serait d'ailleurs important de les retirer. Merci madame pensez Monge. Puisque j'ai défendu cet amendement, c'est vrai que c'était tout simplement, on disait que la dotation supplémentaire devait être donné de façon égale ou de si l'objectif maintenant et la convergence des 2 dotation ben disons-le et on le fera donc en planification sur 10 ans puisqu'il y a un écart mais comme on n'avait pas perçu que c'était l'objectif, enfin les objectifs quoi ils ne sont pas transparents, c'est quand même un petit peu difficile de se déterminer, nous on pensait qu'on devait garder l'égalité de de la dotation ah bien sûr que comme il y avait plus de dotation pour le rural vous dit que c'est une demande pour diminuer le rural, mais au départ c'est pas une demande pour diminuer le le rural, c'est pour dire que les dotations supplémentaires doivent être répartis à égalité, alors j'entends sans être une grande spécialiste que vous êtes dans une trajectoire de convergence, bon bah alors si vous êtes dans une trajectoire de convergence si ça devient pertinent et en tout état de cause, pour ne pas quand même que vous puissiez alimenter la guerre justement des métropoles parce que moi j'ai, je vous rappelle que c'est plutôt des banlieues dont j'ai parlé, hein, alors la métropole c'est pas il y a de la pauvreté, il y a des besoins aussi dans la dans la métropole, donc je retire cet amendement pour pas avoir à une fausse interprétation qui est en filigrane de vous, de vos interventions. Merci, cher collègue, et donc le 364 et retiré le 490 madame Loisier. même l'impression que je ne vais pas leur retirer parce que moi j'entends votre argument madame la Ministre, qu'en fait, qui interdit au Parlement, enfin, qui suggère au Parlement de ne pas s'autoriser ce que vous-même vous vous êtes autorisés à savoir de pondérer l'affectation de la DSR, et j'insiste sur le fait que, il me semble absolument nécessaire de sanctuariser, en fait, la part qui reviendra au 10000 communes les plus défavorisées de France, je vous dirais que si nous ne votons pas cette répartition qui est dans le Champ de nos compétences légitime, hé bien je nous invite à nous retrouver dans quelques semaines après, effectivement, la motivation par le CFL et puis nous constaterons sont les 10000 communes les plus défavorisées de France. Merci, chers collègues, je vais donc mettre aux voix l'amendement 490 rectifié, je ne vois pas de main qui se lève, 490 rectifié, qui a reçu, donc un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est. Qui Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 489 rectifié, madame Loisier. Merci madame la présidente, madame la Ministre, donc à la suite de la réforme de la dotation d'intercommunalité, un mécanisme de lissage, a été mis en oeuvre afin de limiter, en fait, les variations individuelles à travers un tunnel de 95 garantie minimale et de cent dix hausse maximale, cette situation crée de fait des effets de transfert massif du secteur rural en situation cumulé d'écrêtement vers le secteur urbain en situation cumulé de garantie à titre d'illustrations pour les seuls EPCI de moins de 30000 habitants 125 d'entre eux, bénéficieront en 2023 d'une dotation d'intercommunalité inférieur à plus de 50 % de leur dotation théorique au regard de l'écart important qui existe entre leur dotation théorique et celle effectivement perdu perçu la mise en oeuvre de ce tunnel conduit à des situations préjudiciables pour de nombreuses EPCI ruraux ou périurbains, en effet, certains d'entre eux devront atteindre plus de 30 ans avant d'arriver à la dotation calculée selon les modalités, issu de la réforme et du tunnel, c'est pourquoi cet amendement propose de fixer le seuil d'écrêtement à 120 % du montant perçu l'année précédente, au lieu des 110 pour atténuer en fait cette cette situation sans remettre en cause l'architecture générale de la dotation ainsi ce seuil plafond de 120 est identique à celui en vigueur pour d'autres composantes de la dotation aménagement du bloc communal, tels que la DSR dont nous venons de parler pour laquelle le présent PLF a proposé de plafonner, pour le coup à 120 % je j'ajoute que, finalement, contrairement à ce que j'ai pu indiquer cette mesure aujourd'hui et et financée de par le vote de l'amendement 373 du Sénat en première partie, qui je le rappelle Index, l'évolution de l'enveloppe des 25 milliards sur l'inflation plus 4,2 % et donc qui nous amène à disposer de crédits supplémentaires passant donc de l'enveloppe supplémentaire de 320 à 798 je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, en même temps, j'étais en train de digérer la dernière phrase de madame Loisier que j'avais pas intégré dans mon raisonnement et qui me crée un petit doute, c'est toujours désagréable pour un rapporteur spécial d'avoir un doute, ce qu'on doit afficher des certitudes bon alors le présent amendement vise à faire passer de 30 à 61 millions d'euros, le montant de la hausse de la dotation d'intercommunalité élargir son tunnel d'évolution actuelles et caetera, qui passerait de 95 à 110 à 95 à 120 alors il est clair que plusieurs remontées du terrain, vous en avez eu, nous en avons eu évidemment montre que le plafonnement à 10 pour 100 ralentit fortement le déploiement des effets de la réforme de 2019 qui doit permettre de renforcer son caractère Equateur et de remédier à certaines des inéquité entre les différentes catégories de PC, nous avions d'ailleurs approuvé cette cette réforme lors de l'examen du PLF 2019 ce plafonnement à samedi pour % était intervenue en cours de navette par le biais d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale et c'est comme ça qu'on avait réduit ce qu'on alors bon, on peut dire plusieurs choses. D'abord dire que les dotations de péréquation cette année connaissent, on a eu ce débat est-ce que c'est trop est-ce que c'est pas assez, et caetera très bien trop, personne ne le dire mais est-ce que c'est suffisant ou est-ce que on doit faire plus, mais il y a donc une une augmentation de 320 millions d'euros dans ce PLF qui sont financées, c'est sa particularité par par Crédit frais, si on peut dire tout cas directement du gouvernement et non pas par minoration des dotations forfaitaires et donc qu'il couvait ne noter mais votre dernière phrase m'ennuie un peu, je dois le dire parce que je n'ai pas intégré dans mon raisonnement que cet amendement impliquerait de revenir sur ce principe, c'est-à-dire sur le principe de non-minoration des dotations forfaitaires qui est le principe posé pour les intercommunalités, autrement dit, si on applique votre amendement sur les intercommunalités, il y a bien une perception sur les dotations forfaitaires des comité pour financer cette augmentation de 30 à 61 millions d'euros, sur le principe en est donc défavorable, plus exactement, pour être plus positif, une demande de retrait et pourquoi je dis : demande de retrait parce que je vous demande de vous renvoyer, je me permets de vous renvoyer à 3 amendements identiques, qui sont un peu plus loin pour des raisons d'organisation de la séance,

prélève pas, si vous voulez sur sur le les dotations forfaitaires, donc on vous renvoie à ces trois amendements qui soit à peine un peu plus loin 131 429 626 sur lequel on donnera un avis de sagesse, si vous voulez bien retirer le vôtre, vous verrez qu'il porte sur des questions de similaire. Merci madame la présidente, donc on est sur l'amendement 489 modifié de la sénatrice Anne-Catherine Loisier en complément de ce que monsieur le président et rapporteur vient de développer je voudrais à la fois insisté compléter en vous disant les raisons pour lesquelles nous vous demandons-nous aussi de retirer cet amendement, à défaut, nous y serons défavorables, ces 2 raisons, la première c'est rehausser le seuil d'écrêtement supérieur pour le passer de 110 à 120 % aurait en réalité un effet modeste et contre-productif, cela pourrait, certes, permettre d'exempter le plafonnement 86 P. Si dont l'attribution augmentera déjà d'au moins 10 % l'année prochaine, mais 44 d'entre eux verraient leur attribution diminué par rapport à ce qu'ils auraient pu percevoir à droit constant en 2023 en effet, la dotation d'intercommunalité étant répartis à enveloppe fermée, accroître la hausse des attributions de certaines EPCI nécessite de diminuer celle d'autres The le 2ème, élément qui motive notre position, le gouvernement a déjà décidé par amendement au présent projet de loi de finances d'abonder directement de 30 millions d'euros, l'enveloppe de la masse à répartir au titre de la dotation d'intercommunalité en 2023 et non par redéploiement sur les composantes forfaitaires de la DGF comme appliqué les années précédentes, votre proposition priverait des une grande partie de l'abondement Direct. De la dotation d'intercommunalité par l'état de 30 millions d'euros, de vouloir retirer cet amendement, à défaut, nous y serons défavorables. Merci madame la ministre madame Cukierman, vous avez la parole. Oui, je vous remercie, madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, sauf si, bien évidemment, notre collègue Anne-Catherine Loisier retiré son amendement, mais si on nous le voterons moi je me permets à à ce moment-là de la journée quand même que nous ayons une petite réflexion, nous l'avons vécu avant la coupure déjeuner, je crois que nous avons un débat. Dans le cadre du projet de loi de finances, qui devient surnaturel et José espérer malheureusement que peu de gens nous regardent à cet instant là que peu de gens nous regardent, parce que nous avons quand même vécu avant la coupure, le fait de devoir retirer un abonnement et de ne pas le voter, parce que si nous le votions, nous pourrions en faire tomber d'autres qui qui eut été intéressant pour les collectivités, nous sommes là aujourd'hui à à cette heure-là plutôt à négocier, du fait de retirer des amendements pour pouvoir aller rediscuté ensuite et finalement les rendent plus effectif, alors je veux bien que nous laissions entendre que finalement les parlementaires que nous sommes, faisons tout et n'importe quoi avec des montants excessifs mais je veux et je veux le faire, y compris pour le compte rendu puisque les débats que nous avons sont rendus publics, nous sommes aujourd'hui. Des sénateurs contraints dans le cadre du débat de loi de finances sur un certain nombre de logique d'amendements qui nous oblige soit à l'écran, tu es à tel moment du débat soit allez gager de telle ou telle façon, ce n'est peut-être pas la meilleure des orthodoxies qu'il faudrait en matière de comptabilité budgétaire mais puisque nous ne sommes pas à Byzance pour discuter ici du sexe des anges, j'invite vraiment chacune et chacun a nuancé les arguments qui peuvent être données quand on compte les uns sont favorables ou défavorables sur tel amendements parce que on va finir la journée sur des rejets d'amendements qui simplement sont liées au fait qu'ils ne sont, soit pas bien cranté soit pas bien en oubliant comme ligne de mire l'intérêt pour les collectivités et les Français. Merci beaucoup madame Loyer vous maintenez votre amendement. Allez-y. Oui, d'abord je voudrais remercier le rapporteur, Madame la Ministre, pour l'explication apporter quelques éléments alors d'abord dans mon amendement initial, il ne s'agit pas même madame mamie, je peux, je voudrais porteur de prélèvements supplémentaires puisqu'au contraire, on le souhaitait, de venir abonder la dotation complémentaire des 30 millions mais de fait, comme je le signalais comme nous avons voté en première partie, un amendement qui élargit la masse disponible, hé bien ce supplément n'est plus nécessaire, donc il n'induit pas au regard de ce que le Sénat a déjà voté il n'induit pas de complément financier et enfin sur le fond de la mesure, c'est-à-dire une encore une fois une une mesure de justice financière puisqu'il s'agit d'établir un niveau de Crettenand qui est pratiqué pour un certain nombre d'autres intercommunalités et juste les effets modestes, non, non, non, madame, les Miss, moi je me suis j'ai pas j'allais dire un musée non mais en tout cas, essayer de faire la projection sur ce que ça donnerait sur un département comme le mien, à ce jour, seulement 2 EPCI sont au niveau de la dette de de la dotation théorique à laquelle ils pourraient prétendre avec ce système, à 120 % ce serait plus de la moitié des EPCI qui serait au niveau de la dotation théorique à laquelle ils ont effectivement droit merci. Donc vous maintenez votre amendement, vous mettez votre Non je je voudrais dire madame Loyer, que c'est une vision extrêmement positif que vous avez quand on a voté une augmentation des jets de 800 millions j'ai pas entendu le ministre au ban donné un avis favorable et levez le gage, j'ai pas entendu ça,

Merci, Monsieur Vial, vous avez la parole. juste un mot sur ce sujet, je je me rallierait à la sagesse de de la commission sur cet amendement, notamment sur le dispositif je j'entends ce que ce que vous dites avec ma collègue Gatel et et Kerrouche on fait partie des amendements que vous citiez tout à l'heure sur les vous avez donné un avis de sagesse et pour lequel je je vous remercie, néanmoins, il s'agit d'un vrai sujet, cette dotation d'intercommunalité c'est c'est la valise RTL, c'est la somme qu'on qu'on dit aux communes qu'elle pourrait gagner mais qu'elle ne gagneront jamais avec ce mécanisme, ça veut dire c'est c'est 30 ans pour l'obtenir, si tout se passe bien, s'y y a pas d'évolution, d'ici là je voudrais juste dire un mot, Madame la Ministre, et c'est pour ça que je voulais réagir en c'est en entendant vos propos tout à l'heure en disant que c'était un mauvais amendement parce que on, on, on y perdrait plus qu'on y gagnerait, c'est la la formule, je crois que vous avez utilisé juste vous rappeler, Madame la Ministre, que la moyenne de la dotation d'intercommunalité, c'est environ 22 8 euros par habitant, les communautés de communes les plus rurales touche en moyenne seize euros alors que les communautés urbaines sont à trente-quatre euros, madame la ministre, nous avions jusqu'à hier une ministre de la ruralité, je vous félicite pour pour votre promotion mais je je crois avoir compris aujourd'hui que nous n'avions nous avions perdu cette ministre de la réalité. monsieur Vial alors s'il n'y a plus de main qui se lève, je propose de mettre aux voix l'amendement 489 rectifié, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est.

Monsieur Buffet monsieur le Président, à vous la parole. Merci madame la présidente, cet amendement a trait aux critères d'accès à la fraction bourg, centre de la dotation de solidarité rurale qui ont été ces critères en partie cristallisée au 1er janvier 2014 je ne rentre pas dans le détail des communes qui continue d'en bénéficier, ce serait sans doute un peu surabondant au moment de ces débats, mais je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que, en se référant à la date du 1er janvier 2014 la loi omis de considérer la situation très particulière des communes situées en marge extérieure de la métropole départemental de Lyon, créée en 2015, ce qui fait que les périmètres de certains cantons limitrophes qui ont évolué au 1er janvier 2015, indépendamment de la réforme nationale de la carte cantonale, entré en vigueur en 2015, ont perdu le bénéfice de cette dotation, et l'objectif de l'amendement et de réparer une forme d'injustice. Merci, chers collègue monsieur le rapporteur. Oui merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, Monsieur Buffet, de toute façon la prise en compte du d'une date de référence pose forcément des des problèmes, nous en convenons mais c'est un sujet national, mais effectivement, vous évoquez une sorte de spécificité lyonnaise en la matière parce qu'il y en a d'autres bien entendu mais et cette spécificité justifierait donc pour vous un traitement particulier, comme nous n'avons pas pu l'établir, nous avons besoin de l'avis du gouvernement pour connaître la pertinence Madame la ministre, avis du gouvernement. Merci madame la présidente, monsieur le président, François Noël Buffet. Vous proposez d'apprécier les limites territoriales des cantons au 1er janvier 2015 pour les seules communes qui, sans appartenir à la communauté urbaine de Lyon, appartenait au 1er janvier 2014 à des cantons regroupant des communes membres de la communauté urbaine de Lyon vous indiquer que les communes chefs-lieux des anciens cantons ou qui, au moins 15 % de la population de leur canton au 1er janvier 2014 sont restés automatiquement éligible depuis lors, or cela n'est pas exact, le seul critère d'éligibilité à la fraction bourg, centre de la DSR qui a été figée au 1er janvier 2014 et le statut de chef lieu de canton en revanche même si des limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014, le poids de chaque commune dans la population de son canton est réévalué chaque année par ailleurs votre amendement crée une rupture d'égalité problématique. Il vise en effet apprécier les limites territoriales des cantons au 1er janvier 2015 pour les seules communes qui n'était pas membre de la communauté urbaine de Lyon au 1er janvier 2014 tout en appartenant à des cantons regroupant des communes membres de la communauté urbaine de Lyon, or les limites territoriales des cantons ont évolué en de nombreux endroits depuis 2014 en particulier mais pas seulement, lors de la réforme nationale de la carte cantonale de mars 2015 aucun motif d'intérêt général ne permet de justifier que soit introduite une différence de traitement entre les cantons de l'ex-Communauté urbaine de Lyon et les autres cantons qui ont connu une évolution de leurs limites territoriales depuis le 1er janvier 2014 il ne paraît donc pas possible de dégeler l'appréciation des limites territoriales des seuls cantons de l'ex-Communauté urbaine de Lyon, il ne me paraît pas non plus envisageable de dégeler l'appréciation des limites de l'ensemble des cantons, l'objectif du gel au 1er janvier 2014 étant d'éviter les effets de bord sur la répartition de la DSR, bourg bourg centre qu'entraînerait la prise en compte de la réforme. Cantonales de 2015, donc le gouvernement, une position soit de retrait si vous le voulez bien sinon défavorable. Merci madame la ministre, monsieur le rapporteur, même avis.

qui est celui de la création de l'armée. Métropole de Lyon il nous appartient pas ici de revenir sur la pertinence ou non, de la métropole de Lyon et donc vous faites un parallélisme des formes avec des cantons qui, certes, on était tous redécouper mais vous ne pouvez pas comparer un redécoupage dans tous les autres départements de France, qui ont qui ont prévalu au fait que vous aviez redécoupage avec évolution des EPCI et donc y compris des passages en communauté d'agglomération en communauté urbaine en métropole au sens métropole hors métropole de Lyon, si on peut les définir ainsi : je sais plus quoi j'en perds mon latin, parfois, y compris avec la situation très spécifique qui évoque notre collègue, président de la commission des Lois François-Noël Buffet. Qui demeure inévitablement le besoin d'une réponse exclusivement spécifique à la situation de l'ancien département du Rhône et au redécoupage des cantons du Rhône et à la création de la métropole du Rhône et vous ne pouvez pas avoir une réponse, Madame la Ministre, qui est un parallélisme des formes avec tout ce qui s'est passé ailleurs puisque par principe même partout ailleurs, nous avons. Certes subi le redécoupage des cantons certes subi le redécoupage des EPCI et l'intégration d'un certain nombre de communes dans des EPCI d'un niveau supérieur, sachant, sachant que, in fine, nous avons vécu quoi, ils ont vécu puisque la sénatrice libérale que je suis n'oserais surtout pas sa part s'apparenter au département du Rhône, et nous voulons bien garder nos différences, mais en tout état de cause dans le départ du tellement du Rhône il y a eu une évolution particulière qui nécessitent une adaptation de la loi pour prendre en compte cette spécificité, issu de la création de la métropole du Rhône dont j'inviterai simplement mes collègues dépositaire de l'amendement quand même à réagir parce que je pense que ce n'est pas qu'anecdotique, la réponse qui vient de nous être faite. Merci Monsieur le Président, buffet. Et madame la présidente, de remercier Madame Cukierman, je ne saurais dire mieux que ce qu'elle vient de dire Madame hein, la ministre il y a une particularité à Lyon la création de la métropole de Lyon en 2015, il lui a fait changer de nature, elle est de, elle est passée d'un établissement public de coopération communale à un statut de collectivité locale, dans ces conditions là les relations évidemment avec les communes directement limitrophes ont été profondément modifiés effectivement la situation est très particulière, j'en conviens parfaitement, elle est sans doute passé l'équivalent à n'importe quel autre sur le territoire national, elle est très particulière, qui la commune en question ou les communes en question se sont retrouvés avec une perte d'argent mené dont et trébuchantes alors qu'elles y sont pour rien, qu'elles ont rien demandé et qu'elle dépendait en réalité au départ d'une collectivité ou d'une commune principal qui est resté dans la métropole de Lyon, donc c'est bien à un moment, un ajustement qu'il est nécessaire de faire, à défaut de considérer que finalement les communes donc à s'appauvrir, mais là c'est un autre débat. Merci madame Di Folco pour explication de vote. Oui merci madame la présidente, je suis désolé de prendre la parole après le président buffet qui connaît mieux les choses que moi, mais, mais je voulais réagir en disant que, en fait, ce qui ça ce qui ce que nous étudions présentement, c'est en réalité un dommage collatéral de la création de la métropole de Lyon on pouvait peut être pas s'en rendent compte au moment de la fabrication de la loi, ça c'est clair, mais c'est en avançant qu'on apprend les choses et quand il faut faire des corrections, ben il faut être humble et se dire on a fait une erreur, on corrige voilà donc moi ce que j'aimerais simplement c'est que si monsieur le rapporteur veut bien m'entendre, c'est que, au vu des explications. C'est-à-dire que je voudrais attirer l'attention du rapporteur, c'est au vu des explications de Madame Cukierman et du président du fait au moins que monsieur le rapporteur, change son avis et émettent un avis de sagesse, ce qui nous permettrait de voter sereinement. Merci madame Di Falco, monsieur le rapporteur monsieur rénale. il y a des aspects comme toujours dans toute modification qui est faite, il y a toujours des choses favorables et des choses défavorables, donc je pense qu'il faut toujours avoir pesé les choses dans dans ces discussions-là et on ne peut pas dire. Que dans certains cas, on prend le côté favorable et que, pour d'autres choses, on souhaite vider le côté défavorable 2ème sujet : je rappelle simplement que si on ajuste comme vous le dites à enveloppe constante, ça veut dire que tous les autres perdent je le rappelle juste voilà donc au moment des votes vous voyez mais je, je pense que le sujet, métropole de Lyon, c'est un sujet très important qui a été menée qui a donné lieu à des discussions extrêmement forte, je le rappelle d'ailleurs

après on a été mis devant ce truc, il avait un accord, bon voilà, voilà, on a été positif, ce truc, mais après 2 grâce, il ne faut pas venir nous le rattraper et puis le reprendre sur tout le monde, voilà c'est mon avis. Merci monsieur rénale, alors s'il n'y a plus de demandes d'explications de vote, je vérifie quand même, hein, je vais mettre aux voix l'amendement 479 rectifié, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est. Alors,

Qui s'abstient, il est adopté. Six amendement faisant l'objet d'une discussion commune. Parce que le rapporteur. Avant de commencer la présentation de ces six amendement, monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous allons effectivement maintenant examiner plusieurs amendements relatifs à la réforme de la dotation de solidarité rurale proposée par l'article 45 cette réforme visant à remplacer le critère de longueur de voirie communale qui compte pour 30 % dans le calcul des fractions péréquation ici de la DSR par un critère de superficie pondéré par la population et la densité comme toute réforme des dotations, celle-ci fera nécessairement des gagnants et des perdants, ce constat est imposée, nous devons collectivement comme face à tout projet de réforme des dotations nous poser de questions: premièrement, la modification des critères est-elle juste et deuxièmement l'ampleur des transferts qu'elle entraîne est-elle suffisamment limité pour ne pas fragiliser les collectivités perdantes, s'agissant du premier aspect, les travaux du comité des finances locales ont mis en avance de bonnes raisons de ne plus utiliser le critère de la voirie en effet la dessert n'a pas pour vocation de compenser la charge particulière d'entretien des routes, mais les charges générales auxquelles font face les communes rurales, la longueur de voirie était utilisé comme un indicateur réputé entre autres refléter ses charges, or ce critère poser un problème puisqu'il introduisait un biais pénalisant comme une membres de communautés de urbaine ou de métropole qui était tenus de transférer leur route à l'Interco, c'est la principale raison pour laquelle le CFL a travaillé là une solution de remplacement, avec un critère plus général de superficie pondéré par la population dans cité par ailleurs le critère de voirie aurait tendance, assez paradoxalement, mais à favoriser les communes rurales les plus urbanisés. J'en arrive à la seconde question sur les effets concrets de la réforme, d'après les simulations présentées par le CFL qui a plusieurs fois à travailler sur ce sujet, les effets sont limités, s'agissant de la DSR péréquation la masse financière déplacer représentent moins de 2 % du montant global de la fraction s'agissant de la DSR cible, celle-ci représenterait 6 % du total fesses seraient en pratique inférieur, car l'article 45 propose en parallèle d'appliquer un tunnel d'évolution à la fraction cible en tout état de cause, il conviendra de relever que dans un contexte où l'enveloppe globale de DSR est en constante augmentation, les perdants ne seront en réalité que de moindre gagnant pour toutes ces raisons, la commission des finances n'a pas souhaité revenir sur cette réforme découlant expressément des délibération du CFL je demanderai donc en son nom, le retrait de tous les amendements poursuivant cet objectif qu'ils suppriment secrétaire ou en institut, d'autres où on en rajoute d'autres voilà je vous remercie pour votre. Merci, monsieur le rapporteur, nous allons pouvoir maintenant débuter l'examen de ces amendements en discussion commune en commençant par le trente-neuf rectifier terre monsieur Delcros. madame la présidente, madame madame la Ministre, comme l'a rappelé le rapporteur Charles Guené la question porte sur la répartition de la DSR non pas sur le montant de la DSR, mais sur sa répartition et seulement pour les fractions péréquation et cible. ça ne concerne pas du tout la fraction bourg centre dont on a parlé tout à l'heure actuellement cette répartition pour les par péréquation et cible repose sur 4 critères dont un critère de voirie qui n'est pas prépondérant parce qu'il n'intervient qu'à hauteur de 30 % donc il est loin d'être pro-prépondérant, même pas un tiers de la répartition se fait en fonction du critère longueur de de voirie, ce qui est proposé dans le projet de budget que nous examinons, c'est finalement de supprimer secrétaire de longueur de la voirie et de le remplacer par un critère qui qui prend en compte à la fois de la densité de la superficie, ce qu'on peut entendre, mais tout ça, pondéré par un coefficient de population, or les autres critères autres que la voirie aujourd'hui, autre que la longueur de voirie prennent déjà en compte le critère de population, je trouve que venir renforcer le critère de population dans le cas de la répartition de la DSR, ça me paraît être une mesure qui ne tient pas du tout compte de la réalité des territoires, la longueur de voirie, la longueur de voirie, ça fait partie des carafes titre des caractéristiques des des communes, ça fait partie des charges générales des communes comme ça a été exprimé tout à l'heure, nous savons que dans les communes rurales très faible densité de population, mais il y a souvent beaucoup de superficie et beaucoup de longueur de voirie, on en a parlé ce matin, à travers une proposition qui a été fait pour créer un fonds spécifique pour la voirie, on sait que c'est un sujet vraiment important et que les petites communes ont beaucoup de mal à faire face à l'entretien à la rénovation de leur voirie je défends cette idée que prendre seulement à hauteur de 30 % le critère de longueur de voirie, comme c'est le cas aujourd'hui, ça me paraît être le minimum pour tenir compte de la réalité de ce que vivent les communes rurales. Merci Monsieur Delcourt le 472 rectifié monsieur jeudi. Madame la présidente, madame le Ministre, mes chers collègues, j'dirais dans le sens des propos de Bernard Delcros, à l'instant, prendre en compte le critère de de de densité, et donc de population c'est d'une certaine manière, favoriser les communes les plus denses, donc les les communes les plus urbanisés, c'est, c'est une évidence, et d'ailleurs. Les chiffres des simulations nous le démontre, puisque globalement, les communes de moins de 1000 habitants sont perdantes, particulièrement les communes de 500 à 1000 habitants, parce qu'elle permet à la fois sur la DSR et sur la la DSR cible ADC péréquation et pour les moins de ça semble habitants le père sur la DSR cible péréquation pardon à peine compensée par la DSR cible donc, globalement, il y a une perte et qui est liée au au fait effectivement qu'on ne prend pas en compte les charges liées à la après dans la superficie et dont un critère effectivement qui permettaient de l'appréhender était le critère d'avoir correspondant et on l'a dit ce matin à de réelles charges, on va à l'encontre des objectifs de cette DSR, qui était de renforcer la péréquation et de permettre aux collectivités de disposer des moyens nécessaires pour faire face à leurs charges et faire en sorte que leur population soient traités de manière équitable, visiblement, et à travers les échanges qu'on a eu ce matin il y a un vrai besoin de réforme de ces dotations de rénovation d'un certain nombre de critères et qui permettent aussi non seulement d'avoir des objectifs, soit 2 objectifs d'équité mais également de lisibilité, on commence à se perdre et les simulations d'ailleurs et le rapporteur spécial l'évoquait tout à l'heure, les simulations

et généralement quand on fait des simulations, on le fait à périmètre constant, ce qui n'est pas le cas, et malgré tout il y a une perte pour les collectivités de moins de 1000 habitants dans les conditions que je viens d'évoquer, je vous remercie donc de leurs collègues ma demande de suppression. Alors, le 475 rectifié toujours identiques. Oui merci madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur oui il s'agit dans dans cet amendement de réparer selon moi une erreur commis le comité des finances locales dans le nouveau mode de calcul de la DSR en supprimant la référence le de voirie puisque ce comité de finances locales a voté à l'unanimité, apparemment la suppression sans la vie des maires ruraux, je le dis très sincèrement les maires ruraux souhaite conserver ce critère voirie parce que de toutes les communes, monsieur le rapporteur, non pas transférer la voirie aux communautés de communes et souvent dans les Budgets de nos communes rurales, la voirie, c'est le principal budget d'investissement et quand vous parliez superficie moi je connais des grandes communes où il y a que des départementales qui traversent donc finalement il y a pas de travaux de voirie mais il y a aussi des communes moins importantes qui ont 25 30 kilomètres de voirie entretenir et moi je trouve que la la DSR était un moyen de compenser justement cette possibilité de financer une part de une part de la voirie, donc je souhaite vraiment qu'on qu'on supprime cet alinéa pour qu'on revienne aux critères de longueur de voirie. Merci, cher collègue, le 724 monsieur bilingue. Merci madame la présidente, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par les orateurs précédents, mais il y a quelque chose qui me surprendre cette dotation est là pour compenser les charges, elle n'est pas là pour améliorer les recettes, or la superficie c'est une recette indirectement par le policier et les charges, le goût ne brûlera le c'est quoi, il y a 3 grosses charges qui caractérise les communes rurales, la première, c'est le Patrimoine souvent ces communes rurales foncier, je suis de la fusion d'anciennes paroisses et elles ont 5, 6, 7, 8 chapelles ou églises, elles ont 4 5 6 cimetière entretenir, c'est le Patrimoine, la 2ème, charge ces lois assainissement avec aussi des captages, 7, 8, 9, 10 captage des traitements d'épuration mais ça fait partie, où ça va partir sur l'et le 3ème poste important des communes rurales, c'est la voirie oui et on se supprime secrétaire alors monsieur le rapporteur, nous avons siégé côte à côte au comité des finances locales et je respecte et je connais très bien cette institution, je rappellerai quand même que sur 32 membres, il n'y a que 2 représentants des communes de moins de 2000 habitants.

Merci madame la présidente, madame la Ministre, la dotation forfaitaire des communes dans sa fraction péréquation et d'une grande importance pour nos communes rurales afin d'assurer des potentialités de fonctionnement des services pour des communes ayant peu de revenus et des bases d'imposition faible, le comité des finances locales a proposé de supprimer la composante voirie qui entrait pour 30 % dans le montant de la DSR et de la remplacer par une composante dépendant de la surface de la population et de la densité de la commune, relativement à sa strate cette proposition présente 2 inconvénients majeurs dont on a fait mention, je n'y reviendrai pas pour permettent de corriger ses défauts, le présent amendement élaboré en collaboration avec l'association des maires ruraux de France propose donc une nouvelle rédaction de l'article L 23 34 22 ans, remplaçant la formule de calcul de la DSR qui se base sur 3 points : 1er point la DSR seraient répartis pour 20 % de son menton proportionnellement à la longueur de la voirie, classé dans le domaine public communal en l'état la rédaction parle de charges de centralité la charge de ruralité existe aussi, il faut aider à la remplir aussi ma proposition vise à remettre cette dotation de voirie pour 20 % du montant de la DSR 2ème point elle sera répartie pour 20 % de ce montant proportionnellement à l'appart superficiel noté il serait dorénavant proposé de supprimer toute référence à la densité et de modérer la croissance due à la population et enfin 3ème point la suppression de la 4ème, composante superficielle de la DSR relatifs à l'écart entre le potentiel financier par hectare de la commune et le potentiel financier moyen par hectare, des communes de moins de 10000 habitants. Merci madame Noël et pour terminer cette série le 634 rectifié Monsieur ah non, pardon, chers collègues. Merci madame la présidente, cet amendement vise à intégrer un critère de taux de logements sociaux dans le calcul de la deuxième fraction de la dotation de DSR dites DSR péréquation en cohérence avec le même amendement portant sur la fraction dite bourg centre notre pays connaît un important déficit de logements sociaux, on le sait tous, et considérant et on considère que la crise économique et sociale induite par l'épidémie de Covid 19 va entraîner un besoin croissant de logements abordables pour nos concitoyens et donc il apparaît pertinent de récompenser les communes rurales qui prennent leur part de la solidarité nationale en produisant de tels logements ce critère de taux de logements sociaux, au regard du taux moyen de logements sociaux des communes de moins de 10000 habitants serait fixé à 15 % avec la possibilité qu'il soit minoré ou majoré de 5 points selon les règles de droit commun comme les autres critères

Oui, simplement, bon je je avais dit que je je demanderais simplement un retrait pour chacun des, des, des amendements mais simplement compte tenu de ce qui vient d'être dit, je voudrais quand même affirmé qu'il n'y a pas eu de coup de force auprès du CFL, je veux dire, le dossier était présenté plusieurs fois et avec des simulations, je veux dire, c'était quand même et et les maires ruraux, je suis au CFL, ils ont été invités, bon, cette fois, visiblement il ne semble pas avoir répondu à cette invitation, mais bon, on ne peut en être comptable, simplement il faut bien comprendre que, en fait, cette ce remplacement par un nouveau critère provient du fait surtout que tous ceux qui ont effectué un transfert de leur varie, en particulier dans les métropoles sont absolument pénalisée par le système et qu'il fallait trouver une solution,

de compenser les charges de voirie mais de compenser les charges de la ruralité en fête, hein, et donc il est apparu que la superficie et quelque chose, combiné avec la densité et bien sûr, pondéré par la population parce que quelque part on ne peut pas prendre que la densité permettait d'atteindre au mieux cette notion de de de charges pour la ruralité et c'est ainsi qu'on a retenu cela on est même allé, on a continué à majorer d'ailleurs pour les communes de montagne on a majoré de 2 fois par 2 fois la superficie bon non, non, mais il faut, il faut le rappeler, je veux dire, ça n'a pas été fait à l'aveugle et les simulations ont à appréhender tout cela et c'est pour cette raison que nous pensons que c'est un critère qui qui qui nous apparaît voilà, nous n'ignorons pas que nous touchons à la symbolique avec. Non, alors écoutez. Si les charges de ruralité se limitait à la charge de voirie, je pense que ça se saurait, mais le problème c'est de savoir si ça représente effectivement les charges de la rue, elle fait je crois que ça imposerait une réforme globale de la fiscalité et surtout de la DGF pour la rendre plus contemporaines et je pense que c'est là que devrait être notre travail, effectivement, je pense que la la réforme qui a été fait et probablement incomplète, mais il fallait bien retravailler cette notion, voilà, c'est simplement une explication complémentaire que je voulais dire.

et 74, donc certains des éléments que je vais indiquer rappelle un peu ce que vient de dire monsieur le le rapporteur en synthèse le PLF propose cette réforme à à la suite d'une délibération, vous l'avez compris du CLF et le gouvernement respecte sa décision, premièrement, deuxièmement, le critère de voir une. Excusez-moi, je n'entends pas ce que vous dites donc, je vous dis simplement notre position c'est de respecter la décision du CFL, deuxièmement, le critère de voirie ne pouvait pas être maintenus, transfert de voirie était obligatoire pour 1500 communes il fallait modifier ce critère, troisièmement le nouveau critère de spatialisation qui reprend une notion défendue par les sénateurs, Charles Guené et Claude Raynal et je salue leur travail qui est secrétaire de spatiale IT qui me semble effectivement plus moderne 4ème élément et on peut ne pas pas avoir partagé les mêmes convictions sans problème à population équivalente, une commune dont la superficie est plus grande sera plus aider et pour finir je vous rappelle et on l'a tous un peu, dit plus de 200 millions d'euros sur la DGF 95 % des communes qui auront une hausse de la DGF ou DGF identique, c'est l'année où il fallait le faire compte tenu de la crise. que le critère de voirie ne pouvait pas y être maintenu l'avis du gouvernement est donc défavorable merci. Alors merci madame la Ministre, alors juste vous dire qu'on a déjà 4 demandes d'explications de vote après la prise de parole de monsieur le président, rénale

voilà de condenser vos propos, ça nous permettra, peut-être, être de ne pas revenir en 2ème semaine donc on commence par monsieur Richard.

nos nos sont très proches et donc on peut, on peut se tromper d'abord intervenir en tant que président, alors on ne va pas s'affoler le le le le thème des collectivités locales au Sénat est un thème important et donc simplement on prévoit que samedi matin, on va se retrouver pour finir tranquillement je sais le dire quand c'est un peu non, non, je dis il y a aucune chance, voilà, il y a aucune chance, donc c'est pas la peine d'essayer de rentrer de toute force de temps qu'on n'a pas voilà et et je sais la passion de tous pour le débat sur ces sujets, donc pas de problème, donc je crois qu'on va se préparer et ce serait un miracle dû à la présidence d'arriver à nous rentrer là-dedans, donc je n'y crois pas beaucoup et il faut s'y préparer ce est pas une menace, et on aura beaucoup de plaisir à poursuivre ce débat

m'avait fait partager un certain nombre d'idées, moi ce que je crois surtout c'est que vous savez commencer et et c'est une, là c'est une application grandeur nature d'une part, on connaît le vote à la sortie, on n'est pas dans un débat sur le vote, sincèrement, on ne va pas convaincre l'Assemblée quasiment unanime de voter contre, donc de on sait lire des amendements et quand on voit qu'ils sont signés par tout le monde on on sait le traduire, bon, donc c'est pas le sujet de mon intervention, sujet de mon intervention, c'est que chaque fois qu'on modifie le moindre bout de quelque chose, hé bien, ceux qui sont

c'est aussi un constat : voilà, il faut se le dire, et c'est compliqué de faire de fonctionner comme ça, si on ne peut pas avoir des débats préliminaires pour essayer de trouver des solutions, bah c'est compliqué, ça va être compliqué, voilà et rassurez-vous, dès l'instant où on aura pris cette position, vous aurez le retour des maires concernés par ce qui avait intérêt aujourd'hui qui vous diront : mais qu'est-ce que vous avez fait, vous êtes revenu sur un accord, on est arrivé à peu près à trouver quelque chose, donc rassurez-vous personne ne sort gagnant de cette affaire, voilà tout ce que je voulais vous dire on gardera, parce que c'est la position de la commission, la vie de retrait, mais on ne regardera pas on se retournera pas pour voir comment la à quelle vitesse on est mis en minorité. Merci monsieur le président, alors Monsieur Richard. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Moi j'ai cosigné un de ces amendements, donc je voudrais très à l'aise, je le voterai et je voterai naturellement les autres également, qui vont dans le même sens, ce qui m'inquiète un peu c'est c'est la position l'exposé des motifs de ses demandes de retrait, notamment monsieur le rapporteur, vous avez justifié cette demande de retrait, Madame la Ministre, l'fait aussi par le fait que c'est le CFL qui qui auraient proposé ce nouveau dispositif de, de, de, de ne pas considérer que c'est une bible, donc on on a ici et le droit de voter autrement, surtout lorsqu'on examine pourquoi il s'agit, semble-t-il, ici, c'est ce que j'ai lu je lis de mieux corriger les situations pour lesquelles le critère de la longueur de la voirie crée des distorsions et si j'ai bien compris moi j'allais poser la question de savoir c'est quoi ces distorsions et si j'ai bien compris ce que nous a dit monsieur le rapporteur, ces distorsions toucherait essentiellement les communes qui ont transféré leur voirie ou métropole métropole permettrait de dire que je me pose la question de savoir si c'est toujours bien lié à la ruralité, tout ça, où sont les communes rurales, pourquoi ne tient-on pas compte plus des communes rurales enfin clairement la DSR, c'est bien cela, on nous a dit aussi, la DSR n'a pas pour objectif de financer l'entretien de la voirie, bien sûr, pas seulement mais la voirie, lorsque vous avez présidé aux destinées d'une commune rurale, vous voyez bien à quel point c'est important, on l'a dit ce matin on malheureusement, Stéphane Sautarel a retiré un amendement qui l'avait proposé que j'aurais d'ailleurs voté visant à créer un fonds spécial sur la voirie, alors Madame le Ministre, j'ai bien compris que, quel que soit le vote, ici on aura derrière 49 3 et on va pas discuter sans ans mais, Madame la Ministre, si vous m'entendez, il faut réfléchir à la possibilité de prendre en compte le critère de longueur d'une voirie d'une façon ou d'une autre un fonds spécial, si vous le voulez ou non mais c'est fondamental, c'est essentiel, les communes rurales en ont besoin, donc, indépendamment du vote il faut Madame la Ministre, que vous fassiez droit à cette demande légitime des communes rurales dans ce pays. Merci, cher collègue Monsieur Sautarel. Merci madame la présidente, madame la Ministre, alors j'ai j'ai j'ai fait grâce de mes 2 minutes de temps de parole puisque j'avais un amendement que j'ai retiré avant la séance qui étaient similaires à ceux de mes collègues pour renforcer le le poids de ceci, mais bien évidemment je, je, je soutiens la démarche et et j'espère que le débat permettra permettra effectivement, la voirie, hé bien un un poste de charges majeur dans les charges de la ruralité, ça a été dit, inutile de le de le rappeler et et j'espère que l'amendement que j'ai retiré avec difficulté ce matin mais mais j'espère qu'il sera dans une démarche constructive pour que nous puissions au cours de l'année 2023 bâtir une réelle réponse sur un fonds spécifique pour les communes rurales, au terme de la voirie, je veux aussi rappeler que tout ce qui touche à la spatialisation qui effectivement peut présente un intérêt me semble plus répondre à une préoccupation de ressources que de charge, c'est-à-dire que d'examiner à l'échelle spatiale par exemple la richesse pour corriger des écarts qui sont incompatibles avec la question de la population qui est pas en rapport avec certaines charges pourraient présente un intérêt, mais quand on veut corriger des postes de charges la voirie et le 2ème, le 3ème poste de charge d'une collectivité, donc je je je défends ces ces amendements et je pense que ça a opéré un transfert au détriment de la ruralité profonde de l'hyper-ruralité, de la vraie ruralité et qu'il serait dommageable de revenir sur ce critère, je vous remercie.

10 heures dizaines de morts suite à cet accident, l'Italie, la commission aménagement du territoire, la reprise de fin septembre, met en place une mission d'enquête sur les ouvrages d'art en France, certains d'entre nous, on faisait partie, a mis en fait les conséquences c'est que on a mis au pied du mur les maires ruraux en leur disant attention, suite à cette mission, vous avez des ouvrages d'art sur votre commune, vous en avez désormais la responsabilité et donc nous sommes un peu responsable de ça donc, indirectement, on a mis nos mères en disant maintenant vous vous avez la la réponse : c'est à vous d'agir et maintenant dans les critères, on va retirer le critère voirie, enfin à mon mes chers collègues, on marche sur la tête. Merci madame la présidente, d'abord, madame la ministre, une observation de forme, j'ai cru entendre dans vos propos que vous parliez de décisions du comité des finances locales, ce qui, moi, le comité des finances locales donnent un avis, les décisions se prennent ici, je crois qu'il faut le rappeler la deuxième observation. C'est que, on parle de ruralité. Une des caractéristiques de la ruralité, c'est un rapport particulier entre le nombre d'habitants et le nombre de kilomètre de voirie, si vous commencez par supprimer la voirie effectivement va difficilement parler de la même chose, la 3ème observation que que je voudrais faire c'est que. Les finances locales et sont quand même terriblement. Est ce que vous croyez vraiment que c'est le moment même si ça peut vous paraître finalement assez secondaire de faire une réforme que vous nous présentez comme une réforme technique mais qui n'est pas une réforme technique et l'un des collègues tout à l'heure à parler de réformes symboliques, je crois que le symbole a aussi son importance : je pense donc, Madame la Ministre, que c'est pas le moment de venir chambouler un certain nombre de critères laisser tranquille les mères en ce moment, ils aspirent à respirer et surtout que vous vous occupiez un peu moins de réglementer et un peu plus de les aider. aider. Nous avons encore six prises de parole et ça ne s'arrête pas, donc je laisse la parole à Monsieur. Et puis on si vous pouviez vous contraindre dans vos prises de parole, ce serait pas mal, merci monsieur n'. Merci madame la présidente, madame la ministre, tout d'abord une confession Digoin n'est pas une commune rurale et donc je ne siège pas dans un conseil municipal de communes rurales, mais j'ai présidé la communauté de communes du Grand charolais et lorsque nous avons réfléchi au pacte communautaire entre nous, nous avons tenu à intégrer la voirie comme compétence communautaire parce que c'est une compétence essentielle pour les communes et en particulier pour les communes rurales et c'est vrai qu'à la fois sur la discussion que nous avons eu ce matin sur le fond spécial voirie proposé par notre collègue Sautarel avec son conditionnement aux communes de moins de 500 habitants et réfléchissant à ce que nous avions fait localement, je peux comprendre les arguments des rapporteurs sur cette évolution qu'effectivement aujourd'hui cette voirie communale, aujourd'hui elle n'est pas forcément gérer tout le temps par les communes, elle peut être par l'intercommunalité et il est vrai que ça induit un certain nombre de différence de traitement d'un territoire à l'autre et donc je comprends tout à fait, ce qui a pu conduire à la réflexion préalable à cette proposition de décision, en revanche, madame la ministre. Après avoir salué votre nouvelle nomination avec vos nouvelles compétences. Permettez-moi de vous dire que si à la première journée de vos fonctions, ici au Sénat, vous commencez à nous expliquer que s'occuper de la voirie dans des communes rurales ce n'est pas moderne, je ne suis pas sûr que vous aurez un grand succès d'estime auprès de beau. Des maires ruraux parce que. Derrière votre argument qui était noté sur votre document préparé par vos services il y a effectivement cet argument qu'on entend partout et tout le temps que la voirie, ce ne serait pas moderne lorsque vous allez en commissions DETR et si l'on vous dit : on ne peut pas prendre les travaux de voirie, parce que ce n'est pas moderne dans beaucoup de départements ou de régions lorsque vous allez demander des subventions pour la voir et on vous dit ah ben non c'est pas moderne, il y a la transition écologique, il y a tellement d'autres choses à soutenir, et on ne vous donne pas de subventions pour la voirie, je crois au contraire que la voirie, c'est un outil essentiel pour garder de la modernité à conclure un cher collègue et donc au-delà du symbole, il y a également la ta grande sensibilité des élus ruraux et les habitants ses sujets, il faut absolument revoir votre copie, Madame la Ministre. Merci, alors Monsieur. Merci madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues, comme disait Fabien, jeune à l'instant, la voirie, c'est quelque chose d'important dans nos communes, tout simplement parce que c'est ce qui sert au déplacement à la mobilité, que ce soit individuel, que ce soit collective, que ce soit les déplacements doux, que ce soit tout en fait, c'est le lien entre la population dans les communes, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important et je crois que pour ce qui concerne la modification des critères des dotations, il faut l'effectuer avec beaucoup de précaution et ce n'est, semble-t-il, parce que ce qui a été fait en la circonstance, puisqu'on sait bien nous les élus, qui représente les territoires ici combien cette question de l'avoir, il est essentiel dans nos communes, moi je veux simplement dire que, au comité des finances locales, il a notamment été argumenter le fait que les élus dans nos communes seraient incapables de connaître la longueur de voirie, moi je trouve cet argument qui a été évoqué tout à fait anormal en tout cas je crois qu'il faut faire les confiance aux élus, ils savent de quoi ils parlent quand il gère les communes parce que ils sont près de, de, de l'argent des des contribuables et donc ils le font avec parcimonie, donc je, je dis simplement qu'il est important que en garde ce critère de la voirie dans nos le mode de calcul de nos dotations. Si Monsieur Pointereau puis Monsieur Delcros. Delcros. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, moi je vais vous dire je ne retirerai pas mon amendement, je sais pas ce que fera mon collègue Delcros parce que, c'est pas le comité des finances locales qui décide ici, c'est le Sénat, c'est là notre assemblée, le comité des finances locales peut donner un avis éventuellement mais il a pas décider pour nous,

et puis je pense que finalement il faut il faut vraiment que cette longueur de voirie soit reste un critère défini dans la DSR, alors je suis désolé, monsieur le rapporteur, mais je pense que, au regard de tout ce qu'on vient de dire, il est important de pouvoir conserver parce que finalement, comment faire simple quand on peut faire compliqué, c'est un peu salée, on veut changer les critères, mais ça va poser d'autres problèmes, où il y aura des effets de seuil, il y aura les les perdants des alors qu'on a un critère qui est déjà là depuis très longtemps, je pense qu'il faut qu'au vraiment conserver la longueur de voirie, merci à vous. Si Monsieur Delcros. Madame la Ministre, c'est vraiment à la ministre en charge de la ruralité, que je voudrais m'adresser au-delà du vote auquel nous allons auquel nous allons procéder parce que ce n'est pas par hasard si des voix si on débat d'abord longtemps sur sujet et si des voix s'élèvent sur tous les bancs sur tous les bancs du Sénat parce que évidemment il y a le travail du coup du comité des finances locales, je, je, je n'y reviens pas mais ce que vous entendez là c'est la voix des territoires, on est dans la chambre des territoires, ce qu'on fait remonter, c'est le vécu sur le terrain des sénateurs au quotidien tout au long de l'année dans leur territoire, et notamment dans les territoires ruraux et aujourd'hui. Le critère voirie c'est pas le critère principal de répartition de la DSR, c'est un critère parmi d'autres, même pas majoritaire qui compte à 30 les autres critères prenne en compte la population il y a 4 critères : si demain on remplace critère de la longueur de voirie par un critère qui fait encore entrer en ligne de compte la population, ça veut dire qu'on aura 4 critères fondés sur sur un la population et le potentiel financier, la population est l'effort fiscal, la population avec le critère qu'on fait rentrer, même s'il y en a d'autres, il y a la population qui intervient et et le nombre d'enfants entre 0 et ses armes, c'est directement lié à la population, donc on a un seul critère sur un sujet qui est majeur dans les communes rurales qui est la principale préoccupation des maires ruraux, on peut vous le dire, on le vit au quotidien, tout au long de l'année, donc s'il vous plaît au-delà du vote d'aujourd'hui, entendez-nous essayer de prendre en compte cette demande qui vous est faite, je pense à peu près à l'unanimité par le Sénat pour maintenir le critère de longueur voirie telle qu'il est aujourd'hui merci. Oui, madame la ministre de la ruralité, j'ai connu la DETR au départ, votée par enfin c'était essentiellement des communes rurales aujourd'hui dans mon département, 272 communes, 267 ont droit à la DETR, la dotation de solidarité rurale par ces nouveaux critères reviendra une dotation essentiellement pour les villes parce que c'est là où il y a le plus d'habitants, c'est là où il y a plus de jeunes, on fait des lois pour les territoires ruraux et on s'empresse dans le temps de les détruire, c'est inacceptable. Si Monsieur Madame Espagnac. Oui, madame la Ministre, moi je voudrais déjà vous féliciter pour votre nomination, je connais votre capacité des coupes et donc j'en appelle à vous parce que on parle de ruralité, on parle de montagne aussi, je donne un exemple : quand on est une petite commune en montagne avec 70 kilomètres de voirie, comment fait-on quand tu en effet on ne peut plus abondé sur la DETR même sur la réserve parlementaire, il fut un temps où on pouvait aider les communes sur la réserve parlementaire, ce n'est plus le cas, voilà donc moi j'en appelle à votre bon sens, je le connais et donc c'est pour ça que je me permets de vous saisir parce que il n'est pas possible aujourd'hui de soustraire ce critère qui est essentiel, voilà donc je certains de mes collègues, on a parlé par de critères de modernité, moi je vais vous dire vraiment, c'est un critère de sécurité pour les habitants, au quotidien, je rappelle que la montagne, il y a de la neige, il y a plein de choses, et nous avons besoin de de voirie qui sont en état et donc j'en appelle à votre bon sens merci. La parole est à Madame Cuq Hermann. Oui merci madame la présidente, madame la Ministre, simplement pour dire, et peut être sans surprise mais avec quelques explications que nous allons voter ces amendements, tout d'abord parce que comme je l'ai dit ce matin, la question de la voirie et. Tu intrinsèquement liées au développement, y compris des plus petites communes, et alors on peut continuer disserter. Sur ce qui est du fait d'être moderne ne ne pas être moderne, je vais le dire très tranquillement, ici parce que je pense que l'on peut me taxer de beaucoup de choses sauf être de celles qui ne défendrait pas les services publics demain mais il y a une réalité. C'est que le service public du transport collectif, madame la Ministre, je m'excuse, je le fais rarement mais juste si je vous dérange, vous le dites, c'est que à un moment donné, on ne fera pas du service public collectifs de transport de partout et dans toutes les communes et donc nous aurons besoin. De toutes les façons de partout, d'avoir des voiries de qualité pour assurer le déplacement et la mode mobilité pourquoi parce que nous avons collectivement un impératif qui est de tenter, non pas d'empêcher ce serait certainement trop orgueilleux de dire ça mais en tout cas de l'illimité demain l'aggravation de la fracture territoriale dans notre pays et j'oserai vous dire madame la ministre. ça ne va peut-être pas plaire à certains ici, mais vous savez, je me souviens il y a quelques années, Tous ceux qui ont voulu remettre en cause les critères territoriaux pour ne garder que les critères de population, ça n'a jamais été une réussite. Et ça n'a jamais été une réussite parce que ça ne répond pas à l'enjeu 1er qui est d'accompagner la vie des femmes et des hommes qui vivent et qui travaillent sur notre territoire, et je crois que c'est de cela que nous avons besoin comme leitmotiv, comme finalement phare pour nous guider et sincèrement oui nous voterons ça un moment parce que la proposition que vous faites n'est pas adéquate aux besoins des populations. Merci Madame Gatel vous avez la parole. Si madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, je suis désolée qu'on rallonge le temps mais nous on avait rien demandé, donc on aurait pu gagner du temps, si on n'est pas ouvert ce débat qui est quand même un vrai sujet, Madame la Ministre pardonnez-moi avec l'amitié que j'ai pour vous on ne va pas vous décrire ce qu'est la ruralité, vous en êtes encore si je filais parce que vous êtes encore ministre, bon on a un sujet très simple est-ce qu'on peut se parler en français, y compris au comité des finances locales, une dotation de solidarité rurale c'est une dotation de solidarité rurale la ruralité se caractérise par un habitat dispersé très étendu, parce qu'il y a des fermes et donc pour rejoindre la ferme au bourg, il y a des routes et que les routes sont extrêmement moderne puisque maintenant mais des unités de méthanisation dans les exploitations agricoles et il y a des camions qui doivent circuler il y a un seul critère sur la dotation de solidarité rurale qui est vraiment rural c'est la longueur de voirie, plus vous êtes petits, plus vous avez de la longueur de voirie : il n'y a aucune subvention sur la voirie, alors qu'on vienne bricoler un truc pour y remettent des habitants et de la densité c'est venir introduire ce que j'appelle un vice caché dans une dotation qui est clairement ciblé clair et que mes collègues l'ont dit aujourd'hui la voirie elles dépendent de la déclaration des élus ruraux mais Madame la Ministre, ils sont allés à l'école, les maires ruraux, ils savent mesurer une longueur de voirie et si l'administration n'a pas confiance, elle envoie un contrôleur. Alors en plus vous avez inventé un critère extrêmement compliqué, ça ne va pas, quant aux communes qui aurait confié la voirie en métropole je aurais pas de plus désagréable que je ne l'été mais les trains, les métropoles ont des dotations largement supérieur aux communautés de communes convient conviendrait de rééquilibrer, donc moi je pense que c'est tellement flou qu'il y a plusieurs loups dans cette affaire et qu'on gagnerait à rester là où on en été. Merci, merci, merci, chers collègue Madame Doineau. Merci madame la présidente, je voudrais tout d'abord saluer votre nomination, Madame la Ministre, et vous dire tout simplement, alors je sais pas si vous m'écoutez je voulais saluer votre nomination Madame la ministre et vous dire tout simplement que, il y a la France D RER mais il y a aussi la France des territoires ruraux et que pour faire du lien, nous avons besoin de bien et que, au détour de de de cette question, il faut vraiment changer les choses et revenir sur cette décision, parce que ça ne peut pas convenir au tout début, j'ai été maire d'une commune rurale et je sais combien ça pèse sur nos Budgets et donc n'enlevait pas ce critère, ce serait une abord une aberration merci.

il est défendu. Oui, pardon, cet amendement concerne l'éligibilité à la DETR, les communes sont, depuis, depuis qu'elle a été créée d'ailleurs, il y a un certain nombre de critères d'éligibilité à la DETR parmi les critères d'éligibilité, il y en a un qui concerne le potentiel financier pour être et léger pour une commune de plus de 1000 habitants, pour pouvoir être éligibles à la DETR, elle doit avoir un potentiel financier par habitant inférieur à 1 virgule 3 fois le potentiel financier moyenne de la strate et puis les intercommunalités sur monter en puissance ont été éligibles à la DETR, sauf qu'au au passage on on a, on a oublié quelque chose en route, si je peux dire, parce qu'aujourd'hui vous avez des intercommunalités des grandes comité d'agglomération de plus de 75000 habitants éligibles à la DETR pour lesquels on n'applique pas le critère du potentiel financier alors qu'on va l'appliquer à une commune de 2200 habitants, ça veut dire qu'on exclut des petites communes, d'un peu plus de 2000 habitants de la DETR au motif du potentiel financier alors qu'on explique en en applique pas ce critère pour des grandes Interco de plus 115000 habitants, donc, cet amendement, il vise simplement à corriger cette injustice et appliquer le même critère pour les grandes Interco que pour les communes de plus de 2000 habitants. Merci monsieur Delcros 637 monsieur Marie. Oui, nous venons d'avoir une très longue discussion qui a abouti, un vote quasi-unanime de notre assemblée pour préserver les moyens des communes rurales, hé bien, l'amendement qui est défendu la par mon collègue Delcros et et moi-même va tout à fait dans le même sens et et vise à restreindre l'éligibilité des EPCI à la dotation d'équipement des territoires ruraux en introduisant un un nouveau critère d'éligibilité, le présent amendement propose d'exclure les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1 virgule 3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des EPCI de leur catégorie, il s'agit ainsi d'appliquer à ces établissements publics de coopération intercommunale un critère de ressources qui serait proche de celui qui est déjà prévu pour déterminer les JT des communes tout en prenant en compte les différences de potentiel fiscal entre catégories de PC, c'est un moyen de resserrer ce que j'évoquais tout à l'heure l'éligibilité à la DETR des communes et des EPCI qui en ont le plus besoin, on y reviendra d'ailleurs dans de prochains amendements tout à l'heure. monsieur Marie alors, nous passons à l'avis de la commission et peut être avant que monsieur le rapporteur, nous donne son avis quand même vous dire que. Si nous continuons à ce rythme, donc la discussion s'arrêtera à 20 heures avant l'article 45 bis pardon et les amendements qui suivent, hé bien seront réservées pour examiner samedi. Voilà. Donc, au moins comme ça tout le monde est informé, donc maintenant, monsieur le rapporteur. Très bien, nous poursuivons sur un nouveau débat alors l'introduction d'un critère de potentiel financier pour le bénéfice de la DETR. de, c'est de faire en sorte que l'éligibilité des EPCI à la DETR soit tenus par un critère de potentiel financier, comme c'est déjà le cas pour les communes, pour la la commission, il nous paraît pas opportun de durcir l'éligibilité, la DETR, à plus forte raison s'appuyant sur des critères de richesse fiscale car si les indicateurs financiers sont évidemment indispensables faute de mieux, comme modalité de calcul de répartition des dotations de fonctionnement mais compte tenu de leur caractère très largement périmée, nous sommes plutôt opposés à un accroissement de leur influence sur les dotations d'investissement qui ne sont d'ailleurs pas ce sont des dotations d'investissement et il ne faut pas leur faire jouer le rôle de dotations de péréquation, c'est-à-dire qu'il y a un risque de mélange entre finalement la possibilité d'obtenir des des dotations d'investissement et d'autre part, le système de péréquation, je vous rappelle enfin que le préfet dispose toujours de la possibilité et je crois qu'il le fait de la possibilité de tenir compte de la situation financière des communes, entre autres, et donc des EPCI dans ses choix d'attribution, donc finalement ce que je veux dire que c'est que très souvent dans notre assemblée, on est pour la simplification pour trouver des solutions là encore proposé avec le rapporteur général permettant de trouver, avec peu de critères des solutions on vient encore une fois, rajouter du nous-mêmes un élément supplémentaire de complexité, alors qu'aujourd'hui le préfet et les commissions d'attribution en tout moyen de d'allouer sur les communes sur les EPCI dans le cas précis qu'en ont le plus besoin pour ce qui concerne la mienne, j'ai vérifié, c'est toujours le cas, c'est-à-dire que, on tient compte évidemment de la capacité de l'EPCI ou la capacité, évidemment, de la commune à financer ces investissements et on vient de voir donc venir rajouter des critères supplémentaires, je crois que c'est contraire à notre philosophie depuis toujours. Merci, monsieur le rapporteur oui. Dans la décision commune, il y en a, il y en a un deuxième et comme il il est pas écrit de la même façon, il revient au même principe donc, même réponse et demande de retrait. Madame la ministre, avis du gouvernement. Madame la présidente, je vous remercie donc sur ces deux amendements et en complément de ce que vient de dire monsieur le président et rapporteur, en fait, cet amendement pourrait conduire notamment à exclure, près de

Oui, juste un petit mot pour dire qu'il s'agit pas de créer un système supplémentaire, il s'agit d'appliquer aux grandes comité d'agglomération de plus de 15000 habitants, les mêmes règles qu'aux petites communes qui ont un peu plus de 2 1000 habitants, c'est tout, on invente, on en invente rien. Et effectivement, ça ferait sortir un certain nombre de PCI de l'éligibilité du coup ça reste ça renforcerait l'enveloppe pour les autres, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui pour les communes, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour les communes. Donc, vous le maintenez un monsieur d'elle qu'on est d'accord. Donc je mets aux voix. Il y a une explication de vote monsieur Non, à force de bloquer les choses et et de trop les contraindre le le risque c'est qu'on est moins Jean éligible que d'enveloppes et je m'excuse mais quand vous sortez, autant de PCI de la possibilité de la possibilité de l'éligibilité, vous avez tout simplement un risque à ce que l'enveloppe soit pas consommer ah je évidemment que ça existe, tu peux dire Renaud Bernard, mais c'est la réalité. Alors, s'il n'y a plus de demandes d'explications de vote, je vais mettre aux voix l'amendement. 209 rectifier, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté. Ah, on va recompter mais il faut bien lever la main parce que la très honnêtement, tout le monde n'a pas levé le bras donc on recommence, si vous voulez, qui est pour.

Qui est contre.

Merci madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, cet amendement vise à rendre les délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attribution du FPIC, il vise à favoriser le développement des modalités alternatives de répartition interne du FPIC au sein du territoire et en cela, cet amendement s'inscrit n'est-ce pas dans le droit fil des analyses développées notamment dans l'ex-Ceylan rapport sénatorial du 10 gainé Reynal d'octobre 2021 et intitulé pour un fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, plus proche des réalités locales, il existe 3 frein à une plus grande mise en oeuvre de répartition dérogatoire, mais j'ai vu, voici le détail en tout cas, cet amendement propose donc aux exécutifs locaux d'avoir la possibilité de faire en sorte que les délibérations puisse par tacite reconduction, demeurait valable tant qu'une délibération au contraire souhaité localement ne rendent pas caduc, qui conduit à ce que les délibérations ne soit plus fondée sur les des répartitions en valeur absolue mais sur des côtes par de répartition je précise amendements été déposés par Madame Micouleau. Merci monsieur Anglerre, le 318 monsieur Brisson identique. Oui, madame la présidente, c'est avant de vandalisme Joseph est identique à celui de Brigitte Bill Coulon étaient parfaitement défendus par Jean-Claude anglais. Merci monsieur Brisson le 468 qui est aussi un identique c'est Monsieur Bénard Roche qui le prennent. Oui, tout à fait je ne rajouterai rien à la démo la défense qui a été présenté. Merci, monsieur le rapporteur, avis de la commission. Bon, dans la réalité, comme cela a été cité, il y a un excellent rapport de mon collègue gainé de moi même donc je vous y renvoie et dans les préconisations nous préconisions ceux-là, donc on ne peut pas y être hostile, ça, ça va de soi, on y même on aura donc un avis de sagesse comme je l'ai indiqué tout à l'heure sur cette position, une sagesse assez favorable, cela étant dit, nous avons dit ça dans les objectifs, il n'en demeure pas moins vrai que nous avons un petit souci constitutionnel sur possible, en tout cas sur cette affaire dans la mesure où il y a le le le principe de libre administration des collectivités territoriales est apprécié de manière assez assez par le Conseil constitutionnel et il considère que il faudrait renouveler assez régulièrement le cet accord et non pas avoir une vision pluriannuelle de l'accord, donc il faut le savoir, c'est pour cela que nous donnons à titre nous nous pensons qu'il est utile de donner un signal positif à ces amendements et de le voter, et en même temps je sollicite, Madame la Ministre, pour savoir si elle veut bien au-delà de ça, et compte tenu d'un éventuel vote de notre assemblée, pouvoir s'engager à à travailler le sujet pour que, ils trouvent une solution constitutionnelle un peu plus, un peu plus solide sans doute que cet amendement. Il avis du gouvernement.

318 et 468 vous proposer de rendre pluriannuels les délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et des reversements au titre du FPIC afin de favoriser le développement des modalités alternatives de répartition interne du FPIC au sein du territoire si votre amendement peut permettre de concourir à une meilleure appropriation de la répartition interne du FPIC par les ensembles intercommunaux et de simplifier les procédures de répartition alternative du fait qu'il pourrait en revanche poser des difficultés dans des situations spécifiques en effet d'un exercice à l'autre en fonction de l'évolution des indicateurs financiers des territoires des mouvements du périmètre intercommunal, les montants des contributions et des attributions au titre du FPIC d'un ensemble intercommunal peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse, de même le contexte politique ayant prévalu à l'adoption d'une répartition alternative du FPIC et la situation individuelle des collectivités locales et d'un établissement intercommunal peuvent profondément changer nécessitant de revoir les modalités de répartition interne du FPIC dans ces conditions, il est préférable que les ensembles intercommunaux possède en amont tous les éléments nécessaires, y compris les résultats de la répartition du droit commun pour prendre une décision dérogatoire éclairé au demeurant, la procédure d'adoption relève du niveau réglementaire, je partage néanmoins l'objectif que vous recherchez demeure ouverte à approfondir la réflexion sur ce sujet pouvant aboutir sur une évolution des dispositions réglementaires régissant l'adoption des répartitions dérogatoire, comme l'a suggéré, monsieur le président et rapporteur. Donc ces retraits ou défavorable pour vous madame la Ministre, oui madame la présidente, merci, et pour la commission, une sagesse. Sagesse favorable de la commission alors je mais aux voit les trois amendements. Identique 229 318 468 qui ont reçu une sagesse favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ils sont adoptés le 586 Madame Cuq Hermann. Merci madame la présidente, Madame la Ministre je j'oserai vous dire que je suis un peu embêtée avec la présentation de cet amendement. Sans faire ici de la légitime qui et et revenir sur l'organisation de nos travaux, mais de fait, dès lors que les amendements précédents ont été adoptés, celui-ci pourrait devenir caduque, mais comme il n'a pas été cranté initialement sur les mêmes alinéa que les précédents et que pour autant il parlait de l'âme du même objectif qui est aujourd'hui de la question de l'évolution du FPIC et finalement de 100 nécessaire refonte pour pas dire de sa création absurde on son origine et de, comme toute création de départ qui porte en elle un pêché originel, peut toujours être corrigé mais jamais finalement répondre et solutionner. Ah la difficulté j'ai précisément précédemment déjà dit que j'en avais perdu mon latin, j'oserais dire maintenant qu'on pourra en perte son grec mais plus sérieusement, parce que je crois que depuis ce matin, nous sommes confrontés à une vraie difficulté, c'est-à-dire. Que nous avons un débat qui fait que les parlementaires que nous sommes sommes saisis dans nos territoires sur un certain nombre de problématiques que nous rédigeons et que nous déposons parfois, y compris en lien avec les associations d'élus, un certain nombre d'amendements que chacun va positionner là où il le seul à 800 pertinent et que nous aurions besoin, pour le coup, et j'ai aussi interpeller monsieur le président de la commission des finances. Parfois à des vraies discussions avec les auteurs des amendements pour voir comment est-ce qu'on peut les regrouper ensemble et avoir une discussion intelligente intelligible collectivement sur un sujet commun, tout comme à l'inverse, parfois on pourrait avoir une discussion intelligente intelligible pour nous inviter à repositionner des amendements pour s'empêcher que un amendement soit retiré parce que de fait, il pourrait faire tomber d'autres amendements qui ne sont pas sans rapport d'puisque j'ai utilisé mon temps de parole et je m'en excuse auprès de mes collègues, que personne n'a envie de revenir samedi matin j'économiserait le temps du président comme de la ministre, en retirant mon amendement, après vous avoir présenté, je vous remercie. monsieur le rapporteur, c'est un rédactionnelle. Le 1046 il est défendu, c'est un rédactionnel, madame la ministre, avis du Gouvernement favorable merci je mets donc aux voix l'amendement rédactionnel du rapporteur le 1046 avec un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté. Le six cent Merci madame la présidente, alors après avoir longuement et justement parler de DSR on va parler un petit peu de dotation politique de la ville, je rappelle que la dotation politique de la ville, c'est une dotation d'investissement qui est qui est versée aux communes qui remplissent simultanément 3 conditions : avoir avoir fait partie, au moins une fois au cours des des 3 dernières années des communes les mieux classés au titre de la DSU, présenter une forte proportion de population résidant en quartiers prioritaires de la politique de la ville et faire partie du périmètre de la politique de la ville, ce dernier critère est apprécié au travers de l'existence sur le territoire communal d'une convention pluriannuelle conclue avec l'ANRU au 1er janvier de l'année précédente, précédant la répartition, chaque année, plusieurs communes perdent leur éligibilité à la DPV en raison de la fin de validité de la convention qu'elles ont conclus avec l'ANRU et ce, alors même que perdure sur leur territoire des dysfonctionnements urbains que la DPV a pour vocation de contribuer à corriger aussi se présent amendement ce gel, donc la appréciation de l'existence d'une convention ANRU active sur le territoire communal au 1er janvier 2021, de sorte que les les communes qui auraient dû perdre leur le bénéfice de cette dotation politique de la ville en 2023 en raison de la fin de leur de leur convention rue demeureront éligible, si elles remplissent les 2 autres critères merci. Merci Monsieur Rambo, monsieur le rapporteur, vous savez la parole. Un peu. Merci donc le présent amendement vide vise à suspendre l'appréciation de l'existence d'une convention ANRU active sur le territoire communal au 1er janvier 2021 pour déterminer l'éligibilité à la DPV alors de manière générale on y aurait sans doute pas fait droit mais pour pour la période que nous connaissons un tel moratoire peut sembler opportun alors qu'une réflexion d'ensemble sur le zonage des politiques de la ville est à l'étude pour l'année 2023, mais on va évidemment, Madame la Ministre, pour nous confirmer que c'est bien le cas et que ça permettrait à ce moment-là, effectivement, d'attendre d'avoir les nouveaux zonage afin de relancer avant de relancer ceci et d'éviter que des pertes et comme une paire de la la DPV en attendant, donc on est un peu dans dans OK, quelque chose d'un peu particulier pour un moment particulier. Madame la ministre, avis du gouvernement. Merci madame la présidente, oui monsieur le président et rapporteur, c'est bien le cas avis favorable du gouvernement. Donc, avis favorable du gouvernement favorable de la commission, je mets aux voix le 689 avec ses 2 avis favorable qui. Pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté. Le vingt, il est défendu par monsieur le rapporteur. Un moment de coordination. Avis du Gouvernement avis du Gouvernement sur l'amendement de la commission favorable. Retrait sinon rejet s'il vous plaît. Demande de retrait sinon défavorable. Je mets aux voix l'amendement de la commission qui a reçu un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est. En ce. Je refais voter qui est pour l'amendement de la commission. Qui est contre qui s'abstient-il être adopté. 3 amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune 46 rectif. Merci madame la présidente, je défends un amendement proposé par notre collègue Borchio Fontimp et plusieurs autres sénateurs les critères financiers, fiscaux, utilisé pour le calcul de la dotation d'intercommunalité des EPCI à fiscalité propre ont été bouleversés par la suppression de la taxe d'habitation, évidemment, mais aussi d'une partie significative des impositions économique la plausible : suppression de la CVAE annoncé par le gouvernement vient perturber à nouveau les modalités de calcul de cette dotation pourtant ni les lois de finances pour 2021 et 2022, ni le PLF pour 2023 ne comporte de mesures de correction des critères financiers et fiscaux des intercommunalités, aucune mesure spécifique sur le sujet n'est énoncé cet amendement propose donc de sécuriser les impacts des dernières réformes fiscales sur l'ensemble des intercommunalités en leur garantissant de percevoir au moins 100 % de la dotation par habitant perçu l'année précédent précédent pardon en 2023 et 2024 ce qui leur permettra d'avoir un peu de visibilité et, je vous rends une minute madame la présidente. Si cher collègue, alors nous passons au 428 identique. Madame Gatel. Merci madame la présidente, donc les réformes récentes de fiscalité, taxe d'habitation CFE-était FB et demain la CVAE ont des conséquences sur les critères financiers et fiscaux pour le calcul de la dotation d'intercommunalité des EPCI pour neutraliser ces réformes fiscales sur les indicateurs financiers, notamment des officines il y a eu un groupe de travail qui s'est mis en place pour permettre

à fiscalité propre, il y en a 421 qui sont concernés par une garantie de dotation d'intercommunalité en 2022 dont 299 qui ont vu cette garantie enfin diminuer sérieusement ce qui fait une perte de plus de 6 1000000 560000 euros, donc ce que nous demandons par cet amendement et dans l'attente d'une étude d'impact approfondie, c'est de sécuriser les impacts des dernières réformes fiscales en garantissant de percevoir au moins 100 % de la dotation par habitant perçus l'année précédente, en 2023 2024, ça donne de la visibilité, Madame la Ministre, ça ne coûte pas un centime, je vous remercie. Collègue monsieur Marie pour le 600 vingt-cinq toujours identiques. Oui, c'est exactement le même, il a été élaboré avec l'AMF et donc il est défendu. Merci monsieur Marie je passe maintenant à l'avis de la commission sur ces trois amendements. L'avis de la commission aussi une demande de retrait sur ces trois amendements, alors quand je vois le nombre de signataires, je commençais à m'inquiéter.

que la dotation d'intercommunalité, fait déjà l'objet d'une garantie qui n'est certes pas à 100 % son montant ne peut baisser de plus de 5 % par rapport à l'année précédente, ce dispositif joue en pratique le même rôle que la fraction de correction pondéré par un coefficient dégressif mis en place, s'agissant des éthers comme en fait, c'est si on adoptait cet amendement c'est faire pour les intercommunalités, un système d'une garantie à 100 % qui n'existerait que pour les intercommunalités

2ème sujet ça coûte pas un Euro a dit Françoise Gatel alors à l'État, c'est vrai, mais aux autres PCI, bien sûr, ça coûte, c'est-à-dire que ceux qui gagnent, hé ben évidemment gagneraient moins

l'heure, je mets aux voix, pas d'explication de vote hein je mets aux voix les trois amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement ou retrait si certains souhaitent les retirer donc. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient ils sont adoptés. 3 amendements identiques qui font l'objet d'une discussion.

a pas. Moi je veux bien les faire revoter comme tout à l'heure, mais je vous garantis que ici on voit clairement les choses, il y avait massivement plus de voix pour que on. Alors je recommence le 131 rectifié bis alors c'est Monsieur Vial qu'il défend. Oui merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes, mes chers collègues, cet amendement concerne la dotation d'Inter communalité et revient sur le débat que nous avons eu suite à l'amendement de Madame Loisier tout à l'heure, c'est, c'est en fait la question de de la différence entre potentiellement et concrètement, on a un certain nombre de de communauté de communes qui, potentiellement, devrait toucher une certaine dotation d'intercommunalité en fonction de critères qui ont été fixées et concrètement qu'il ne la touche pas potentiellement certaines devrait toucher le double de ce qu'elles touchent réellement et concrètement, elle touche la moitié de de ce à quoi elles auraient droit, c'est donc une question de de justice que que d'essayer de de pallier à cela

des fleurs déplafonner ce ce rattrapage pour les communautés de communes rurales les plus fragiles et donc nous mettons des critères pour les communautés de communes de moins de 20000 habitants qui ont un potentiel fiscal par habitant inférieur au potentiel fiscal moyen et en faisant cela, nous permettons à à ces comités de communes les plus fragiles de pouvoir rattraper dès l'année prochaine la dotation auxquelles elles ont normalement le droit, mais qu'elle n'aurait concrètement pas si nous n'arrivions pas à mettre en place ce ce système de rattrapage ça ça concerne un peu plus de d'une cinquantaine de comités de communes donc c'est c'est un effort qui est somme toute modeste, mais qui est fait, c'est un un amendement de justice pour permettre à ces communautés de communes, de toucher plus rapidement la somme auquel elles auraient le droit. Ma solidarité à Cédric Vial qui a brillamment défendu les choses mais je voudrais juste rappeler un principe, c'est qu'un moment, on a évoqué avec justice et justesse la nécessité de faire converger les dotations selon les catégories d'interco, l'écart étant très important entre les métropoles et les communautés de communes, l'intention était bonne mais à un moment, le chemin est pavé d'un certain nombre de prise de conscience qui a fait que pour maintenir et ne pas pénaliser les métropoles dans leurs dotations en quelque sorte, on est venu pénaliser les plus petits et les plus faibles, donc nous en fait, c'est un effort de justice que nous demandons, encore une fois un rééquilibre au sein de l'enveloppe, je vous remercie. je souscris l'argumentation qui a été développé par mes 2 collègues précédemment, je n'ajouterai que 2 éléments tout d'abord quand on prend en compte les hypothèses qui ont été évoqués à l'instant à l'instant avec les données DGF 2021, il se serait 62, communauté de communes qui auraient été concernés, pour un montant total de 8 1000000 200000 euros en 2000 22 et et cette mesure, c'est le 2ème élément ne représente pas de dépenses supplémentaires pour le budget de l'État, car elle sera financée en une année par l'accroissement annuel de la dotation d'intercommunalité et de boulevard sera donc pas l'enveloppe de la dotation d'intercommunalité en 2023 et c'est donc une mesure qui va effectivement dans le sens de plus d'égalité et de justice entre nos intercommunalités en particulier à l'égard des communautés de communes. monsieur Marie avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, enfin je sais pas trop si ça vaut le coup, maintenant, de donner des avis. je le dis en toute tranquillité, hein, mais, mais non, mais à un moment donné, je vous le dis, il faudra regarder ce qu'on vote et en fonction de ce qu'on vote, faire la liste des intercommunalités concernées de part et d'autre, vous allez avoir des surprises non, non, ça ne marche pas mais c'est comme ça, voilà, mais quand même, je le dis donc, elle a la garantie à 100 % c'est ahurissant, mais cela étant dit celui-là, on était par contre sur un avis favorable le coup le hé oui, non, non, mais voilà, il faut savoir attendre les trucs là, là, effectivement, c'est une mesure d'égalité, là c'est une mesure en faveur des EPCI les plus les les plus

Merci, merci, monsieur le rapporteur, Madame la Ministre à vie du gouvernement.

petits un petit rapide message parce qu'on manque de temps, le dispositif est ciblée sur près d'une cinquantaine de communautés de communes à un coût estimé, comme ça vient d'être dit à 7,5 millions d'euros seraient directement imputés au sein de l'enveloppe de la dotation d'intercommunalité avec un effet d'éviction sur les autres EPCI des donc il faut nécessairement mesurer les conséquences, comme ça vient d'être dit, ce dispositif bénéficieraient à des EPCI dont la dotation augmentera déjà de 10 % en 2023, ce qui n'est pas négligeable, merci. Si Madame geste monsieur Villach. Merci madame la présidente, je voterai bien sûr favorablement, mais on vient de voir des chiffres édifiants, quand même, on ne vous avez expliqué durant des années et on continue à nous expliquer qu'il faut se regrouper parce que plus on regroupe plus on fait des économies d'échelle et plus les finales, je peux pas être avait rigueur et qu'est ce qu'on constate que ceux qui ont beaucoup regroupés ce comme beaucoup de population, ils reçoivent plus de dotation de l'État que ceux qui sont plus modestes taille alors là pardonnez-moi, je suis suis rural qui a pas fait de grandes études et j'ai de la difficulté à comprendre. Alors merci, monsieur Villach, la parole est à monsieur Richard. Richard. La présidente dans la Ministre, mes chers collègues, j'ai cosigné cet amendement et je m'apprêtais j'ai préparé un long travail à les défendre mais puisqu'on a un avis favorable du du du rapporteur et puis une sagesse du gouvernement, très franchement, je m'abstiendrai pour faire plaisir, précisément, monsieur le président de la commission rapporteur spéciaux. Ah. Merci monsieur Richard je mets. Donc, on voit les 3 amendements identiques : 131 419 et 626

Merci madame la présidente, l'article 250 de la loi de finances pour 2019 à réformer la dotation d'intercommunalité, cette réforme avait notamment pour objectif de supprimer les inégalités liées à la répartition des enveloppes distinctes par catégorie de le PCI ces derniers et un des hommes et des degrés d'intégration fiscale proche, hop, il existe cependant un frein à ce rattrapage qui râle un petit considérablement l'évolution de la dotation intercommunalité de certains EPCI notamment en outre-mer, cela est dû au système de plafonnement de la dotation n'était communalité un EPCI ne peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieur à 110 du montant perçu au titre de l'année précédente, ce plafond permet ainsi d'appliquer progressivement le montant de la dotation d'intercommunalité ciblés par la réforme de à chaque EPCI afin de ne pas déséquilibrer l'enveloppe globale de la dotation d'intercommunalité dans ces territoires d'outre-mer, 11 intercommunalité sont concernés par ce plafond en 2022, on constate que le montant cibles de la réforme de la dotation d'intercommunalité et parfois très éloigné du montant réellement perçu par les communautés, compte tenu de cette règle de plafonnement, afin de permettre aux intercommunalités d'autres maires de Guadeloupe, Martinique Mayotte Guyane et de la réunion de bénéficier justement de ce déplafonnement George Strait ses collègues que vous puissiez voter cet amendement pour un montant qui a de 13 1000000 421763 euros. Merci madame Jasmin, monsieur le rapporteur. Oui, ma chère collègue, donc il a plusieurs aspects mais effectivement faut votre amendement évidemment a été déposée avant l'acceptation de l'amendement précédent l'amendement précédent répond pour partie à votre souhait et comme nous sommes dans une vision sur ces sujets là une vision nationale là l'amendement que nous avons propos de déplafonner pour 2023 pour les communautés de communes de moins de 20000 habitants pour le montant qui a été indiqué, y compris, y compris outre-mer y compris, donc je pense que l'amendement en question correspond largement à à vos demandes et donc je vous demanderai le retrait pour votre amendement. Merci, madame Jasmin. Merci madame la présidente, donc je tiens compte des avis à la fois de du rapporteur et de Madame la Ministre, et je crois que ce sera suivi d'effet, effectivement, merci. Vous le retirer, je voudrais dire merci madame le 627 et retirer 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 492 rectifié madame loisir. Merci madame la présidente, madame la Ministre, donc la lignée à 42 du du présent article prévoit une neutralisation de l'effort fiscal uniquement cet amendement vise donc en fait à parachever la démarche du gouvernement et à étendre le Champ pour neutraliser l'ensemble des indicateurs financiers et ainsi éviter de pénaliser notamment les communes qui ont investi en effet, nous l'avons dit les réformes fiscales successives génère des effets de bord périphériques des effets de bord exogène, qui sont largement lié à la réforme de la taxe d'habitation et qui, de manière synthétique amène les communes situées dans un département impliquant un taux de TFPB plus faible d'être pénalisé en fait sur leur potentiel fiscal et des des effets également contre contre Peer Equateur liées plutôt à la DMTO et qui peut conduire à l'augmentation du potentiel fiscal d'une commune et donc la rendre ainsi inéligible à la fraction cible DSR dont nous avons beaucoup parlé du fait d'un effort d'investissements importants en 2022 on pénalise donc les communes qui investissent afin d'apporter de la lisibilité et de la stabilité au bloc communal dans un contexte financier que l'on s'incertain, cet amendement propose donc, dès l'âge d'élargir la neutralisation en dès 2023 à l'ensemble des indicateurs financiers je souligne que les départements de France ont procédé au même dispositif en sollicitant la neutralisation intégrale et pérenne des conséquences de la réforme fiscale sur leurs propres potentiel financier et j'ajoute que je me ravie que monsieur le rapporteur et déposé un amendement identique pendant la pause méridienne j'ai je j'espère que cela l'amènera à à donner un avis favorable à mon amendement.

Alors il y en a plus, en discussion commune, donc nous passons à l'avis de la commission.

à l'intégration de ces nouveaux indicateurs sur pour les ressources des des communes et il n'est pas sain de prolonger éternellement les choses et c'est une façon d'envisager un jour, quand même, de modifier la fiscalité locale si, mais si on ne tient jamais compte de ce qui est fait, on y arrivera pas, et ce que je voulais dire c'est qu'on ne peut pas mettre sur le même plan la réforme du du du potentiel financier simuler et adoptée notamment par le CFL avec celle de la réforme de l'effort fiscal qui est inscrite dans la loi avant même d'être simulée malgré le biais évident de la nouvelle formule qui exclut les produits intercommunaux, alors je voudrais attirer votre attention, c'est que votre amendement est incompatible avec l'amendement rédactionnel que je propose, madame Loisier hein, ensuite, et qui lui propose la neutralisation de l'effort fiscal, qui est donc à un très importante parce que ça sous tend l'ensemble du système, c'est la 2ème, raison pour laquelle je vous demanderai de retirer cet amendement, compte tenu de l'importance celui que présente la commission. Merci. Merci, monsieur le rapporteur, madame la ministre, un avis du gouvernement sur ces deux amendements. 492 Madame de la même façon que la commission, je vous invite à le retirer parce que nous porterons un avis effectivement favorable sur l'amendement suivant qui va être présenté par monsieur Gainey 47. Merci madame la ministre Madame Loisy. Merci madame la ministre, monsieur le rapporteur, juste une petite explication, donc en fait mon mon amendement propose la neutralisation de l'ensemble des indicateurs financiers je que propose exactement le vôtre, monsieur le rapporteur. Monsieur Cazeneuve et peut être avant en explications de vote, puis comme ça, monsieur le rapporteur pour répondent globalement c'est peut-être mieux. Merci madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues, effectivement, on voit bien que cette réforme des de la fiscalité locale est extrêmement difficile, en particulier lorsqu'il faut intégrer les critères de pondération mais là, manifestement, il y a une erreur du temps l'appréhension de l'ensemble des critères tout simplement parce que on a pris de nouveaux critères tenant compte de la suppression, notamment de la taxe d'habitation, bien entendu on a intrigué les les DMTO mais on n'a pas intégré dans la réforme, les effets du coefficient correcteur, or il paraît légitime puisque le coefficient correcteur a pour ambition de pouvoir corriger les inégalités, il paraît anormal que celui-ci ne soit pas intégrées dans le calcul des dotations et donc il est absolument nécessaire que celui-ci soit intégré, et que donc on remette à plat les l'ensemble du dispositif. Merci Monsieur Calvez, monsieur le rapporteur. Oui, simplement en réponse à votre demande de précision, le problème c'est que votre amendement neutralisent tout alors que celui de la commission fait neutre aller simplement les les deux seulement l'effort fiscal et fait tourner le système c'est pour ça que bon je je n'aurais pas toujours le même caractère d'injonction dans mes demandes de retrait, mais celui-là sera vraiment extrêmement gênant si jamais vous ne le retiriez pas et très honnêtement Alors je pense que chacun s'est exprimé Madame Loisy vous le maintenez nous le mettons votre. Vous le maintenez oui. Il n'a pas été discriminant pour les départements, je vois pas pourquoi il le serait pour le le calcul du bloc communal, donc je le maintiens. Merci donc je vais mettre aux voix l'amendement 492 rectifié, qui a reçu, donc un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, je me vois l'amendement 1047 de la commission présentée par monsieur Gainey qui est pour. Qui est contre, il est adopté. Le 491 rectifié, madame Loisier. la quête d'une meilleure justice fiscale entre nos collectivités selon nos projections, donc 2000 communes seraient de moins de 500 habitants serait ça déjà été évoquée serait impacté par une baisse de leur DGF et donc cet amendement vise en fait à créer un filet de sécurité DGF pour les communes de moins de 500 habitants en leur garantissant un montant de DGF 2000 23 au minimum égal à celui perçu en 2022. Oui merci madame la présidente, alors donc votre amendement en fait vise à introduire une garantie de non-baisse de la DGF pour les communes de moins de 500 habitants qu'on vient en 1er lieu de noter qu'une telle baisse devrait être rares compte tenu de la hausse de la DGF devant d'ailleurs bénéficier en 1er lieu aux communes rurales en second lieu, l'application du critère unique de population sans aucun critère de ressources ou de charges ne nous nous paraît un difficilement justifiables bon la Commission à privilégier d'autres dispositifs pour soutenir les communes face à la crise énergétique et avec un filet de sécurité élargi et simplifié, on on demande plutôt un retrait mais reconnaissons que l'amendement est très sympathique pour les communes de moins de 65. Car la. Merci monsieur Gainey avis du gouvernement, Madame la Ministre. Défavorable, madame la présidente. Elles on considère que la commission un avis de sagesse, si j'ai bien compris. Favorable retrait demande de retrait à l'heure, je mets aux voix le. 491 rectifié, qui a reçu une demande d'euros de retraits donc défavorable de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté. Je mets aux voix, l'article 45 qui est pour.

Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à corriger partiellement, tout du moins une inégalité en termes de dotations forfaitaires, dans le cadre de la DGF, vous le savez, le montant de la dotation forfaitaire varient du simple au double, selon la taille de la commune, on est à Soissons autour de 60 euros pour les communes de moins de 500 habitants alors qu'on est à plus de 120 euros pour des communes de plus de 200000 habitants et cette situation n'est n'est n'est pas justifiée il y a eu un, un rapport du gouvernement en 2019 qu'le reconnaissait, en disant, je cite : le poids des charges des communes de moins de 500 habitants semblent sous-estimer et donc si jusqu'à présent, le gouvernement a a reconnu que cette situation n'était pas satisfaisante, il n'a pas pour autant pris des mesures pour le corriger, il s'est même opposé à des amendements qui ont été adoptés en ce sens, précédemment dans dans dans cette assemblée, renvoyant toujours à des travaux ultérieurs qui n'ont jamais eu lieu et donc je dépose cet amendement qui a pour objet de de réduire l'écart qui, comme je le disais, est aujourd'hui de à de de le réduire de 1 virgule 5 à deux, c'est-à-dire que la dotation minimale passerait de 64 euros 46 à 96 euros 69, j'ajoute que c'est une année tout à fait propice pour le faire puisqu'il y a une augmentation de la DGF, donc ça permet de, de dégager des sommes pour donner un peu plus aux communes rurales sans pour autant retirer aux autres communes, je le dis parce que les autres années on nous opposait le fait qu'on allait dépouiller les uns pour améliorer le le sort des autres j'ajoute enfin que cet amendement était répond à une demande très forte et récurrente de l'association des maires ruraux. Si cher collègue, avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, cet amendement vise à modifier l'application du coefficient logarithmique à la population, c'est effectivement pour la, la première fois que nous le retrouvons lors de cette mission c'est vrai que bon, il est plus mesuré, puisque donc il dirait il proposerait de réduire à 1 5 cependant si s'il n'est pas parfait ce ce coefficient est encore le moins mauvais des systèmes, trouver ce jour dans la mesure où il est corrigé par bon nombre d'autres systèmes, et à ce moment-là nous retrouverions d'autres collectivités autour de la table qui viendrait demander l'application d'autres critères. Bon 13 heures très objectivement il ne paraît pas opportun de bouleverser, à ce moment, les équilibres de cette dotation forfaitaire qui est reconnaissons-le assez précaire et menacée d'obsolescence, hein, il faudrait vraiment remettre à plat, globalement la DGF sinon on sort pas en attendant, il faut reconnaître que la solution d'un renforcement de la DSR de 200 millions d'euros nous paraît constituer quand même à un instrument plus favorable, plus Direct et mieux ciblé pour le soutien à la ruralité que que que ce que vous demandez. Merci madame la Ministre. Demande de retrait pour les mêmes raisons que la commission bien avis défavorable, madame la présidente. La Ministre donc monsieur Moret, vous ne retirez pas votre amendement très bien je monsieur Maurer, explications de vote. Oui, juste pour regretter évidemment le la position du du rapporteur c'est jamais opportun, chaque année on nous dit ça et chaque année on nous dit : on verra plus tard, le gouvernement là il fait pas beaucoup d'efforts et justifie même pas, il dit défavorable, bon, d'habitude on a au moins désengagement de mise en place de commissions de travaux qui n'aboutit jamais, hein, mais au moins on on enrobe un petit peu le refus là c'est c'est rêves bonjour viennent d'être évoqués bah excusez-moi ces réseaux ne me paraissent pas bonnes et je je ne vous conseille pas ma mamie, si je peux me permettre de vous donner un conseil, d'aller porter ce message à l'assemblée générale des maires ruraux. Merci monsieur Moret, je vais donc passer aux explications de vote, en commençant par Madame Cuq Hermann. Oui merci madame la présidente, madame la Ministre excusez-moi messieurs, mais c'est un peu l'Arlésienne, donc je ne sais pas si l'Arlésienne est belle mais à force d'en parler tout le monde se l'imagine, mais personne ne l'a jamais vu, même pas touché et donc finalement, nous sommes là, c'est le principe de la légende messieurs mesdames. On est exactement dans la même situation ici, c'est-à-dire que chaque année, on parle de ça, de véritables réformes et du bus du besoin de revoir la répartition de la répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes rurales et les communes urbaines, c'est pas le moment parce que bien évidemment, ben oui, c'est pas à 17 heures alors qu'il faut qu'on ait fini la mission à 20 heures parce que sinon on doit tous revenir samedi matin qu'on va poser ici le débat, et donc c'est pas le moment aujourd'hui c'est pas le moment au projet prochain projet de loi de finances rectificative c'est pas le prochain et puis dans un an, on va se retrouver comme on s'est retrouvé l'année dernière, comme ça fait des années qu'on se retrouve en se disant que ce pas le bon, et pour autant, les inégalités, paradoxalement, elle, elle continue de se creuser et sans faire un fil conducteur de notre journée, Madame la Ministre, mais vous voyez, très simplement, si on reprend le pourquoi, finalement, de la différence entre les communes rurales et les communes Urban urbaine remontant aux années 50 60 de ces inégalités, oui, nous avions des routes communales qui n'étaient pas forcément entretenu goudronnées et etc, nous avons des problématiques d'eau d'assainissement qui n'étaient pas les mêmes, mais aujourd'hui on en est plus là et depuis ce matin, on en parle, par exemple, la question du kilomètre de dans les communes rurales, elle se pose de façon bien plus forte, hé bien plus indispensable qu'elle ne se posait précédemment et donc l'enjeu de la dotation, elle est indispensable, puisque depuis ce matin, on nous dit que c'est un vrai sujet, mais ça ne peut pas être pris en compte sur la création d'un nouveau fonds la création, l'augmentation de la DETR, la prise en compte dans la décision, donc ça peut jamais pris en compte et là il est 17 heures de ça peut toujours pas être pris en compte, nous personnellement, nous voterons cet amendement parce qu'à force que ce ne soit jamais pris en compte, c'est une réalité réelle au quotidien pour les élus.

je voudrais quand même rappeler qu'en 2021, le Sénat avait adopté cette disposition qui avait échappé à à l'Intelligence qu'on reconnaît, tous aux députés et que de la même manière, en 2019 Madame la Ministre, le gouvernement avait dit : ah, mais c'est bien sûr Free qu'on s'occupe d'une chose, c'est la distorsion de dotations entre la enfin, entre les communes selon leur taille, je suis d'accord, on ne va pas faire ça, autour d'un amendement, mais il faudrait quand même qu'on se demande pourquoi il y a autant d'amendements qui porte tout le temps sur le même sujet, qu'en même temps on nous dit : la ruralité, c'est très important et nous on dit : bah, donnons-leur un peu d'argent et tout à l'heure, il y a eu dans le texte, une proposition de revoir le le critère de de voirie en l'affectant davantage aux communes plus dense donc est-ce que sincèrement on peut se poser entre 2 PLF et prendre l'engagement de regarder avec courage au CFL comme au Sénat, ce sujet parce que ça devient fou parce qu'on répare, on rustines on sait plus ce qu'on fait et on invente des des usines à gaz, donc soyons sérieux Madame la Ministre, si vous voulez pas d'un amendement à 17 heures, mais nous, on a déjà voté il va peut-être être voté quand vous reviendrez nous voir l'année prochaine pour le même exercice, il y aura moins d'amendements viendra pas le samedi, et ce sera peut-être plus pertinent, merci. Monsieur du plomb, vous avez la parole. Madame la présidente, madame la Ministre toute l'amitié que je porte à Charles, je ne peux pas accepter le l'argument qui consisterait à dire : nous sommes conscients de la situation. Nous trouvons qu'elle n'est pas normal mais repoussant la plus tard parce qu'il est urgent d'attendre, ça moi, pour moi, c'est absolument pas un argument, je pense qu'au contraire. Cet amendement a véritablement de grands avantages, le 1er c'est qu'il n'a jamais été autant d'actualité qu'est-ce qui fait qu'une commune puisse par son budget, gérer convenablement l'amélioration du cadre de vie de ses concitoyens, c'est qu'elles aient suffisamment de ressources, je m'excuse mais ce gouvernement a supprimé une part importante des ressources qui pouvait être fait sur nos communes avec la suppression de la taxe d'habitation, alors vous allez me dire, elle est compensée, certes, certes, sur la base de 2017, à chaque fois qu'on a une augmentation de la population, on a plus l'augmentation de cette base et l'augmentation de cette taxe, donc par définition, si on veut revenir à quelque chose ou on est sur un système où on donne pareil à tout le monde sur 2017, par exemple pour la taxe d'habitation, hé bien il s'en est normal de faire la même chose sur la dotation globale de fonctionnement et le 2ème argument c'est que je trouve que cette année, il faut absolument le mettre dans la loi à la sortie du Sénat parce qu'au moins le gouvernement, en appliquant le 49 3 le 49 3 portera à lui seul la responsabilité de ne pas avoir pris cet engagement-là vis-à-vis des maires et il s'en expliquera puisque, dans le 49 3 vous avez la chance de pouvoir décider seul de ce que vous gardez de ce que vous enlevez ou de ce que vous pouvez reprendre hé bien en le votant on vous permettra de vous décider et on jugera derrière. Il me suis du plan, la parole est à monsieur Merci madame la présidente, chers collègues, Madame la Ministre, effectivement, à 17 heures, je ne sais pas, peut être le moment par un amendement de modifier, mais il y a des années que nous, elle, dans le fond, cette différence de traitement financier au niveau de la DGF avec en rural qui vaut la moitié d'un urbain, c'est quand même surprenant alors que Chawn mairies nous avons gravés les mots de liberté, d'égalité, de fraternité, mais bon c'est ainsi le rural il vaut la moitié d'une banque, alors qu'elle a déjà fait, a été créée au début des années 70 ans se comprenez ça je comprenais pas ce que c'était quoi, la commune rurale, un peu de charbon pour le poids à boucher les trous dans la rue et ma foi, à quelque chose près, quelques pour le tableau et quelques papiers c'était ça aujourd'hui, les besoins des habitants des communes rurales, ils ont rejoint les habitants des communes de la ville, moi j'ai été élu en 1983 si j'avais dit à mon congé municipale, vous voyez, dans quelques années on va faire une cantine scolaire, ils m'auraient ri au nez si je leur avais dit dans quelques années, on ne va ouvrir une crèche, ils auraient appelé aussitôt l'hôpital psychiatrique pour me faire interdit et pourtant c'est ce qui s'est passé le rural et le rural n'est plus une communauté où on vivait, où les enfants aller manger chez la grand-mère à midi parce que le rural a pris des habitudes du monde urbaine et il faut en prendre en compte parce que les communes rurales ont quasiment aujourd'hui les mêmes besoins que les communes urbaines, Madame la Ministre. Merci madame la présidente, madame la ministre, la la succession d'amendements que nous discutons depuis ce ce matin, vise à réduire les inégalités, à corriger les effets négatifs et les dommages collatéraux des réformes successives qui ont eu lieu et et montre une chose, c'est que le système est à bout de souffle. Le système ne fonctionne plus et c'est la raison pour laquelle les uns et les autres nous déposons un certain nombre d'amendements pour en corriger telle ou telle effets négatifs, c'est ce qui est fait au travers de cet amendement que nous allons voter, mais de grâce Madame la ministre, vous venez d'arriver, il faut vous laisse un peu de temps mais prenez l'engagement de mettre à plat l'ensemble du dispositif repartant d'une feuille blanche et essayons de construire quelque chose, prenons le temps de le faire, rassemblons l'ensemble des forces politiques et l'ensemble des associations d'élus, il y aura nécessairement des heureux et des mécontents, assumons-le, mais en tout état de cause, il faut aller vers plus de lisibilité, vers plus d'équilibre vers plus d'égalité et il faut aussi au regard de ce que nous avons connu ces dernières années, prendre en considération la situation de la vie de nos concitoyens dans les communes rurales et ces communes rurales aujourd'hui souffrent plus que les autres, il faut donc effectivement mettre sur la table et dispositions et les dispositifs qui permettent de les aider et d'assurer à nos concitoyens ruraux des qualité de vie qui soit à la hauteur de ce qu'ils attendent.

certains de mes collègues que depuis presque un quart de siècle, que je me préoccupe de fiscalité locale certaines réalités ne ne m'échappe pas, cependant, je voudrais dire que

l'obsolescence de critère de de qui multiplie par 2 les, les, les ressources pour les les collectivités les plus peuplées et puis bon, au fil du temps, on s'est aperçu que cette fiscalité qui était assise sur des réalités, il y a environ un demi siècle, hé ben ont évolué, ce ne sont plus forcément les mêmes, et lorsque tout à l'heure vous discutiez du de la longueur de voirie je partageais aussi de que vous disiez parce que je suis à rural aussi et je connais bien les choses simplement, dans la la charge agrégé du territoire où j'étais il y a 40 ans quand j'ai commencé à m'occuper des choses, la voirie, c'était 50 % de la dépense aujourd'hui c'est quinze quand tout va bien, donc, les choses ont évolué et on ne peut pas garder des symboles asseoir les choses de cette manière-là sans arrêt simplement et ce que je voudrais vous dire, c'est dans le le temps qui s'est écoulé, j'ai moi aussi participer à des tentatives de réformes, je me souviens d'une il y a 2 ou 3 ans, qui ont vu combien c'était et on a vu dans. Dans ce ce même hémicycle des gens partout parce que chacun a regardé sa dotation historique. Et tout s'est fixé sur la base de la dotation historique ont procédé et non pas sur la dotation qu'il faudrait, je suis pour une remise à plat complète de la fiscalité locale et sur d'autres critères, notamment sur celle de 2 critères de de de charges synthétique pour les territoires afin qu'il soit doté sur ces bases là au titre d'une péréquation généralisée et que par ailleurs on puisse satisfaire les dynamiques dans les autres territoires et c'est à cela qu'il faut qu'on arrive, mais y êtes-vous prêt, j'ai pas le sentiment, on y est prêt intellectuellement, mais dès que les résultats sortent on on en veut plus, alors il y a un problème, même si on a dit qu'on prendrait un tunnel, d'où une un lissage sur 5 ou 10 ans, mais c'est ce qu'il faut faire et il faudra le faire alors voilà, bon à partir de là, c'est la réponse que je voulais apporter sur ma mes considérations personnelles, ceci étant, je suis au bord de la commission des finances, et j'essaie de de remplir modestement mon mon rôle et c'est pour ça que je vous ai demandé un retrait en l'état actuel des choses, monsieur le rapporteur, je vais donc mettre aux voix l'amendement 152 rectifié, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté. Après l'article 45 16 amendements qui font l'objet d'une discussion commune et nous commençons avec le 140 ah pardon, une parole. Merci madame la présidente, alors nous rentrons sur un nouveau sujet nous allons maintenant examiner plusieurs amendements et sous-amendements relatifs à la DGF des communes nouvelles, c'est un autre sujet, mais qui concerne beaucoup moins de communes en réalité donc, nous partageons tous la volonté des auteurs de soutenir le développement des communes nouvelles hein, mobilisant pour ce faire et leviers juridiques et financiers adéquats, la loi prévoit déjà un certain nombre de dispositifs d'incitation financière, avec notamment la dotation d'amorçage ou encore le pacte de stabilité pour les 3 premières années suivant la création, on peut également citer les dispositifs d'éligibilité dérogatoire à la DSR ou la DPE elle introduit respectivement 2022, et dans le texte du présent PLF, faut-il aller plus loin, comme le pense évidemment certains un collègues pour encourager davantage le mouvement et peut-on faire mieux, alors, comme toujours, en politique, et tout ce qu'on peut toujours faire mieux, néanmoins les pistes proposées par les différents amendements ne nous paraissent pas encore abouti et se heurte notamment à des obstacles d'ordre technique ou juridique, ces amendements ont en commun de prévoir que certaines dotations versées à la commune nouvelle qu'il s'agisse de la dotation forfaitaire ou de la DSR, soit au moins égale à la somme de ces mêmes dotations qui aurait dû être versé aux anciennes communes la Ministre nous confirmera, mais il semble techniquement impossible de reconstituer ainsi de telle dotation fictive pur pour des communes qui ont cessé d'exister juridiquement de telle sorte que ces amendements apparaissent en réalité inopérant mais je laisserai la Ministre développer sur ce point, puisque c'est là, il y a une partie administrative là-dessus, ça me paraît assez clair, si les communes n'existe plus, il n'y a plus de documents, s'il y a plus de documents, c'est on ne peut plus retrouver la somme de des communes qui n'existe plus, ces amendements prévoient en outre un nouveau mécanisme de garantie d'évolution de leur DSR qui serait indexée sur celle du montant national de la dotation, une telle mesure poserait de très sérieux problèmes d'équité vis-à-vis des autres communes et pourrait même s'exposer, selon nous, à une censure du Conseil constitutionnel sur ce fondement les communes nouvelles deviendraient en effet les seules communes pour qui l'évolution de leurs dotations de péréquation serait complètement décorrélé de celle de leurs indicateurs financiers alors après très sincèrement cette assemblée, nous apprend à modifier nos points de vue. Bon, puisqu'elle vient de de voter une garantie de non-baisse de la dotation d'intercommunalité. à ma grande surprise, mais c'est pas grave, donc si elle vient de le faire, c'est-à-dire d'avoir une vision totalement décorrélés de tout après tout on peut continuer pour les communes nouvelles voilà on peut poursuivre sa cette même voie mais on ne peut pas vous dire à la commission des finances que nous sommes évidemment défavorable, non pas à l'idée, c'est-à-dire non pas à l'idée qu'il faille continuer à trouver des systèmes pour créer des communes nouvelles c'est sûr qu'il y a un enjeu autour de autour de ça, même s'il n'est pas toujours très partagées, hein, ce qu'elle a comme une nouvelle, quelque fois ne rassure pas on va dire, mais pour ma part et pour la part de la Commission plutôt ouvert, simplement il faut trouver le système qui va bien et donc peut être le préparer, je, je le dis à ceux qui ont écrit, demandes de morts et et je parmi les gens qui ont écrit à Françoise Gatel, c'est à dire la présidente de la de la commission donc de la délégation aux collectivités, donc qui c'est, je pense, se rapprocher quand il le faut, des des cabinets et d'DGCL pour trouver les termes exacts qui permettront de faire passer telle que ces amendements sont rédigées en tout cas, ils sont d'une part, inopérant, d'autre part, dangereux par rapport à une censure du Conseil constitutionnel et donc très naturellement j'appellerai à leur retrait, mais j'ai bien compris que la tendance au retrait est assez peu développé aujourd'hui. aujourd'hui. Le rapporteur, madame la ministre, vous avez la parole. Merci madame la présidente, oui, je vous ai demandé la parole parce que plusieurs amendements proposent d'inciter au au développement des communes nouvelles et je voulais vous dire à quel point le gouvernement et pour. pas les 16 amendements, mais nous avons 16 amendements et je voulais vous dire parmi lesquels et pour être en totale cohérence et je le redis pour Monsieur malheureusement, Monsieur le Sénateur, est parti quand je me permets de dire défavorable en cohérence avec la commission des finances, et pour ne pas vous infliger exactement les mêmes arguments, donc c'est pour ça que je me permets de temps en temps et pour aller vite, de vous de d'arrêt et d'aller à la conclusion, quand le gouvernement est en phase avec les recommandations de la commission Un dispositif de maintien parmi ces 16 amendements de maintien de la dotation globale de fonctionnement des communes nouvelles à hauteur des montants perçus en 2000 22 et au niveau de la somme des DGF des communes déléguées dont elles sont issues, sur le plan technique, comme ça vient d'être dit, je le confirme, cette mesure n'est pas applicable, vous l'appuyer sur des communes disparu car fusionner, or les les nombreux indicateurs utilisés pour répartir à DGF de façon juste et objective n'existe plus sur le périmètre des communes fusionnées qui n'existe plus juridiquement géographiquement institutionnellement institutionnellement et fiscalement, donc le dispositif serait donc totalement et irrémédiablement inapplicable le calcul des dotations ne pourrait tout simplement pas être effectués sur le principe, je ne suis pas favorable à tous ces dispositifs car il viendrait modifier en profondeur le pacte de stabilité dont bénéficient les communes nouvelles ce dispositif complet et très incitatif a été réformé récemment, en 2020 et se traduit concrètement par les mesures suivantes pour les communes nouvelles, je me permets d'être longue, je ne parlerai qu'une seule fois pour les 16 amendements, elle perd elles perçoivent une garantie spécifique visant à neutraliser une baisse de leurs dotations forfaitaires et de leurs dotations de péréquation suite à leur fusion, deuxièmement, elles perçoivent une dotation d'amorçage de six euros par habitant perçus pendant 3 ans, pouvant atteindre 10 euros par habitant pour les petites communes, troisièmement, elles pourront bénéficier en 2023 d'une éligibilité dérogatoire à la DSR la DSR lorsqu'elle dépasse les 10000 habitants, mais peuvent être qualifiés de rural, les communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes d'un ou plusieurs EPCI bénéficier en outre des anciennes dotations de l'EPCI en conséquence les 787 communes disposant du statut de commune nouvelle bénéficier en 2022 d'une attribution moyenne de DGF s'élevant à 219 65 euros par habitant, contre 165 euros par habitant pour l'ensemble des communes, soit 32 % de plus vous proposez notamment de remettre en cause le principe d'éligibilité dérogatoire à la DEA DSR introduit par la loi de finances 2022, ce dispositif permet de soutenir les communes nouvelles gardant des caractéristiques rural. Enfin, votre amendement court un fort risque de censure par le Conseil constitutionnel, en instaurant de manière pérenne, une différence de traitement entre les communes nouvelles et l'ensemble des autres communes, il en va de même entre les communes nouvelles votre amendement favorisant celles ayant maintenu des communes déléguées au détriment de communes plus intégrée, les pistes, comme cela a été dit, ne nous semble pas assez abouti assez abouti, pardon pour les mêmes raisons que monsieur le rapporteur, l'indiquer, je veux souligner l'importance que je porte, que le gouvernement porte.

recevoir au ministère pour monter un groupe de travail pour en discuter et pour voir comment nous allons pouvoir ensemble développer nos communes nouvelles, je vous remercie. Merci madame la ministre, alors nous allons pouvoir procéder à la. Présentation des amendements, à commencer par Monsieur Vial. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est un peu original de présenter des amendements après qu'il ait après la vie du du gouvernement et de la Commission, mais je, je m'y essayer.

des lapins dans des sacs, on a, on a vendu aux communes nouvelles une une organisation et il y a une variante avec le chat, mais ces chinois il y a, on a vendu aux comme une nouvelle, un certain nombre de, de, de dispositions

elles perdent des dotations à perte de la DGF elles perdent des subventions auprès de de tous les financeurs et aujourd'hui on se demande pourquoi, et la Cour des comptes viendront rapport et explique

c'est quelque chose qui se base sur des choses qui existent, donc je vais répondre un peu à, à votre proposition vous propose 3 choses notamment premièrement de stabiliser la la la la DGF afin de garantir aux communes nouvelle qu'elle n'ait pas de perte de DGF, c'est la moindre des choses si on veut que des communes nouvelles se créent, et on s'appuie sur les communes nouvelles qui ont des communes délégué ça existe juridiquement comme une déléguée et donc on on peut geler sur cette base là, deuxièmement pour les les communes qui ont déjà fusionné, on s'appuie sur le montant de 1022, c'est un chiffre qui existe la DGF 2001 2 on la gèle, c'est une garantie, simple et le il y a un 3ème point dans cet amendement, qui permettent de garantir la la le versement de la dotation de compensation de de l'EPCI pour les communes, communautés voilà je vous remercie, mais vous voyez, on s'appuie sur des choses qui existent pour favoriser, c'est comme une nouvelle, comme vous le souhaitez, madame la ministre, et nous aussi. Messieurs Corbizet. Oui, pardon madame la présidente, madame la Ministre, la cause sera tellement bien défendu par la présidente Gatel que mon amendement est défendu. Il me suis Corvisier Madame Keitel. Comme la présidente, madame, je remercie mon collègue pour la pression, je voudrais remercier le collègue Cédric Vial qui a bien défendu le principe alors Madame la Ministre, vous m'épatez totalement parce que vous êtes totalement pour, mais au final, vous êtes gravement contre mais vous nous proposez gentiment d'aller prendre le thé discuter comme une nouvelle chez vous, alors c'est sympa mais excusez-moi, on ne fait pas une loi de finances avec ça, quant au président Reynal, moi je suis très touché de la tension qu'prennent mais sérieusement, cher Claude, mais à la fin, à force de nous dire : ben oui, mais votre truc, il est pas opérant, moi je regrette, c'est très opérants parce qu'il a déjà opéré, je veux dire pourquoi à à l'Assemblée nationale, ils ont adopté un amendement maintenant la dotation élu local pour les comme une nouvelle à partir de celle perçue par les communes déléguées alors moi, il faut qu'on m'explique pourquoi ce qui a été opérant à l'Assemblée nationale ne l'ait pas au Sénat et puis je dirais quand il y a une volonté, il y a un chemin et soyons sérieux. Non mais ah bah tout le monde est d'accord avec moi, voilà, formidable, ça m'arrive rarement, et je termine, et je termine non mais Madame la Ministre est-ce qu'on peut être grave et sérieux et en même temps je crois qu'on l'a tous, c'était en 2014 80 communes françaises n'ont pas eu de candidats aux élections municipales en 2020, c'est cent dix hé bien, continuons à emprunter ce chemin, et on verra, on n'aura plus à parler d'argent parce qu'il y aura plus d'élus, il y aura plus de communes et ce sera le désert et on aura une grave misère sociale et moi je souhaite vraiment que les communes nouvelles reste une liberté d'initiative, donner aux élus, il ne s'agit pas de l'imposer mais quand il y a des élus courageux et audacieux qui se payent des moments très difficiles pour garantir l'avenir de leur collectivité est-ce qu'on les aide ou est-ce qu'on les enfonce. Alors, le 434 terre c'est un peu une évolution, enfin moi je dis qu'il y a toujours ce vice caché dont Cédric Vial a parlé qui n'avait pas été vu et pas été dit à propos de la DSR, du fait d'évolution législative et. Sincèrement, chers amis, est ce qu'on peut comparer une commune de 2000 habitants historiquement de 2 1000 habitants avec 6 communes qui se sont regroupées pour faire 2000 habitants, donc ce que nous ce que nous proposons aujourd'hui c'est que les comme une nouvelle ronde dans des dispositions de droit commun, sans les sanctionner, il s'agit là, pour les communes nouvelles qui serait créée à partir de 2023, de bénéficier d'un mécanisme de sortie sur 4 ans de la dotation de solidarité rurale et le sifflet ainsi proposé est extrêmement responsable et on retrouve de l'incitation.

la somme des cosignataires est supérieur à la majorité, dont le Sénat a besoin pour adopter cet amendement donc le sud, le suspense est relativement limité si par, par contre, j'aimerais bien quand même, Monsieur le Président, parce que vous avez tout à l'heure pris la parole pour donner votre avis sur les amendements, avant qu'ils ne soient défendus et vous avez donné un avis défavorable, l'ensemble des amendements, il me semblait avoir vu un avis de sagesse, d'accord, donc on aimerait quand même avoir votre avis sur les différents amendements qui qui pourrait peut-être, être différenciées et notamment sur celui-ci qui qui permet de régler là aussi un vice caché, comme l'a dit Madame Gatel, sur un nombre relativement restreint de de communes nouvelles, mais on ne pourra pas, on ne à avoir des communes nouvelles, on ne pourra pas inciter à la création de comme une nouvelle si on n'est pas capable de corriger ce ce genre de règles et en plus c'est une peine qui vient, qui tombe sur ces communes par des modifications législatives qui sont intervenus après qu'elles aient pris la décision de, de, de, se créant comme une nouvelle, nous nous devons, en tant que représentation nationale de régler ce type de problème pour redonner confiance finalement aux élus locaux dans la politique du gouvernement dans le et dans la représentation nationale quand il s'engage dans un dispositif on doit au minimum tenir les engagements qu'on leur a donné quand on les inciter à y rentrer. l'amendement a été défendu par la présidente Gatel et par notre collègue Vial et je défends celui que j'ai déposé effectivement avec mon mes mon collègue Franck Menonville et et l'ensemble des indépendants. Il s'agit pas pour répondre à la à la critique, qui a déjà été faite par le président rénale d'inciter à la fusion ou de donner un cadeau aux comme une nouvelle, il s'agit de réparer une injustice, ou, pour reprendre l'image que je ne connaissais pas du sac de de réparer un truc qu'on avait pas vu et il se trouve qu'il y a des communes nouvelles qui se voit non seulement pas inciter mais mais qui touchent une DSR inférieur à ce qu'il touche la quantité quand ils étaient les communes des délégués enfin les unes à côté des autres, donc je crois qu'on peut tous se quand même considérer ici que on ne va pas donner une DS est inférieur à des communes nouvelles, simplement parce qu'elles ont fusionné, alors même que c'était quand même pas l'objectif et que c'est plutôt à mon sens, si elle le souhaite, positif, de travailler ensemble, donc il s'agit de réparer modestement une injustice, un truc qui n'avait pas été vu et, là, l'amendement est très modeste, puisqu'il prouve, il prévoit non pas de la réparer définitivement de non pas de façon pérenne mais de sortir de façon lissée sur 4 enfin en sifflet de cette injustice, donc c'est très modérée, comme un moment.

il convient de réfléchir aux raisons pour lesquelles de nouvelles communes ne souhaite pas s'y engager le mécanisme des communes nouvelles a été initiée il y a déjà quelques temps, une dizaine d'années, j'appartiens à un département qui est pilote en la circonstance en la circonstance, il s'agit du département de Maine-et-Loire et beaucoup de fusions de communes on était ont été opéré sur la base du volontariat, avec un projet de territoire, ce sont celles qui fonctionnent le mien à l'heure actuelle, un certain nombre de communes envisage parfois de défusionner mais c'est c'est dès lors qu'il n'y avait pas de projets de territoire et donc votre proposition de commission tombe à pic, je crois que c'est le moment de faire un arrêt sur image de regarder un petit peu ce qu'il en est sur cette question du comme une nouvelle parce qu'il y a un certain il y en a un certain nombres qui qui fonctionne correctement, d'autres qui ont des difficultés, c'est le : c'est le sens de cet amendement. Merci Monsieur Bigot le 694 madame Cukierman. Oui merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Je je crois que les arguments qui ont été exposés tout d'abord sont importants parce qu'au moment de voter ces dispositions, il nous appartient effectivement. Tout d'abord avec humilité parfois de pouvoir se dire qu'il y a eu quelques erreurs et que nous avons comme seul objectif de continuer de garantir l'égalité entre les différents dispositifs et donc de gommer comme ça a été dit par Madame Gatel par Monsieur Vial les différents vices qui pourraient aujourd'hui subit ce subsister dans les différents dispositifs, la question n'est pas de revenir sur le débat autour des communes nouvelles, nous l'avons eu et dans le temps imparti, je ne pourrai en faire de de résumé. Pour notre groupe, l'enjeu n'est pas d'inciter ou de des inciter l'enjeu est tout simplement de partir d'un conseil d'une réalité : aujourd'hui les communes nouvelles existe et, parfois, et on va se le dire tranquillement parce que ici, ce n'est pas le paradis sur terre, elles existent, parce que, on les a. Inciter fortement conseillé fortement encouragé, on leur a fait découvrir que tous ensemble, c'était mieux pour garder telle ou telle service public et que comme par. La magie soudainement tous les élus étaient tous d'accord pour créer ensemble une commune nouvelle et qui l'ont créée, tout va très bien, mais à part ça, madame la marquise, il faut quand même que je vous dise. Que cela pose encore des soucis aujourd'hui et que donc venir fragiliser ce qui s'est constitué, volontairement, volontairement, et je ne réouvre vraiment pas le débat ici, nous l'avons eu de longues heures précédemment seraient en tout cas remettre en cause le rapport et la confiance que peuvent avoir les élus y compris dans l'accompagnement que l'État leur fait au quotidien pour le déploiement. De la mise en place de ces communes nouvelles dans notre dans mon département, il en existe un certain nombre de je crois qu'aujourd'hui la question est de sécuriser cette existant plutôt que le fragilisant. Le fragiliser, d'où le sens de notre amendement et Madame comme j'ai débordé, j'en profite pour dire que le prochain amendement sera également défendu et au lieu de 4 minutes, j'aurais fait deux minutes 10 pour les deux. remercie, cher collègue Monsieur kaput, le 580. Alors, si vous m'y autorisez, je vais défendent le 580 est le suivant, c'est-à-dire le le 300 de rectifier en même temps et ce d'autant plus qu'en fait le 580 et le repli du 300 de donc je pense que la la séance, les amis, dans, dans, dans le désordre en pensant sans doute que le le le premier était le repli de celui d'avant, mais en fait c'est le le repli du dernier on est sur la même logique et ce ce ce Vous le verrez, a été déposée par les quatres sénateur du Maine-et-Loire, parce qu'il. Démarre par une problématique du Maine-et-Loire, de la commune de Douai en Anjou doué en Anjou : c'est une, c'est une commune qui, à l'origine était composé de Doué-la-Fontaine 7000 habitants et des communes environnantes, qui sont toutes de moins de deux elles fusionnent, elles arrivent à une commune de 11000 habitants, comme toutes les autres communes, elle pense qu'elles vont garder une DSR du même niveau et là elles découvrent cette année qu'vont perdre 800000 euros de DSR parce que. Du jour au lendemain, pour une raison très simple, parce qu'on leur dit que la densité de leur population de la commune centre parce qu'elle fait 7000 habitants est trop dense. On est à Douai en Anjou, enfin faut je vous invite à y aller, on est vraiment dans la ruralité du sommet roi, donc on est, on a des critères de densité qui sont vraiment à apprécier de façon très particulière, c'est la raison pour laquelle le premier amendement, c'est-à-dire le 302 qui est deuxième, en fait, la propose et qui a été déposée par mes collègues Bigot et noirs et de roches propose simplement de rajouter aux critères de pour le maintien de la DSR de très peu dense et on aura ajoutant ou de densité intermédiaire puisqu'il semble, on semble considérer que ce type de communes à une densité qui est intermédiaire et non pas très peu dense, et le deuxième est un amendement de repli qui, si jamais on maintenait une sortie progressive en 5 ans.

vous n'ignorez pas néanmoins que le fait pour certaines communes de se regrouper en commune en comme une nouvelle ne leur a pas fait perdent leur caractère rural et c'est le cas dans un certain nombre de communes du Maine-et-Loire, vous voyez que ce département est particulièrement mis à l'honneur dans les discussions de ce jour, comme à chaque fois que nous évoquons les une nouvelle. Et donc, lorsque nous avons voté lors du précédent loi de fil à la précédente loi de finances 2022, de permettre à certaines communes qui dépasse les 10000 habitants de continuer à bénéficier de la DSR, nous avions bordée ça accompagné ça d'un certain seuil sur la densité de population cette densité devait être dense ou très peu dense, très peu dense, nous vous proposons un aménagement pour prolonger, en fait, ce le bon sens qui a conduit nos débats de de l'époque en disant il y reste, certaines communes il y a des effets de bord en fait sur cette sur cette mesure et nous vous proposons d'étendre ça a une densité, un tout petit peu plus fort forte, c'est-à-dire très peu dense ou de densité intermédiaire, ce qui permettrait d'intégrer certaines communes, la commune de en Anjou bien sûr dans le Maine-et-Loire, mais probablement d'autres communes en France qui seraient concernés, je vous remercie. Merci, cher collègue, et maintenant le 400 4. Chez Bicou oui, c'est le 3ème, sénateur du Maine-et-Loire à intervenir pour le sujet, pour les mêmes motifs, et comme ça a été brillamment défendu avant, je ne m'éterniser pas sur le sujet en reprenant ce qu'ils ont dit et que je partage complètement. Merci le 142 rectifié bis monsieur Vialat. de répondre à des effets de bord qui ont été créés par par cette réforme, toujours sur les communes nouvelles en effet un certain nombre de de communes nouvelles qui dépasse le le seuil de de 10000 habitants deviennent inéligibles à à la DSR, ça représentait environ 32 communes nouvelles.

de solidarité urbaine, donc là à la DSU lorsque ceci a été fait il y a pas eu de simulation qui ont été faites, elles ont été faites depuis, notamment le par le l'association des des maires de France et on s'aperçoit en fait que voulant aider un certain nombre de communes, on les enfonce encore un petit peu plus parce qu'on on leur fait perdre la DSU, qui étaient souvent bien plus importante que la DSR qu'on leur accorde, en contrepartie, donc là encore c'est c'est une peine supplémentaire qu'on met sur le dos de ces communes sur les 32 qui étaient concernés jusqu'à présent, ça concerne à peu près 13 communes nouvelles, donc vous allez dire c'est c'est pas énorme, mais là encore, c'est la promesse qu'on fait à ces communes, on leur met encore une charge supplémentaire sur le dos, donc il semblerait nécessaire de revenir sur cette situation et de permettre à ces communes notamment de continuer à percevoir la DSU pendant un temps limité, si vous voulez, et si vous maintenez votre invitation au ministère, Madame la Ministre, vous nous direz : d'abord ce qu'on mange et ensuite on pourra mettre au menu ce ce genre de pour discuter précisément de la manière dont on pourra faire sortir ces communes dignement de ce dispositif. Je vous remercie, Madame la présidente, je vais être très rapide, on a donc un, un problème de glissements parfois pour certaines Interco, qui sont plus éligibles en DSR qui pourraient être léger bander assumer, on n'est pas sûr de tout ça, donc il y a 13 comme une nouvelle qui redeviendrait éligibles à la DSR en 2023 mais perdront leur et j'y militer à la DSU voilà, ces nouvelles dispositions que vous proposez aggrave leur situation, compte tenu du risque cette proposition fait prendre nos comme une nouvelle concernés nous proposons par cet amendement de conserver la perception de la DSU pour c'est comme une nouvelle dans l'attente des premiers résultats sur la DSR de ces communes nouvelles en 2023, c'est la mise en application de l'histoire du chat dans le sac. Merci, et enfin le 585. Non mais comme comme déjà dit monsieur Madame Gatel ont tout dit et donc je me range à leurs explications que je partage il faut pris jusqu'au menu, Madame la Ministre. Merci madame Luc Hermann alors ben maintenant, nous pouvons passer aux avis sur ce l'ensemble de ces amendements. Alors là, je ne vais pas donner un avis, par amendement, puisque on a fait une une présentation commune au départ et cette présentation commune, je pensais que c'était compris dans mon propos vos demandes de retrait pour tous les amendements et j'ai même fini d'ailleurs en disant que j'avais,

évidemment ça ne rien dans vos interventions ne répond au au fait que ces amendements ne peuvent pas être mises en oeuvre, bon petit souci au problème constitutionnel évident il y a pas de souci non plus c'est pas on fait comme si on avait pas vu il y a pas de souci, mais, mais, en même temps je vous dis que malheureusement ça va s'appliquer comme ça, donc le sujet important c'est comment, effectivement, on est capable, un jour ensemble de rédiger un texte qui fonctionne est-ce qu'on en est capable, voilà, c'est ça notre sujet tout le reste, ce sera votée il y a pas de souci, il y a pas d'inquiétude, mais sera inopérant, après avoir fait notre débat, ce qui reste important, c'est que nous sommes tous attachés à trouver des solutions pose les communes nouvelles, ça, ça reste vrai et ça doit rester l'aspect positif et utile de notre débat, quel que soit le vote, par ailleurs, bon et j'ai beaucoup aimé Cédric Vial l'argument : le gouvernement ne nous a pas fourni de simulation, j'attends les vôtres sur tous les amendements là son vote, je ne suis pas tout à fait certain que tous nos amendements, fasse l'objet de simulation, mais bon, mais je trouve amusant de pour, une fois de l'utiliser dans l'autre sens, je l'avais jamais tenté mais vous savez, c'est des perspectives, enfin je crois qu'il faut. Il ne faut pas trop user Madame Cukierman, chers collègues, à mon avis, alors vous allez me dire que c'est parce que vous avez dit : ah, je vous connais, mais quand même, vous l'avez dit qu'il aurait des maires

de manière générale, moi je connais ce débat des communes nouvelles dans mon département, j'en ai été figurez vous vous en doutez, sans doute un peu promoteur comme ici d'ailleurs, j'ai un succès limité voilà, c'est-à-dire que les communes, vous voyez par exemple 5 communes au hasard de 10, 15, 20 habitants et cetera où tous les maires, m'ont dit qu'ils étaient intéressés ben après avoir interrogé le 15 habitants, ils ont dû ben on garde notre mairie notre cimetière notre truc, on fait rien,

de ce que certains découvrent n'était inconnu au départ rien, donc il y a, il y a des il y a des avantages et des inconvénients, comme dans tout, tout groupement to truc il y a des avantages, il y a des inconvénients, c'est la même chose et donc en tout état de cause, ces amendements. Vous allez les voter et le point important ce qu'on va se retrouver après pour trouver des amendements qui tourne et on essaiera de le faire, merci. Y'monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, vous dire bon, je n'ai pas été comprise par Françoise Gatel ce n'est pas grave on se retrouvera malgré tout pour travailler, j'ai beaucoup apprécié les prises de parole qui visait à accepter de travailler ensemble, ce que je veux dire en résumé très court : anticonstitutionnalité, vous pouvez ne pas être d'accord, moi j'arrive et on reçoit vos amendements vendredi 11 heures moi j'arrive dans ce midi. je travaille hier pour préparer cette séance des services me dire c'est anticonstitutionnel, bien sûr que, ils peuvent se tromper, mais en attendant, moi je vous dis que je fais confiance et que quand on me dit : anticonstitutionnalité oh quand on me dit madame la sénatrice inopérant et quand on me dit aussi du pacte de de stabilité aussi auxquelles on est attaché, certains de ces amendements ne sont pas opportun, moi, je viens vous dire en introduction et en motivant la position du gouvernement pour lequel voilà c'est c'est 3,3 raisons qui font que je pensais que l'on pouvait travailler ensemble mais je continue en conclusion à vous dire, et là je n'ai pas été comprise, donc je le redis à quel point le gouvernement soutient les communes nouvelles mais écoutez, madame la sénatrice, est ce que ça peut passer par des amendements de soutenir. Soutenir ne veut pas dire que on est d'accord pour les raisons que je viens d'invoquer, j'ai pas les reciter qu'on est d'accord avec ces, ces amendements donc ce que je vous propose, c'est de mettre en oeuvre ce soutien efficacement par un travail comme ça a été dit par monsieur le rapporteur ensemble et dès la semaine prochaine et ça pourrait être poursuivi si on travaille bien, pendant 2 heures par un déjeuner merci beaucoup. Merci madame la présidente, madame la mise bon juste hein. Très sincèrement, d'abord, bon effectivement, je m'en excuse, on n'a pas à se prendre à partie, comme je l'ai fait tout à l'heure peut-être, monsieur le président de la commission des finances, simplement, chacun a son caractère, chacun a son mot, donc on peut tous se se jouer des choses sur ce qu'il faudrait dire et dans quels termes je crois que, par contre, nous pourrons une nous pourrions nous retrouver l'un et l'autre sur le fait que, par exemple, une fois que les communes nouvelles ont été créées par la législation, nous pourrions constater l'un et l'autre que l'accompagnement indispensable qu'aurait dû être celui par exemple des services de l'État, qui aurait dû être celui de la DGFIP, aux côtés de ces différents élus, y compris pour les accompagner en matière de prospective financière et de projection de ce à quoi ils auraient vu étant parfois lacunaires je n'oserais dire absente madame la Ministre parce que, là encore, on me dirait que je suis dans l'excès, donc, en tout cas, lacunaires a fait parfois que, aujourd'hui, un certain nombre d'élus ont pris des décisions en lien ou pas, avec leur population certaines parfois en lien avec leur population qui font que nous sommes dans des difficultés qui amène effectivement les différents amendements être déposée parce que, in fine, et dans la réalité dans dans la vraie vie, je m'excuse de cette expression, qui n'est peut-être pas très érudit pour cet hémicycle mais en tout cas dans la vraie vie, tout, tout n'a pas été maîtrisée, tout n'a pas été mesuré qu'aujourd'hui nous avons des élus qui sont constatés à ses choix, madame la ministre. Très simplement. On vous a entendu je crois que. J'aimerais pas être personnellement à votre place effectivement en 2 jours, reprendre un hein la mission collectivités territoriales. C'est un défi, voudrais vous dire mais vous avez tout ce qu'on va dire que ça avec beaucoup d'excès, vous savez la constitutionnalisation là le rapport à la caution été de tels amendements du pacte de stabilité. Sachez, des fois vous en démarquer nous sommes ici pour faire de la politique et laissons à d'autres le soin d'arbitrer, en tout cas, sachant travailler plus de 2 heures, s'il le faut et nous sans chantage, nous passerons tous un bon moment dans l'intérêt de nos collègues, collectivités. Si cher collègue, nous avons une demande de parole de d'abord Madame Goulet ensuite monsieur kaput et monsieur de oui, madame la présidente, madame la ministre, vous avez, vous nous avez dit tout l'intérêt que vous portiez au travail collectif, alors c'est peut-être un détail pour vous mais pour nous ça veut dire beaucoup est-ce que vous pourriez travailler à voir avec vos services le nombre de grands électeurs des communes nouvelles en France parce que nos préfets ont beaucoup de difficultés à connaître d'ores et déjà, le nombre de grands électeurs et voyez-vous, c'est un sujet qui nous intéresse, donc ça fait pas partie d'un amendement et comme je vous l'ai dit, c'est peut-être un détail pour vous mais pour nous ça veut dire beaucoup. Merci, cher collègue. Alors Monsieur capuche. Merci madame la présidente, non, juste 3 mots la première évidemment pour remercier la ministre pour son invitation à travailler ensemble et nous serons bien évidemment présent, le 2ème, le 2ème mot effectivement alors, il faut faire attention quand on a des des amendements comme ça qui viennent de tous les bancs, c'est quand même qu'il y a un bon sens du Sénat qui représente ce bon sens des élus locaux

on n'est pas tous des constitutionnalistes ici et je ne sais pas si tous les amendements sont conformes à la constitution, je l'espère, je le pense, il y en a un sur lequel je peux on peut tout soumettre d'accord, c'est le 380 que j'ai déposé, celui qui a été déposée par mes deux collègues, il s'agit juste dense à la densité peu dense, très peu dense ou de densité intermédiaire, donc ça concerne toutes les communes de France, il y a aucune différenciation pérenne entre les comme une nouvelle et les autres, donc celui-ci sans être constitutionnaliste, je peux vous affirmer de façon certaine qu'il est parfaitement conforme à la Constitution, donc celui-là, mes chers con, vos collègues, j'ai il y aura pas de problème, il y a pas de problème sur les autres et celui-là encore moins. Ce qui a pu Monsieur Delage. Merci madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, moi, je voudrais vous faire part de ma perplexité sur ce débat depuis 2 heures parce que tout à l'heure, on a eu un débat très intéressant sur la DGF, on est tous d'accord pour dire que ça fonctionne pas mais quand par hasard, on fait bouger un curseur l'année d'après, on revient en se disant, la, la, mon Dieu, il y en a qui ont perdu, on n'entend jamais ceux qui ont gagné, où tout le monde serait gagnant alors que l'enveloppe et constante, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de de le reconnaître et là je je suis frappé sur sur ce débat que que nous avons où on veut corriger les effets que nous n'avions pas vu d'un vote sans doute un peu précipité sur les communes nouvelles, c'était génial, les communes nouvelles, on allait ensemble, on avait plus fort, c'est comme les EPCI sauf qu'à la sortie, quand il y a pas plus de sous, il y a toujours le même nombre de kilomètres de route il y a toujours le même nombre d'élèves, donc je ne sais pas comment une réforme de structure peut multiplier les sous, alors je voudrais former un voeu, Madame la Ministre, vous nous invitez tout ça déjeuner, moi ce que je souhaite, c'est que l'année prochaine on ne se disent pas la même chose que l'année dernière, parce que l'année dernière on s'est quittés sur ce débat en disant, promis juré, on va travailler pendant l'année qui vient, et l'année prochaine, lors du vote du budget, nous trouverons une voie de passage, je constate que nous ne l'avons pas cette fois-ci, pour ma part, j'ai signé aucun amendement et je n'en très aucun tant que nous n'auront pas été capables, ensemble, de se dire que faire une réforme, c'est accepter tout mettre sur la table, accepter qu'il y ait des perdants, accepter que des gagnants, mais la réforme il y a que des gagnants, je n'y crois pas. Très rapidement, madame la présidente, madame la ministre nous on prendra les 2 comme le fromage et le dessert, c'est-à-dire on prend les amendements et l'invitation. Travailler, je vous en remercie, mais le fait que, sur tous les bancs oh portes cela ça a du sens, monsieur le président de la commission évident avec amitié et respect, je partage tout ce que vous dites et je suis sensible à votre proposition pourra même se rapprocher de vous pour travailler l'anticonstitutionnalité, alors moi j'ai une confiance éperdue dans le DG, celle qui est là et ça me donne l'occasion de lui rendre hommage, moi j'ai beaucoup travaillé avec lui, non, non, mais sur 3DS et sur engagement et proximité à chaque fois, il nous a trouvé des solutions donc Monsieur le DGCL et le roi des opérant donc encore quelques jours à la direction des collectivités, il va nous inventer la la solution très sincèrement, donc je vous remercie et je veux juste dire que ce ne sont pas les élus des communes nouvelles qu'ont découvert des nouveautés qui n'aurait pas vu, c'est que les lois de finance successives et les réformes sont venus impacter les prévisions qui étaient faites donc c'est pas eux qui sont aveugles, c'est qu'encore une fois on a changé le monde, alors même qu'on leur a dit que cette réforme, elle se déroulait dans un cadre merci beaucoup et à très bientôt à tous Merci madame la la présidente, madame la ministre, je voulais aussi souscrire aux propos de Madame Gatel et de beaucoup d'autres collègues, en effet, lorsque la loi a été présenté, c'était une proposition de loi sur les communes nouvelles, moi je me souviens, tout à fait être avoir parlé à cette tribune et avoir appelé à la prudence et avoir dit dans mon département, je ne ferai aucune propagande, je dirais que c'est un outil qui existe mais qu'il faut faire attention, je sais que dans certains départements, les préfets se sont faits militant en essayant de multiplier les communes nouvelles comme si c'était nécessairement mieux je crois que la solution des communautés de communes qui s'est développée au fil du temps, qui maintenant est généralisé, présente le grand Avantage de respecter l'identité de la commune, on peut faire tout ce qu'on veut, les Français ont la commune dans le coeur, quelle que soit la taille de la commune et ça permet de travailler ensemble tout en respectant cette entité et si naturellement des élus veulent faire une commune nouvelle, ils peuvent le faire, cela dit, je prends la suite de Madame Gatel pour dire que je pense qu'il est possible de trouver des solutions, il n'est pas vrai qu'il y a aucune possibilité de prendre en compte les évolutions qui sont intervenus et de sorte d'aberration par rapport à la DSR qui ferait qu'on serait moins rural du fait qu'il y aurait eu une communauté de commune, donc j'appelle de mes voeux avec un gars pour sans à Gap, le fait que, vraiment, on y arrive parce que je crois que ce serait justice par rapport à des élus qui n'ont pas pu mesurer parce que les lois de finances futur n'était pas encore voté, ce qui se passerait exactement. merci monsieur le questeur Monsieur Vial. par ces amendements, on a essayé de faire des propositions pour régler un certain nombre de problèmes, on a, on est tous conscient : ici, ça a été dit je veux je veux pas y revenir, que le problème perdure et perdurera qu'on vote ou pas, ces amendements et donc on est tous très favorables à trouver une solution, comme nous y invite d'ailleurs la, la, la Cour des comptes, et elle est pas la seule

sinon il faut arrêter le dispositif par contre je pense qu'on a un engagement et désengagement à tenir auprès de ceux qui ont déjà fait le choix soit convaincu par le militantisme de certains préfets c'est vrai ou du gouvernement, en tous les cas où des dispositifs qu'on leur avait proposé à l'époque et qui au final

j'envisageais en fait de de me rallier à la sagesse de la commission si vous avez eu des avis un peu plus nuancé, j'étais prêt à retirer un certain nombre d'amendements, si si, on a, on avait obtenu d'autres on on a un avis qui tombe de cette manière et sans aucune nuance, je ne me vois donc pas dans la possibilité de nuancer, moi-même et donc je maintiendrai tous ces amendements. Merci, cher collègue, alors je pense que là, tout le monde s'est exprimé et que nous allons pas au pouvoir passer au vote sur ces amendements, alors tout d'abord, nous avons une série de 3 identique 141 400 à 432 qui ont reçu évidemment 2 avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour.

Nous passons à l'amendement 253, il est présenté par Monsieur Féraud. Merci madame la présidente, et c'est moi, j'ai l'impression que mes collègues sont perturbées par le nombre d'amendements qui sont tombés, donc je présente l'amendement 253 la loi de 1999 qui crée la couverture maladie universelle a supprimé la participation obligatoire des communes aux dépenses d'aide sociale des départements et parallèlement à la minorer la dotation forfaitaire de chaque commune et augmenter celle des départements, la loi de finances pour 2022 ah elle supprimer la mention de la ville de Paris dans la rédaction de l'article 23 34 4 du collègue du code général des collectivités territoriales, mention qui permettaient de traiter équitablement l'ensemble des communes et la ville de Paris, dans le calcul de leur potentiel financier du fait de son statut particulier cumulant compétences communales et départementales, la ville n'a ainsi pas vu ça DGF communal minoré Nice DGF départemental augmenter en conséquence son potentiel financier communal n'a pas été minoré, comme c'est le cas pour les autres communes et le niveau de recettes pris en compte, a été minoré pour les autres communes, sauf pour la ville de Paris, cet amendement vise donc à revenir sur cette suppression intervenue en 2022, sans aucune concertation avec la ville et aboutissant un traitement défavorable pour que la Ville de Paris et le même traitement que l'ensemble des autres communes françaises, je vous remercie. madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues Monsieur Féraud, vous entendez par votre amendement, revenir sur la suppression de l'amélioration du potentiel financier de la ville de Paris, de la participation obligatoire de la de la commune aux dépenses d'aide et de santé au département de Paris constaté donc en 2007, ce retraitement se justifiait par le fait que désormais cette collectivité exerce des compétences départementales et lorsqu'on considère que, que par ailleurs, la réforme de la TH a une incidence très favorable au potentiel financier de la ville de Paris

Merci, monsieur le rapporteur, donc Madame la Ministre. Je vous donne un avis défavorable de la part du gouvernement et et je retiens les arguments présentés par le rapporteur. Merci Je mets aux voix Monsieur Féraud pour explications de vote. Merci madame la présidente, une nouvelle fois. La ville de Paris n'est pas traitée équitablement avec l'ensemble des autres communes de France, il faut le dire, je suis content d'entendre dire que vous considérez, Madame la Ministre, parce que j'aurais aimé vous entendre sur le sujet, considéré que le potentiel financier de la ville de Paris est suffisant, mais moi je veux le dire peut paraître un détail pour vous, mais voilà, pour nous, c'est essentiel pour reprendre ce que disait Nathalie Goulet et la chanson tout à l'heure, je pense que l'ensemble des communes, des collectivités, des territoires ont le droit d'être traité en équité, Paris et les Parisiens également. Merci Monsieur Féraud. Il n'y a pas d'explication de vote. Je vais mettre aux voix, donc l'amendement 253 qui a reçu 2 avis défavorables qui. Qui compte. qui. Qui compte. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 4 631 et c'est monsieur ah il est retiré. Alors 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 57 madame Noël. Merci madame la présidente, madame la ministre, il s'agit d'un amendement que j'avais déjà déposé en 2020, qui avait été adopté grâce aux voix de nombreux collègues sur tous les bancs de cet hémicycle et j'espère renouveler l'exploit à l'image de l'amendement adopté tout à l'heure par notre collègue Hervé Maurey, cet amendement a pour but de revoir le calcul de la répartition de de la part de dotation forfaitaire pour diminuer les inégalités entre urbain et rural aujourd'hui compris entre 1 et 2 l'écart entre les montants alloués aux plus petites communes et aux plus grandes serait ainsi réduit à 1 virgule six grâce à cet amendement,

proposent un coefficient de, de, de 1 5 au lieu de 2 1 6 mais mais j'ai du mal à comprendre qu'il n'ait pas été mis en discussion commune avec l'amendement tout à l'heure de notre collègue Hervé Maurey, qui a été adopté et donc je m'interroge sur la compatibilité de ces amendements, du coup je je je vais retirer mon amendement comme j'ai j'ai apporté ma voix à celui de mon collègue Hervé Maurey tout à l'heure, mais j'en profite de quelques-uns secondes de paroles qui ne soit accordées, Madame la Ministre, pour solliciter la même invitation comme mes collègues, intéressés par les communes nouvelles parce que les communes anciennes ou toutes les communes sont tous intéressés par la question de la voirie dont on a beaucoup parlé, et donc je compte bien qu'on ait aussi une réunion de travail sur la voirie, comme vous le proposez sur la question des communes nouvelles merci beaucoup. monsieur Sautarel et donc le 169 et retiré avis de la commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, oui effectivement, en écho à ce que vient de dire monsieur Sautarel ces trois amendements qui sont très proches de de celui de qui a été adopté de de monsieur Moret sont virtuellement satisfait donc je je vous propose de les, de les retirer ou de considérer qu'ils sont satisfaits, quoi, parce qu'effectivement, on aurait pu effectivement les discuter ensemble donc, sinon je vous demanderai de retrait et un avis défavorable, mais comme vous avez voté le Moret. Alors Madame la Ministre.

pas si Madame Vermeillet. Merci madame la présidente, cet amendement a pour objet de protéger les communes de moins de 1000 habitants, les empêchant d'être frappé par une DGF négative le mécanisme prévoit de supprimer pour ces communes, la ponction sur la fiscalité opérées lorsque le montant de la DGF n'est pas suffisant pour acquitter la contribution au redressement des finances publiques, il doit ainsi permettent de protéger les collectivités qui bien souvent rurales se voit, en plus de ce prélèvement sommé de contribuer à la péréquation par la contribution au FPIC c'est notamment le cas des des territoires touristiques de montagne dont plus de 50 pour 100 des hausses de fiscalité sont attribués à ces de prélèvements, donc cet amendement évite les DGF négative. Oui, je rappelle que, en fait 438 communes sont concernées par une j'ai j'ai DGF négative, dont 236 de moins de 1000 habitants, simplement le fait d'avoir une DGF négative n'a rien d'un d'incongru, hein, c'est quelque chose qui résulte de là d'un phénomène mécanique et le problème, c'est que c'est pas parce qu'une commune et petite que qu'elle est pauvre et quelque part, ça veut dire que on va peut être avantagé des, des, des communes qui ont une DGF négative parce qu'elles ont des ressources phénoménales par ailleurs sous prétexte qu'elles sont petites, elles vont être dispensé d'un effort que l'ensemble des collectivités supporte donc je ne peux que vous demander un retrait sinon être défavorable. merci alors Madame Vermeillet, explications de vote. Elle va être très courte, j'entends monsieur le rapporteur, mais symboliquement une DGF négative, c'est pas possible, voilà donc je le maintiens, cet amendement.

cet argent face à quelque chose de complètement délirant, et je suis désolé mais il y a aujourd'hui, Madame la Ministre des communes dans mon département comptait DGF négative et qui ne sont pas riche voilà et qui sont pas riches, alors il y en a plein qui sont à zéro depuis quelques années maintenant et qui sont pas riches non plus, alors peut-être, elles ont un potentiel fiscal élevé mais il faut regarder aussi la qualité de leur population, donc on sait bien que sur la DGF il y a un gros travail mais des des AGF négative, là je trouve que c'est le pompon, donc moi je voterai cet amendement. Alors je mets aux voix l'amendement de Madame Vermeillet. Qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour.

allez-y, chers collègues. Madame la présidente, un ministre le présent amendement vise à intégrer un critère de taux logements sociaux dans le calcul de la première fraction de la dotation de solidarité rurale dites bourg centre alors que notre pays connaît un important déficit de logements sociaux et considérant que la crise économique et sociale induite par l'épidémie Covid 19 va entraîner un besoin croissant de logements abordables pour nos concitoyens, il apparaît pertinente de récompenser les communes rurales qui prennent leur part de solidarité nationale en produisant de tels logements alors que le gouvernement souhaite par ailleurs que les collectivités locales jouent un rôle central dans la relance de notre économie, une telle mesure peut être de nature à inciter les maires de ces communes à produire du logement social, ne serait-ce que pour maintenir leur taux. Merci monsieur Stan, là on passe à l'avis de la commission. Parce que je suis. Oui, madame la président, mes chers collègues, il s'agit là donc d'intégrer à un critère de taux de logements sociaux dans le calcul de la fraction bourg, centre de la DSR c'est vrai que c'est pas véritablement incohérent avec la vocation d'un d'un bourg centre mais bon, quand on sait que la notion de centre est très variable, dans notre dans l'Hexagone, il serait sans doute nécessaire de faire des des évaluations et une une concertation plus large, mais enfin bon tant donné qu'on a rajouté d'autres critères, alors qu'on ne rejetait d'autres je je fais une demande de retrait, mais bon

Mon amendement le le pic, il propose que le principe du droit commun à appliquer aux collectivités, les départements, régions d'outre-mer hors Mayotte déjà en vigueur pour ce qui concerne le dispositif de prélèvement soit étendue aux dispositif de renversement du SMIC, ce qui permettrait d'accorder la même valeur aux critères de répartition du FPIC sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, pour éviter que des EPCI de l'Hexagone éligible jusque-là ne se retrouvent exclues par l'augmentation du nombre de PCI ultramarins éligible, il est proposé de faire passer la part les EPCI éligible au versement du FPIC de 60 % à 62,6 % le second demande que soit modifié les modalités de renversement du fric d'hommes en rendant l'ensemble des EPCI de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Martinique et de la Réunion éligible, et non plus les seuls 60 % des plus pauvres. Merci, et le second. Le 649 défendu très bien avis de la commission, monsieur le rapporteur. mes chers collègues, le le présent amendement donc vise à aligner sur le droit commun, les modalités de versement au titre du FPIC FPIC nous semble que un tel dispositif serait inéquitable pour les ensembles intercommunaux de l'Hexagone, dans la mesure où ceux d'outre-mer ne voient pas leurs ressources d'octroi de mer prise en compte donc l'octroi de mer et quand même un gros différentiel et je vous le savez, chers collègues, aux patients et depuis longtemps pour le 2ème, le 649 qui vise à augmenter de 33 à 60 % le taux de majoration de la population prise en compte, là aussi, on n'a pas évidemment de de, mais enfin il s'agit d'une enveloppe fermée d'un milliard donc comme d'habitude, ce qui est donné aux heures non plus et t'enlevé aux autres. je crois que ce sont des discussions qu'il faut avoir préalablement avec le gouvernement, qui éventuellement après un chiffrage peut revenir vers l'Assemblée pour faire voter, cela est peut être pas par un amendement dans plutôt des demandes de retrait sur les deux amendement. Merci, monsieur le rapporteur, même avis, Madame la Ministre. Absolument, madame la présidente, mais oui, même à bien. Alors Monsieur passion vous maintenez vos amendements vous les retirer. est une recette de fiscalité indirecte et dans l'Hexagone, les recettes de fiscalité indirecte ne sont pas prises en considération quand il s'agit de calculer le flic. Merci les 648 et 649 sont donc retirés merci Monsieur patients alors le 700 de rectifier Merci madame la présidente, madame le Ministre, chers collègues, c'est un amendement qui avait déjà été déposée il y a quelques années et qui se propose d'organiser le ruissellement des métropoles vers ce qu'on peut appeler leur arrière- pays en mettant en place le 1 % métropoles, vous savez que chacun dans nos territoires, les métropoles concentrent la richesse intellectuelle, la richesse financière, les investissements et qu'il est nécessaire parfois que la solidarité, qui n'est, qui n'est pas si naturel que ça, qu'on renvoie souvent des contrats de réciprocité, certaines collectivités et je pense notamment à des grandes villes françaises ont commencé ce travail mais il met bien du temps à à rentrer dans la réalité, et donc ce que l'Association des Petites Villes de France a proposé déjà à plusieurs reprises, c'est de créer une occasion d'organiser cette solidarité du de la métropole vers l'arrière pays. Merci, cher collègue, avis de la commission. Oui, c'est un amendement que l'on a vu quelques fois. Il vise à instituer un fonds régional de solidarité inter-territoriale alors dans le détail, 1 % des recettes tirées de la fiscalité professionnelle par la métropole seraient prélevés sur cette dernière mis à chaque année à la disposition de la conférence territoriale, l'action publique afin de financer des projets structurants alors bon ce c'est un dispositif supplémentaire parce qu'il y en a déjà beaucoup, un tel dispositif semble donc. Redondant par rapport au pic auquel les métropoles contribue très largement, ensuite on on peut dire que la métropole et l'activité métropolitaine contribue beaucoup ressources départementales qui ont justement vocation à revenir vers les projets territoriaux et puis on peut indiquer également que la la suppression probable de la CVAE limiteraient d'ailleurs a fortement la portée d'un tel font parce qu'alors on ne sait plus exactement ce que l'on donnerait si c'est une part de TVA après, enfin, c'est plus de Donc défavorable notre position sera défavorable, même si nous sommes très en faveur de l'Inter territorialité de la solidarité des territoires ruraux et des territoires urbains, mais, pour les raisons invoquées, particulièrement le fait que l'c'est c'était à n'est pas une instance décisionnelle, la position du gouvernement est défavorable. Merci madame la ministre, pas d'explication de vote si Monsieur Hervé. Oh, je vais maintenir la l'amendement malgré la demande de retrait de de la part de monsieur le rapporteur, on ne peut pas hein seulement invoqué la solidarité, dire qu'il faut que les élus l'organisant en entre eux alors que nous voyons très bien que il y a des des territoires dans lesquels elle l'étant en passe de devenir réalité. Dans d'autres, ça n'est pas absolument pas le cas, les démographes les économistes montre aujourd'hui que dans notre pays la métropolisation, c'est la concentration de la croissance de la richesse de et et y compris sur le plan sociologique, j'entendais tout à l'heure que les métropoles qu'on qu'on sente les pauvres mais enfin faut faut regarder aussi la réalité non il y a, il y a, il les périurbains, les territoires ruraux en proximité sont aussi des territoires qui sont des rives Touaregs parfois sociologiquement en souffrance, c'est pas la gentrification, elle se fait essentiellement aujourd'hui dans les centre-villes des métropoles, bien plus que dans la ruralité, proche de, de, de, de ces, des risques de rupture donc je maintiens cet amendement je pense madame la madame la Ministre, si vous avez encore un peu de temps parce qu'on a vous avez vous voulez bosser, j'ai comme une nouvelle, mais je pense que sur ce thème : thème : là, il y aurait de quoi organiser un groupe de travail sous votre égide pour réfléchir à ça. Alors la parole est à monsieur Marie. Merci madame la présidente, madame ministre-là l'amendement de mon collègue Loïc Hervé Loïc Hervé a un grand mérite, c'est qu'il pose la question de la coopération entre les métropoles et leur environnement immédiat, la solution du un % est une solution parmi d'autres, elle n'est peut-être pas la meilleure, comme l'a rappelé le rapporteur spécial puisque d'autres moyens de concourir à la solidarité financière existe mais il est impératif de revisiter les dispositifs existants aujourd'hui les pôles métropolitains n'existe pas ou ne fonctionne pas et et quand ils existent, il concerne quelques compétences partagées, qui ne sont pas financés, or il y a des exemples qui fonctionnent, si vous prenez la métropole de Rennes qui a mis en place un dispositif de collaboration avec l'ensemble des communautés de communes, de son environnement, si vous prenez, y compris celle dans laquelle je suis à Rouen, il y a des possibilités, le seul problème c'est qu'aujourd'hui, il faudra arriver à structurer cela et à le rendre obligatoire, car autrement les métropoles restent campés pour certaines d'entre elles sur leur territoire sur leurs compétences et ne discute pas avec l'ensemble des communautés de communes environnantes, ce qui pose un véritable problème, on pourrait citer différents sujets le 1er d'entre eux étant celui des transports par exemple. Alors Madame la ministre souhaite prendre la parole, mais je voudrais dire que si vous souhaitez encore il y a une possibilité de finir la mission avant 20 pour 20 heures à condition de faire du trente amendements à l'heure, donc ça veut dire ramasser, vous avez le choix, ministre. Oui merci madame la présidence, je voulais juste répondre favorablement à l'appel à réflexion et groupes de travail par contre pas la semaine prochaine mais en janvier, sur 2 sujets : le sujet de la coopération territoriale entre les métropoles et les territoires ruraux cette réconciliation d'été des territoires, donc on posera tout en janvier, une réunion de travail, et il est parti, monsieur le sénateur, mais on va aussi en janvier, de travailler sur la voirie, je vois la masse d'amendement qui a été proposé sur ce sujet, donc voilà, je réponds favorablement ces 2 groupes de travail complémentaire à celui des communes nouvelles. Donc je mets aux voix cet amendement ou on le retire, on le maintient, hein, on est bien d'accord, je mets aux voix cet amendement qui a reçu 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté. Nous avons trois amendements en discussion commune 515 monsieur Iacovelli. Oui, madame la présidente, madame amis chers collègues je cet amendement et est porté au nom de plusieurs communes des Hauts-de-Seine concernant le calcul des indicateurs de richesse comme le potentiel fiscal et le potentiel financier qui ont été modifiés dans la loi de finances pour 2021 et pour 2022 pour intégrer les effets des réformes fiscales de 2021, notamment la suppression de la taxe d'habitation de la division par 2 de la CFE- et de la taxe foncière sur les propriétés bâties des établissements industriels. La répartition des dotations et de péréquation horizontale des communes et intercommunalités : d'une part et des départements, d'autre part, impose de calculer les indicateurs distingue pour la ville et le département de Paris qui forment une collectivité territoriale à statut unique là les lois de finances prévoit un calcul dérogatoire des indicateurs de richesse de la ville et du département de Paris qui conduisent à ne pas appliquer le même traitement qu'aux autres collectivités auxquelles elles sont comparées à l'échelon communal d'une part, et à l'échelon départemental, d'autre part, concernant la répartition des dotations et des péréquation horizontale, la ville de Paris a certes bénéficié d'un traitement spécifique pour la compensation de la suppression de la taxe d'habitation, laquelle a été intégralement compensée par une part de la TVA, ceci étant, cette particularité n'interdit en rien de calculer le potentiel financier de la ville et du département, selon une règle similaire aux autres communes et aux autres départements, garantissant ainsi l'égalité de traitement entre les collectivités de chaque échelon dans les dispositifs de péréquation de la couronne parisienne, c'est notamment un enjeu important, s'agissant de la répartition des contributions au Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France dont Paris représente 61 % en 2022 par cet amendement, je vous propose donc, mes chers collègues, de modifier le calcul du potentiel fiscal et financier de Paris, ainsi que ses indicateurs pour qu'ils soient calculés de la même dans les mêmes conditions que les autres villes et les autres départements et à garantir ainsi l'égalité de traitement de la répartition des dotations et des fonds de péréquation, je vous remercie. sénateur Iacovelli a déjà dit l'essentiel, il faut de l'équité dans dans le calcul, or aujourd'hui, il y a un déséquilibre entre Paris et les communes de leur proche couronne qui est et qui est due à la situation ancienne de Paris, qui était à la fois, ville et département, ça n'est plus le cas aujourd'hui, ce que nous souhaitons c'est que il y ait un calcul des nouvelles bases pour que toutes les communes soient traités avec équité et surtout pour éviter que les villes périphériques de Paris contribue à proportion de façon plus importante afin de compenser la contribution réduite dont bénéficie encore Paris, voilà, c'est l'essentiel de notre amendement merci madame président. à madame Lavarde. Oui merci madame la présidente, donc effectivement, comme l'ont dit à mes collègues, cet amendement concerne l'ensemble des communes d'Île-de-France, et pas uniquement les communes des Hauts-de-Seine, donc ça serait pour dire que d'autres personnes ici peuvent être concernés puisque indirectement le calcul du potentiel financier de la Ville de Paris, a des répercussions sur la répartition du skiff et comme le dit très justement la page 6 du document qui a été présenté au comité des élus du Trift en raison de la diminution de son potentiel financier, la contribution de la ville de Paris est en légère baisse alors une légère baisse pour Paris se traduit mécaniquement par une hausse qui peut être très importante pour les autres communes contributrices et celle notamment qui arrive juste derrière la ville de Paris alors en l'état, en fait, ces trois amendements font la même chose sur la première partie, à savoir vous venir revente filer la disparition de la TH au niveau de la ville de Paris comme cela a été fait pour les autres communes de France, par contre, quand on fait ça, il y a un effet incident sur le calcul du potentiel fiscal, du département de Paris qu'il convient de corriger parce que si on ne le fait pas, ça a des conséquences sur un autre fonds de péréquation qui est le Fonds départemental alors c'est ce que fait aussi mon amendement, il le fait d'une manière qu'on peut juger un peu parfaite mais j'avoue que, pour avoir cherché pendant plusieurs semaines, j'ai pas trouvé de solution parfaite, mais il me semble important de souligner là en tout cas ça peut permettre de travailler pendant un an, cette question en avançant et pour les communes et pour les départements. Merci madame Lavarde monsieur le rapporteur monsieur Gainey. Madame la présidente à la ministre, mes chers collègues, oui, ces trois amendements une vocation commune, c'est vrai que certains indicateurs financiers ont avantagé la ville de Paris comme on l'évoquait tout à l'heure et l'amendement revient donc à créer une sorte de de coefficient correcteur fictif, bon nous sollicitons l'avis du gouvernement pour savoir si vraiment pas mieux faire des des travaux complémentaires pour aboutir à un accord négocié sur ces bases-là, plutôt que de faire ça ici, mais peut être avez-vous. Merci madame la présidente, madame et messieurs les sénateurs, dans le prolongement de ce qui vient vous êtes dit par le rapporteur. Les modifications que vous proposez ne nous semble pas aboutir au résultat souhaité le potentiel financier de Paris pourrait en réalité être minorée par rapport à son niveau actuel, ce qui augmenterait la contribution des autres communes OFS R. sur ce type de sujet et afin de bien évaluer l'ensemble. Des impacts, comme cela vient de vous être dit il nous semble indispensable de prendre le temps d'échanger afin d'aboutir à une solution partagée, j'ajoute que la Ville de Paris pourrait utilement être associée à ces réflexions, donc je rejoins la demande de retrait merci.

Merci madame la présidente, madame la ministre, je, je, je suis très impressionné par le soutien politique que vous accordez à mon collègue Iacovelli, à quelques mois des sénatoriales, je pense que ça va lui rendre un grand service, je pense qu'il va être, il va être très heureux en revanche

aujourd'hui, il y a une disparité de fait entre la contribution parisienne et la contribution des communes, comme le disait très justement ma collègue Lavarde qui est, qui est le résultat de du du statut particulier de Paris aujourd'hui, il faut absolument aplanir tout ça est revenir à une règle commune, c'est-à-dire que la contribution parisienne soit calculé comme toutes les compromissions des des communes, franchement c'est pas compliqué et les élus trouveraient que ça serait une mesure tout à fait légitime merci madame la présidente.

ne sont pas sans rapport avec l'amendement que j'ai présenté tout à l'heure et qui a été rejetée, puisque si on modifie les critères dans l'article L 23 34 4 du code général, ça ne peut pas être à la tête du client, donc ça doit être quand cela et montage Paris comme ça, quand cela le désavantage alors ça peut paraître peut être un peu baroque, le débat, ce débat qui là est entre les Hauts-de-Seine et Paris, qui n'ont pas la réputation d'être dans les départements les plus pauvres de France, je tiens quand même à rappeler une chose, c'est que Paris et ses 2 1000000 100000 habitants, si je vous dérange pas. Bah, Cécile. Soit 40000 euros de DGF en tout et pour tout et versent plus de 700 millions d'euros de péréquation nationale et régionale, donc il faut rétablir aussi la réalité des chiffres par rapport au potentiel fiscal et financier mais aussi par rapport à la solidarité et au fait que Paris participe à la solidarité nationale entre les collectivités. Alors, moi, c'est juste pour préciser que ces questions sur les le modalités de répartition du c'est pas la première fois que j'en parle dans cet hémicycle, je pense que j'en parle à chaque PLF l'année dernière j'avais déjà eu des discussions avec le la DGCL parce que j'avais porté antérieurement à un calcul enfin un amendement qui visait le double compte de la CPS dans calcul du la DGCL enfin les services avait reconnu que j'avais raison mais qu'il était il fallait par porte remettent ce sujet sur la table ce qu'on doit avoir une réforme pour la réforme ne venant pas, là on vient sur des montants qui sont substantiellement plus élevé que ce double compte de la CPS qui est qui concernait certaines communes, celles qui avait une ancienne taxe professionnelle très élevé,

donc déjà pour l'année dernière, je me souviens que quand nous avions parlé des indicateurs et que vous étiez venu ajouter certains critères comme les droits de mutation pour venir rehausser le potentiel financier de la ville de Paris qui se trouvait sinon minoré en appliquant le droit on m'avait répondu que ça n'aurait une incidence que sur la ville de Paris, au regard du poids de la ville de Paris dans le poids des DMTO nationaux, c'était certainement vrai si on en oubliant que dans une ville de Paris, il a, villes et départements sur les DMTO, donc si on reprend attise la part que de la ville de Paris et qu'on la compare à la part des DMTO des autres villes, la comparaison n'est peut-être plus tout à fait vrai et c'est peut-être ça qui explique que quand on a calculé le Street en 2022 devant le comité des élus, on a cette phrase, le potentiel de la ville de Paris, financer la ville de Paris ayant diminué les autres communes sont appelées à contribuer et ce que je voudrais dire ici, c'est qu'on a quand même un vrai problème démocratique dans la répartition de ce fonds, le comité des élus du Sri font un tableau qui ne dit rien du calcul du calcul de l'indicateur synthétique, alors je vais pas le répéter ici la formule compliquée mais donc, on ne sait pas comment les variations se font d'une année sur l'autre entre les différentes communes contributrices et c'est la même chose pour celles qui perçoivent donc si cette boîte noire, on ne peut pas l'ouvrir devant le Parlement qu'elle ait pas plus ouvert, devant le comité des élus qu'est-ce qu'on fait et vous allez nous dire : on va se revoir dans un an, sauf que dans un an, les communes contributrices elles auront continuer à payer en 2000 22 et en 2023.

Ah pardon, excusez-moi chers collègues. Je voudrais surtout pas rallonger excessivement les débats, mais il faut quand même puisqu'on a, on a des éléments très, très précis et on est désolé de monopoliser un petit peu le débat concernant les communes d'Île-de-France, néanmoins, pour que les collègues étaient un petit peu ça en tête, l'ensemble du fonds dont nous parlons aujourd'hui, c'est 350 millions la ville de Paris contribue à hauteur de 183 donc, non, mais je voudrais juste que vous n'aviez pas l'esprit l'idée que, voilà que Paris, c'est terrible, c'est vrai que ce ne sont que des sénateur des Hauts-de-Seine, qui se sont exprimés, donc du coup on a un effet loupe sur la situation des Hauts-de-Seine, donc je pense que dans un mécanisme qui était extraordinairement complexe, d'ailleurs, en vous écoutant chers Christine Lavarde je pense que vous nous aviez perdu à la à la 8ème phrase je pense qu'il faut y travailler de manière très sérieuse, mais qu'on ne peut pas me semble-t-il, remettre à plat l'ensemble du dispositif du Sri et les les modalités de répartition entre telle ou telle commune comme ça mais voilà je tenais quand même à ce que vous sachiez qu'elle était le montant des contributions de la ville de Paris par rapport au à l'ensemble du fond.

quand ça nous arrange et faire voter quand ça nous arrange rapidement et donc en l'occurrence, moi je pense que, aujourd'hui, on est dans une situation Christine Lavarde là très bien argumenté, ça ne concerne pas d'ailleurs que les Hauts-de-Seine et d'ailleurs, je rappelle que, dans les Hauts-de-Seine, il y a pas que des communes riches, il y a aussi des situations difficiles, dans un certain nombre de nos communes et ça concerne toute l'Île-de-France, les 8 départements d'Île-de-France, et donc on a besoin effectivement aujourd'hui d'avoir une équité entre les différentes communes qui composent l'Île de France et c'est pour ça que je pense que, en tout cas pour ma part je maintiendrai l'amendement. Merci monsieur Iacovelli alors je vais mettre aux voix les amendements identiques : 515 et. 693 qui ont reçu un avis. Un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui. du gouvernement qui. S'abstient ne sont pas adoptés, je me vois le 37 rectifié bis qui a reçu 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté. Alors je vous propose de faire une suspension de séance à deux à de 5 minutes à la demande du gouvernement.

Allez, la séance est reprise. Le 696 monsieur Julia. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est toujours le fond de solidarité des communes de la région Île-de-France, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus simple les communes qui sont contributrices, elles, elles ont un prélèvement qui aide mensuel, donc l'État prélève tous les mois mais en revanche, les communes bénéficiaires, elles, elles ont un versement par moitié le 31 juillet et le 31 décembre donc, elles font l'avance de trésorerie pour le compte de l'État, ce qu'on souhaite par cet amendement, c'est que bien évidemment, prélèvements et versement se fasse mensuellement, ce qui serait une réforme très simple merci présente je fais court. C'est très gentil merci, monsieur le rapporteur. Avis du gouvernement. Favorable. Favorable donc favorable pour la commission, je mets aux voix l'amendement 696 qui a reçu 2 avis favorable qui est pour.

La dotation de continuité territoriale est un concours individualisé de l'État versée à la collectivité de Corse pour lui permet de mettre en oeuvre le principe de continuité territoriale telle que définie en 1976 en organisant et finançant les dessertes maritimes et aériennes liant la Corse continent. Les modalités de versement de la dite dotations sont précisés à l'article L. 44 25 tiré 26 du code général des collectivités territoriales. Depuis le statut Joxe de 1991 les reliquats de l'enveloppe de la continuité territoriale peuvent être affectés aux infrastructures portuaires et et aéroportuaires, l'article 142 de la loi 2016 1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a étendu cette possibilité aux infrastructures routières et ferroviaires, jusque-là, je dirais que tout cela reste cohérent, or la dernière évolution intervenue en 2017 constitue en revanche une dérive qui met à la fois en péril le bien-fondé de cette dotation, ainsi que le financement des infrastructures de transport. Fruit d'un accord politique entre le ministre de l'époque et la nouvelle majorité territoriale la des spécialisations total de l'enveloppe fait courir un risque au versement de la dotation par conséquent à travers cet amendement, il est impératif de préserver l'affectation de la dotation de continuité territoriale aux infrastructures de transport et de l'actée dans la loi l'objet du présent amendement et de respect chez Alizée, l'enveloppe, il appartiendra à la collectivité de financer directement les autres programmes sans avoir à obérer les financements prévus pour les transports, ce serait une opération neutre pour la collectivité de Corse qui flèche les reliquats sur les investissements concernant les infrastructures de transport et préserverait le bien-fondé du versement de la dotation de continuité territoriale, d'où la nouvelle rédaction proposée afin d'encadrer l'utilisation de ces reliquats pour les réserver aux infrastructures de transport. avis de la commission et de respect, c'est Alizée, le reliquat de la la DCT ça aurait l'Avantage de d'être beaucoup plus en cohérence avec l'objectif initial et en plus ça émane légitimement du terrain, nous ne pouvons qu'à tout le moins, vous donnez une sagesse mais on va voir ce que nous dit le gouvernement. Madame la ministre avait du gouvernement. Merci madame la présidente, donc concernant. L'amendement 126 la dotation de continuité territoriale-là DCT s'établit à 187. Millions d'euros par an, c'est une recette affectée qui vise à compenser les contraintes liées à la continuité territoriale, le montant du droit à compensation était calculé selon les modalités classiques en matière de transferts de compétences, c'est-à-dire au coût historique de sorte que les crédits transférés par l'État correspondait aux crédits inscrits en 1992 au budget du ministère en charge des transports, les dépenses de continuité territoriale se sont fortement réduites entre 2013 et 2019 passant de 189,5 millions d'euros à 161,2 millions d'euros, c'est d'ailleurs pourquoi la loi de finances initiale pour 2017 a ouvert la possibilité d'affecter les reliquats de la DCT à des opérations hors continuité territoriale et notamment la réalisation d'opérations d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l'intérieur et de la montagne, la mesure que vous proposez, Monsieur le Sénateur, étant susceptible de rigidifier les marges de manoeuvre financières de la collectivité de Corse dans un contexte socio-économique fragile, le gouvernement n'est pas favorable à cet amendement et vous en demande, si vous le voulez bien le retrait. De ce nous. Monsieur Panunzi pour explication de vote. Madame la ministre, je pense qu'on vous a mal informé. Et que vous n'avez pas analyser le principe. Il y a une dotation de continuité territoriale qui est versée à la collectivité de Corse pour le transport maritime et aérien de 187 millions d'euros par an. Cette dotation n'est pas consommés en totalité, tous les ans. Et. La loi de 91 qui avait compris le principe. Faisait en sorte que les reliquats puisse être. Consommer. Par des crédits alloués aux routes, aux porcs et aux aéroports aujourd'hui avec la des spécialisation de l'enveloppe, vous avez 50 millions d'euros depuis 2000 2017 jusqu'à 2021, qui se sont évaporés dans le budget de fonctionnement de la collectivité territoriale et qui ne sont pas utilisés sur les infrastructures portuaires, aéroportuaires et routières, donc je demande en toute logique que ces crédits soient consacrés aux infrastructures de transport, comme le souhaite la loi. Si Monsieur Panunzi. Alors, je vais mettre. Oh voit cet amendement 126 qui a reçu un avis de sagesse de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté. 568 il est présenté par Monsieur Delcros. Merci madame la présidente. Dotation sur été rural et réservé aux communes rurales, c'est vrai pour l'immense majorité des collectivités mais il s'avère qu'il y a quelques anomalies, il y a quelques communes qui cumule la DSR et la DSU, ce qui paraît quand même assez curieux, donc mon amendement propose de ne pas pas permettent ce cumul, tout en permettant à chaque collectivité qui cumule de garder la dotation la plus importante. Ce Delcros, monsieur le rapporteur. Oui merci monsieur Delcros, vous savez, chers collègues, que je suis par nature circonspect vers envers tous les non-cumul, mais bon, on peut quand même imaginer que, dans certains territoires, peut être ça puisse s'entrecroiser et qu'il puisse y avoir les deux c'est pour ça, nous considérons que le sujet devrait être un peu plus expertiser parce que ça n'est pas forcément impossible et en tout état de cause, je vous dis d'y penser quand même pour les comme une nouvelle au cas où l'amendement serait accepté parce que dans ce cas il faudrait vérifier les mettre en exception lorsqu'elles ont à la fois de la DSU, hein, d'accord, mais donc plutôt une demande de retraire. Merci madame la Ministre. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur Delcros, alors il me semble que vous venez de voter, il y a pas très très longtemps, le cumul de la DSR et de la DSU, sur les communes nouvelles, là il y a quelques minutes, donc c'est un peu surprenant, mais pas de problème, donc là vous nous proposer d'interdire le cumul de la DSR et de la DSU et la position du gouvernement est défavorable. Je pense que c'est un peu long, cet amendement, d'après nous, et avec les travaux qui ont été faits par les services conduirait à de lourdes pertes pour des communes déjà fragile, je vous. Merci monsieur Corbizet, vous avez la parole et puis Monsieur Delcros. National la présente, je rappelle que l'addition des deux existe parce que je prends l'exemple de ma commune qui était une ville minière et comme vous le savez, la plupart des communes minières Nord-Pas de Calais ou ailleurs à de plus de 10000 habitants faisaient partie des communes les plus pauvres de France et donc on avait des des sommes au niveau de la DSU ma commune toucher un million huit 2 millions d'euros par an d'otite de la déçu mais à part du moment où je suis passé juste sous la barre des 10000 habitants, j'ai commencé à toucher de la DETR j'interroge le préfet me dit est-ce que c'est possible oui parce que, sous la barre des des villes de moins de 10000 habitants, les 30 communes les plus pauvres sous la barre des 10000 habitants, donc les 33 communes seulement on pouvait toucher en plus de la de terre donc cela existe dans le texte. Si Monsieur Corbizet monsieur Delcros. vais je vais retirer mon mon amendement, mais je voulais quand même attirer l'attention là-dessus, je pense que les mécanismes devraient être regardé de près sans enlever de dotation au aux collectivités pour qu'on puisse avoir finalement deux ensemble des joints, d'un côté, la DSU, d'un côté la DSR sans rien retirer à ce qu'ils perçoivent l'idée, c'est pas que les les communes perçoivent moins mais qu'on ait quelque chose qui soit cohérent avec ses dotations. Donc l'amendement 568 et nous passons.

c'est un moment qui sont à Sup à supprimer l'article 45 bis : cet article prévoit l'ajout d'un nouveau critère dans la détermination par les préfets de départements et de régions du taux de subventionnement des attributions de DETR et 2 en 1er lieu l'ajout d'un nouveau critère fondé sur le caractère écologique des projets proposés pourraient entrer en contradiction avec les critères déjà défini dans la loi pour l'attribution de ces projets, il convient de ne pas altérer la procédure d'attribution dont les élus te trouve souvent en particulier par déciles qu'il n'est qu'elle n'est pas d'une parfaite lisibilité. Et par ailleurs le critère particular mon vague et pourrait s'avérer inopérant en effet l'appréciation par le préfet du caractère écologique du projet pourrait ça VRT s'avérer malaisée, s'agit-il par là d'évaluer les conditions de réalisation du projet ou alors son but final faute de clarification nécessaire le présent amendement prévoit de supprimer 7 heures l'éthique, c'est pas parce qu'on peut pas une préfecture envers qu'on fait de l'écologie. Merci, cher collègue, le 409 Monsieur bonhomme. 223 34 36 et 23 34 42 du code un paramètre écologiques qui, pour le moins surprenant pour la fixation des taux de subvention de DETR de des six pour les préfets de départements et de régions, or la terminologie caractère écologique retenue n'est pas satisfaisante à mon à mon sens le mot écologie a plutôt une connotation politique ou scientifique ou que que juridique, véritablement, par conséquent, la définition du caractère écologique apparaît beaucoup trop imprécises, on peut se demander sur quels critères objectifs en effet le préfet va-t-il se déterminer pour qu'un projet soit effectivement écologique et et en plus de cela, s'ajoutent des interprétations différentes de département à département qui peuvent avoir lieu par conséquent cet article vient complexifier inutilement une procédure d'attribution qui n'est pas toujours facile pour les élus locaux de de maîtriser parfaitement, et comme le dit mon collègue, il ne suffit pas d'ajouter des épithètes de les collectionner, sur fond de greenwashing pour être vertueux en matière d'environnement. Merci madame la présidente, en complément des arguments qui viennent d'être développés par nos collègues, je voudrais citer quelques opérations qui sont aujourd'hui dans mon département, financé par la de terre par exemple, l'opération de câblage d'une école pour équiper les écoles en tableaux numériques, par exemple, le renforcement de voirie pour pas pour que les Cars de ramassage scolaire puisse passer dans certaines communes ou par exemple encore la construction d'une maison d'assistantes maternelles, faire rentrer ces projets dont je n'ai pas besoin de développer sur le caractère essentiel dans le critère nouvellement institué de caractère écologique par ailleurs dans les départements, nous sommes en toute Intelligence en situation de nous mettre d'accord, y compris avec les services de l'État et les préfets sur un certain nombre de problématiques à résoudre je dans mon département de la Seine, il y a eu un gros sujet par exemple autour de la défense incendie et de manière intelligente, nous avons décidé ensemble que la DETR DETR puissent financer un certain nombre de travaux pour défendre nos communes contre l'incendie, donc je crois que ce critère est effectivement tout à fait mal et comme l'ont dit, nos collègues, je crois que l'écologie mérite mieux que de devenir un critère qui vise à sélectionner et clairement à écarter un certain nombre de projets de nos communes. Merci madame brûle un avis de la commission sur ces trois amendements. Oui, mes chers collègues, d'abord il faut regarder les choses comme elles sont : cet cet article 45 bis a été introduit à la demande des rapporteurs spéciaux à l'Assemblée nationale, ce n'est pas une proposition du du gouvernement et donc vous savez comment on est, on n'est pas on n'est jamais contre le fait de supprimer un amendement venant de l'Assemblée nationale, je plaisante, je plaisante, parce qu'il y en a qui vont le croire donc donc 1er point 2ème point la formule c'est les préfets tiennent compte du caractère écologique des projets, comment dire, c'est pas très normatif, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est bon, c'est moyennement ambitieux du du point de vue global, c'est-à-dire de l'idée que, de toute façon, sur les projets aujourd'hui, or des consommations la question énergétique la question environnementale elle est quelque part, prise en compte déjà beaucoup au niveau des commissions ce ça existe, nous on avait noté simplement que une telle disposition relever davantage de la circulaire, éventuellement, c'est-à-dire une orientation du gouvernement vers les préfets, orientation, je dis bien que, en tout cas d'un texte de loi et et donc écoutez, puisque vous vous demandez si gentiment on on va proposer de le retirer, on va être favorable à ces quatre amendements. Merci, monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, le gouvernement va être défavorable sur les trois amendements. vous proposer de supprimer l'article 45 bis qui prévoit l'ajout de nouveaux critères dans la détermination par les préfets de départements et de régions du taux de subventionnement des attributions de DETR et de si cet amendement, s'inscrit dans le mouvement de verdissement des concours financiers de l'État. Au concours aux collectivités locales, traduisant ainsi l'engagement du gouvernement en faveur de la transition écologique ne vous moquez pas, s'il vous plaît, il n'est pas question de peindre verdir ni la préfecture, mais bien de verdir nos projets tout en maintenant les critères d'attribution de ces dotations et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires auxquelles elles sont soumises, il permet d'inciter d'encourager les projets vertueux pour l'environnement à travers une majoration du taux de subvention appréciée par les préfets pour la DETR, cette appréciation s'effectuera en outre dans le respect des catégories d'opérations prioritaires et des taux minimaux et maximaux maximaux de subventions, fixé par la commission des élus cette démarche existe. C'est que des marchés éclairagiste par ailleurs déjà dans certains territoires, merci madame la présidente, telle que l'Ariège qui instaurer un bonus transition écologique pour la DETR ou encore la Drôme qui attribue des bonifications dans le cas de la DETR et de la décide, pour des projets vertueux, l'enjeu se situe plutôt dans l'amélioration de l'analyse des projets permettant d'identifier ce qui contribue réellement à la transition écologique l'instruction ministérielle pour les programmations 2023 portera à la connaissance des préfets une grille d'analyse des projets en ce sens, celle-ci permettra, je le pense aux préfectures de mieux analyser valoriser les projets présentés par les collectivités et contribuant positivement à la transition écologique. merci madame la ministre, s'il vous plaît ou ne pas être d'accord, merci madame la Ministre. Au Canada. Alors, nous allons passer aux explications de vote, à l'heure, on nous commençons par Madame Goulet. Ah, la présidente, mais à la ministre, vous qui êtes tellement attachés à la constitutionnalité du droit de de ce que nous votons ici, je pense que le caractère écologique est quand même une notion tout à fait vagues tout à fait imprécise et et tout à fait indigne à mettre dans les dans les hé oui absolument, je pense que je pense que, aujourd'hui, il y a des critères ce critère-là est absolument imprécis, il rajoute à la confusion et dont on a parlé ce matin, je pense que la commission des lois, et son rapporteur ont très bien fait de déposer cet amendement de de suppression que je voterai. Merci madame Boulet Madame Gatel. Madame la présidente, madame la Ministre, il n'y a plus de projet qui ne soit pas pure, d'une manière écologique, aujourd'hui il y a plus amer qu'il le fait parce qu'il y a tellement de normes qui oblige à des des équipements vertueux et c'est très bien et Madame la Ministre, vous avez cité des exemples qui naissent du terrain dans certains départements, les élus et le préfet ont décidé d'organiser les choses comme ça, c'est l'esprit même de la DETR pourquoi est-ce qu'on revient tout le temps à dire, du coup, on va mettre dans la loi cette bonne pratique madame la Ministre, encore une fois, il faut qu'on aille tous faire un tour en Mayenne, avec le président de la République, il dit : liberté, responsabilité locale mais les élus sont vertueux, Madame la Ministre, arrêtons de leur interdire des choses ou de leur imposer des choses qu'le font naturellement, comme Monsieur Jourdain faisait de la Pro. Oui merci madame la présidente, madame la Ministre, moi je soutiendrai bien évidemment ces ces amendements avec l'avis favorable de la commission parce que, comme l'ont rappelé plusieurs collègues la liberté locale est importante, d'autre part, chaque territoire a ses particularités, il y a une commission d'élus qui peut fixer un cadre particulier et je crains qu'avec ce critère de caractère écologique, une fois de plus, ce soit les routes alors que comme on l'a rappelé, par ailleurs, c'est un instrument pour toutes les mobilités qui soient victimes demain dans les arbitrages et DETR de de cette, de ce critère, alors même qu'on n'a pas pour l'instant, construit un fonds dédié au financement de notre voirie communale, donc bien évidemment, je souscris à ces amendements qui me semble sage et de libertés locales merci. Monsieur Hervé. Oui merci madame la présidente, sous le couvert du président de la commission des lois, si la commission des finances est jalouse de la préservation de l'OTAN de l'nord de l'orthodoxie financière, nous nous sommes jaloux de de de l'orthodoxie de la de la rédaction de la loi et de la qualité du droit, nous n'aimons pas les adverbes et le niveau, les mots ne vont pas les verbes imprécis,

des choses et. Bon, on n'est pas loin du greenwashing, pardon de le dire, mais on met dans le droit des un alourdissement et des choses qui ne font rien avancer et l'autre élément qui qui me semble être l'autre argument qui me semble être le plus important, c'est la confiance faites aux élus locaux et je vais prendre un exemple tout simple, dans mon département, la Haute-Savoie en Haute-Savoie, les élus locaux ont décidé dans les critères de la DETR de donner une bonification pour l'emploi de bois local 10 points de d'ETA en plus hé ben ça marche donc allons dans le concret, resto juridiquement précis et abrogeant cet article qui n'a aucun sens. Merci Monsieur Bénard Roche puis Monsieur Bonhomme. Mes chers collègues, je, je, je trouve dommage qu'on n'encourage pas un gouvernement dont on a vu depuis longtemps qu'il est profondément écologistes, c'est vraiment dommage, hein, bon, c'est flou, c'est vague, c'est pas de l'de la loi, enfin quand même, bon on pourrait accepter, en fait, c'est du ripolinage vers quand vous parliez de vers, oui, c'est du ripolinage vers c'est-à-dire c'est du verdissement du verdissement au niveau effectivement de coup de cosmétiques ou de pâture alors moi ce que je propose, effectivement, c'est qu'on fasse un amendement ou un article, madame la ministre, ou une loi avec des vrais critères avec des vrais critères écologistes avec des vrais critères qui permettent d'avancer un vrai article de loi qui tienne la route et qui puisse être appliqué. Si Monsieur Bonhomme puis Monsieur Kader. Oui, effectivement, je veux bien croire qu'on doit faire trop d'inventivité, c'est pas pour autant qu'on doit se rallier à un amendement une modification de la scène nationale, qui me paraît complètement baroque et naturellement ça affaiblit ce qu'on croit à vouloir soutenir les exams qu'on a donné notre collègue d'ailleurs disent que de projets ne rentre pas stricto sensu dans des questions dites écologiques, encore que, il faudrait préciser et c'est là toute la difficulté, ce qu'on entend par écologique et et puis je crois surtout que ça vient masquer un peu le l'essentiel, l'essentiel c'est que ça traduit quelque chose de symptomatique, c'est que le gouvernement fait surcroît de de d'inventivité lexicale et de collection de d'objectifs et d'épithètes pour compenser une difficulté qu'ils rencontrent, comme les autres, c'est-à-dire à verdir nos programmes de politique publique mais en dernier le aussi ah si on avait un doute, effectivement, laissant la souveraineté à la commission pour avis de traiter les questions qui doit être sélectionné dans les opérations. Merci Monsieur Kader, monsieur le président. Oui, madame la présidente, madame la Ministre le nombre important d'intervention sur ce sujet montrent que, il n'est pas du tout à exotique, il y a 41 ans, les lois Mauroy de faire abolissez le contrôle d'opportunité sur les décisions des élus locaux. Contrôle d'opportunité exercé par les préfets des préfets désignés vis-à-vis de de maires de présidents de département de présidents de conseils régionaux élus très concrètement par cette proposition issue aujourd'hui est validé par, par vous même vous recréer de fait ce contrôle d'opportunité sur aucune base sérieuse et je pense que l'abrogation que nous portons, que nous allons porter montre que sur l'ensemble de ces bancs ici présents, de droite à gauche, nous voulons préserver l'autonomie des collectivités locales face à un pouvoir central qui devient de plus en plus. Comment je vais vous dire ça prégnant pour acheter polie donc madame la ministre, nous allons vous mettre en minorité je ne sera pas la première fois, ce soir, mais simplement que ce message puisse remonter là où il doit remonter à savoir auprès du président de la République qui, derrière ses engagements régulier juste thématique semble quand même oublier que les élus aujourd'hui sont le tissu social, le tissu de l'aménagement du territoire, dans notre pays. Merci Monsieur Kahn R. : la parole est à monsieur Laménie. Oui merci madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues, très rapidement, simplement je partagerai 6 amendements à l'initiative de nos brillants collègues de la commission des lois avec le président de la commission des finances, et ses collègues parce que je dirais, la DETR a été institué de mémoire en 2011 la déciles en 2016

je rappellerai en 2017 pour celles et ceux qui étaient là, à l'été 2017, le combat notamment de notre collègue qui était président qu'et c'est président buffet maintenant qu'il est président de la commission des lois à l'époque, c'était le président Philippe Bas, qui s'est battu pour défendre la réserve parlementaire la dotation d'action parlementaire et ça fait aussi partie aussi du lien qu'il y avait et puis de la proximité et la et le soutien aussi à l'ensemble de nos collectivités locales voilà mais je soutiendrai ces amendements. Y'monsieur Laménie monsieur de Lège. Merci madame la présidente, madame la Ministre, c'est vraiment l'impression que vous vous tirez une balle dans les pieds, pour une raison très simple : c'est comment vous allez pouvoir comment le préfet va pouvoir définir la qualité écologique dès que vous allez faire une route et vous avez donné une subvention, vous allez trouver toujours un particulier, une association qui va faire un recours, ça va être exactement la même chose avec les maires, et donc je ne vois pas comment vous pouvez défendre cet amendement, d'autant plus que au départ ça ne faisait pas partie de vos projets, comme ça a été dit excellemment tout à l'heure, c'est pas en mettant écologique à tous les bouts de phrases que vous faites pour autant une politique écologique, donc je crois vraiment que dans cette affaire, vous êtes en train d'entraver la capacité d'action non seulement des mères mais aussi d'entraver la capacité d'action du préfet qui va se retrouver avec une série de recours pour rien du tout.

merci et si il y avait encore des choses à dire, oui, oui. Et je je voulais insister, madame la madame Ministre sur le fait qu'en fait, la DETR est un peu le dernier espace de liberté sur nos territoires ou l'Intelligence des élus et la créativité des élus dans le cas d'un dialogue avec la préfecture

la DETR et le l'ultime endroit où on peut présenter, et vous pouvez avoir un dialogue local et une souplesse, l'aide de l'accompagnement de l'État s'adapte aussi pour une fois à la réalité des territoires dont vraiment garder nous cette soupape de réponse à, à l'Intelligence du de nos territoires et des élus locaux. Madame la Ministre, vous avez demandé la parole pour répondre. de tout ce que vous exprimez et je comprends que vous demandez la suppression de la joue de ce critère écologique mais je veux juste vous dire que ce critère. Ben n'y serait pas que vous nous accusez auriez de manque de cohérence, moi j'appartiens aujourd'hui ah. J'appartiens est ce que vous me permettez d'aller au bout, j'en ai pour moins d'une minute, donc soyez respectueux, autant que je le suis de votre pensée vis-à-vis de ce que je vais vous dire j'appartiens Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, ça fait juste 4 mois et demi 5 mois que je suis au gouvernement j'ai chevillée au corps, l'envie d'ancrer dans les territoires, la transition écologique. On a du mal, c'est difficile, on travaille ensemble avec Christophe Béchu sur Lausanne, on travaille sur plein de sujets sur cette loi climat et résilience aujourd'hui juste une minute, je vous ai dit pas plus, et donc on a mis un critère écologique oui dans la DETR moi j'entends tout ce que vous dites, ce que je dis, ne s'oppose pas ce que vous dites, je vous dis simplement que oui, le gouvernement affiche une volonté par là même de voir colorer l'ensemble des investissements qui sont faits sur fonds d'État dans les territoires et c'est juste, je vous demande d'antan de et de et de respecter une opinion qui n'est pas la vente, moi je suis très respectueux de la vôtre. Merci madame la ministre, hein, alors je vais mettre aux voix, donc ces trois amendements identiques de suppression avis favorable de la commission avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, ils sont donc adopté, donc là de monde en suivant tombe l'article est supprimé, alors je vous signale que nous arrêterons vers 20 nous deux amendements identiques alors le 75 Madame Noël. Merci madame la présidente, madame la miss, nous avons tous remarqué une inflexion ces dernières années de dispositifs contractuels et partenariaux, par l'État, type contrat ruralité ou CRTS qui est qui sont la traduction de la volonté de l'administration d'établir une doctrine, contraignant les collectivités territoriales à s'inscrire dans de tels dispositifs pour solliciter certaines dotations d'investissement à l'instar de la déciles certaines communes et particulièrement en milieu rural se retrouvent parfois exclus du bénéfice de certaines ressources et ainsi contrainte de reporter, voire d'annuler leurs projets d'investissement, le présent amendement a donc vocation à mettre fin à cette doctrine purement administrative en fixant un principe législatives selon lequel la collectivité territoriale ne peut se voir exclues du bénéfice d'une dotation d'investissement au seul motif qu'elle ne s'inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariales impulsée par l'État. Merci le 635 madame la présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est un amendement identique, c'est-à-dire que des modifications législatives et pratique et de pratique dans l'État locale fragilise les communes, la mise en place des dispositifs contractuels partenariaux, par l'État, type contrats de ruralité c'est Arthur sont la traduction de la volonté de l'administration d'établir une doctrine, contraignant les collectivités territoriales à s'inscrire dans de tels dispositifs pour solliciter certaines dotations d'investissement à l'instar de la déciles certaines communes et particulièrement dans mon département qui est rural se retrouvent parfois exclus du bénéfice de certaines ressources est ainsi contrainte à reporter, voire annuler leurs projets, cet amendement instaure donc un principe législatif, selon lequel une collectivité territoriale ne peut se voir exclus d'une dotation d'investissement. Merci l'avis de la commission sur ces deux amendements. propositions, qui est reprise de la donc évidemment un avis extrêmement favorable. Merci l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Madame la présidente de retrait sinon défavorable s'il vous plaît. Merci, alors je mets aux voix ces deux amendements identiques : avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour, qui est contre. S'abstient, ils sont, ils sont

C'est très bien, merci, madame la présidente, donc c'est un amendement porté par notre collègue Jean-Baptiste Leblanc et 62 de nos collègues n'est-ce pas qui concerne la DETR, et donc, cet amendement vise à garantir que les crédits de la DETR, ça tue le débat cet après-midi sont bien destinés à l'équipement des territoires ruraux, voilà donc puisqu'on sort de la Cour des comptes à l'Assemblée nationale en passant par les associations d'élus, le Sénat, comme en témoigne la discussion du récent rapport d'information, l'excellent rapport d'information de Charles Guené et Claude Raynal, sur le rôle de la dotation dotation d'investissement pour les collectivités territoriales, le conseil régulièrement dressées de dérapage de crédit, la DETR, qui bénéficie qui pourrait bénéficier à des grandes aires urbaines, que les des tribus dans le cas de la DETR soit ciblée sur des projets réalisés dans des communes où John rurales au sens de l'Insee puisque l'initie à des critères pour pour savoir ce qu'est la ruralité ou tout le moins, sous des projets contribue hein significativement au développement rural, merci, merci. Si l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente, oui mon cher collègue, c'est, c'est quand même remarquablement essayer par la présentation, mais ça ne reprend pas tout à fait notre rapport lorsqu'on juxtapose les critères que vous évoquez, on va dire de de moins de de 20000 habitants comme une peu dense avec les critères actuels, en fait, on ne retrouve que 4000 communes d'écart, d'autre part, l'analyse de ces taux devrait être réalisé au regard des des caractéristiques de chacun des départements parce que lorsqu'on voit par exemple dans un département comme le mien, comparé à celui du du Bas-Rhin, qui ont à peu près la même somme à répartir, hein, voilà, c'est un excellent exemple, les communes ne sont pas absolument la pas de la même taille et en fait ça viendrait rigidifier

La position du gouvernement est défavorable, madame la présidente. Merci, si ce que vous retirez l'amendement Monsieur à suivre les recommandations de du rapporteur retirer l'amendement. Retirer l'amendement merci alors 3 amendements en discussion commune le 76 Madame Noël merci madame la présidente, madame le Ministre. Force est de constater que de nombreuses communes rurales sont privés du bénéfice de la DETR au profit des villes avec la liste des bénéficiaires, fixé par la loi, outrepassant nettement le seul Champ des communes caractérisées comme telle, selon une étude réalisée par l'Association des maires ruraux de France pour les régions Provence Alpes Côte d'Azur et Auvergne Rhône Alpes ce sont ainsi respectivement 6 2 millions d'euros et 15 millions d'euros de DETR qui, en 2022 ont été reversés à des entités, autre que des communes rurales, le présent amendement modifie la liste des bénéficiaires de cette dotation en prévoyant que seuls, ils seront éligibles les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communal de densité de l'Insee.

et j'ai envie dire c'est le bouquet, quand je leur dis vous avez des communes urbaines marrante une membre d'une métropole qui bénéficie de la dotation d'équipement des territoires ruraux, donc je propose simplement que les communes urbaines marbre d'une métropole ne soit plus l'Égypte à l'attention des équipements des territoires ruraux. Merci le 636 monsieur Marie défendu. Non, pas totalement, c'est le même effectivement que mon collègue Delcros, simplement une précision complémentaire l'amendement présenté par notre collègue Madame Noël concentre la DETR sur l'hyper-rural au risque malheureusement de sortir certaines communes rurales de la DETR, alors que celui présenté par ce Delcros et moi-même avec mon groupe, permet de sortir des communes urbaines m'emmener métropole qui en bénéficient, alors qu'elle ne devrait pas en bénéficier.

aussi mais avec la volonté de rendre inéligible est comme une membre de métropole lorsqu'ils remplissent ce type de conditions je trouve que ce caractère est peut-être un un peu d'escrime en et mériterait d'a d'avoir une étude plus plus appropriée, parce que il n'est pas exclu que dans certaines métropoles, on a effectivement des, des, des communes qui qu'il soit dans dans des cas limites et qui seraient donc qui aura un traitement relativement différents et au nom de quoi parce qu'ils sont dans une métropole on les exclurait la Commission préféreraient de pas rigidifier le système parce que les préfets sont quand même là pour faire leur travail aussi et donc c'est plutôt une demande de retrait Madame la présidente, donc en effet, je vous ai proposé tout à l'heure de travailler sur cette Inter'territorialité, je pense qu'on sera amené à travailler de ce sujet sur ce sujet, à ce jour à sept heures sur la base de ces trois amendements le gouvernement

débat le bon moment le bon amendement le bonjour et la bonne heure et le bon texte puisque manifestement, ça ne fonctionne pas, je je vous proposerai quand même de, de bien vouloir éventuellement consulter et donner des instructions aux préfets pour qu'ils soient particulièrement attentifs à ces cas tout à fait limite dans lesquels il peut y avoir des très gros investissements qui en fait des plumes, le reste du département, à cause de très gros investissements DETR sur des intercommunalités qui serait tangente des 50000 habitants prévues par le texte, je pense qu'on peut, dans l'attente des groupes de travail que vous allez former peut être avoir une attention particulière de la part des préfets et qu'on ait plus de latitude pour l'année qui vient jusqu'à ce qu'on ait réglé ce problème et ajusté en attendant en attendant je vais entrer l'amendement de Bernard Delcros. Merci, alors je mets aux voix l'amendement 76 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Ouais. Qui s'abstient n'est pas adopté, je mets aux voix les amendements 210 et 636 qui ont reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour.

Merci madame la présidente, madame la ministre, cet amendement propose de réserver le bénéfice de la dotation d'équipement des territoires ruraux, perçu par les EPCI au au projet qu'ils réalisent sur le territoire de leur commune membre qui sont elles-mêmes éligibles à à la DETR, il ne modifie donc pas le chant des EPCI et des communes éligibles à la DETR, mais porte seulement sur les projets des EPCI susceptible d'être subventionné.

En réalité, cher collègue, nous avons surtout regarder qu'est-ce que ça a donné quoi ça concerne qui, et alors en recentrant donc à DETR alloués aux EPCI sur les seuls projets réalisés sur des communes membres et le même éligibles à la DETR outre que l'on continue à rajouter des éléments je ai dit à à la fois on se bat pour simplifier et chaque fois qu'on peut complexifier on le propose, mais au-delà de ça, je rappelle que. Les établissements les EPCI peuvent par sera de terre si et seulement si la population n'excède pas à 75000 habitants, il présente un territoire d'un seul tenant, et sans enclave et leur communément des populations inférieur à 20000 habitants, il en résulte que cet amendement vise à exclure des dotations perçues par le PCI, les communes de moins de 20000 habitants, qui auraient un potentiel financier supérieur à une 3 fois la moyenne de la strate puisque celle il y a un potentiel inférieur sont éligibles en tant que commune

par ailleurs pas 1000 et 5350 communes comprises entre 2000 et 20000 habitants, seuls 610 un potentiel financier supérieur à 1 virgule 3 fois la moyenne de la strate et parmi ces 610 certaines sont membres d'un EPCI dont la population est supérieur à 75000 habitants, bon, il en résulte qu'il existe très peu de cas. Et que donc on crée un élément nouveau pour pas grand chose donc demande de retrait.

Merci madame la présidente, madame le ministre, cet amendement a simplement pour objet de déplafonner la participation maximale de, de, de la participation, petite de la DETR, généralement il est fixe à 40 % je propose de le porter à 80 %. Il la visite de la commission, monsieur le président. Oui, chers collègues, on est là plutôt dans le domaine réglementaire, on est certainement pas dans le domaine de la loi d'retrait. Merci madame la ministre, de l'avis du gouvernement, de même un retrait merci ce que vous retirez merci,

mes chers collègues, vous l'avez déjà évoqué, nous avions avant la réserve parlementaire pourrait des petites communes qui avaient des petits projets, or aujourd'hui de plus en plus de préfecture fixe dans leurs circulaires portant portant attribution de la DETR, un montant minimal de dépenses subventionne Naples en dessous duquel les communes ne peuvent susciter cette dotation certaines communes se voient ainsi refuser le bénéfice de la DETR au motif que le coût de leur projet n'est pas suffisant suffisamment élevé le présent amendement entendent donc interdire cette pratique, je vous remercie. Merci, alors l'amendement 79 Madame Noël défendu merci l'amendement 467 Monsieur Bénard Roche. Oui, madame la présidente, effectivement comme l'a dit ma collègue, nous souhaitons améliorer l'attribution de la de la DETR face aux pratiques pénalisante pour certaines communes qui ont été constatés par des élus locaux et l'appareil en fait que de plus en plus de préfecture fixe dans leurs circulaire portant attribution de la DETR, un montant minimum de dépense subventionne able au-dessous duquel les communes peuvent solliciter cette dotation, c'est la raison pour laquelle certaines Covid se voir refuser le bénéfice de la DETR au motif que le coût de leur projet n'est pas suffisamment cela pénalise directement les plus petites communes, orientant les dotations vers de plus gros projet en général portés par des collectivités plus importante le présent amendement qui en fait issus de propositions de la RS, l'association des maires ruraux de France autant donc interdire cette pratique. Merci même Préville inverse. Si madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, donc effectivement je comme mes collègues l'ont dit des préfectures fixe dans leurs circulaire portant attribution de la DETR, un montant minimal de dépenses subventionne able or lorsque vous êtes une petite commune rurale et que vous avez un projet modeste, hé bien, vous ne pouvez pas prétendre à une aide de la part de l'État sous forme de DETR, ce qui est évidemment un frein et pour pour moi qui suis élu d'un département où il y a énormément de petites communes, voire même de moins de 100 habitants, voilà, c'est donc quelque chose qui remonte beaucoup des territoires merci.

pour l'attribution de la DETR pour tous les arguments qui viennent d'être développés et notamment pour que les plus petites communes puissent y avoir accès, mais je voudrais insister sur un point qui est peut être en tout cas je l'espère, un peu plus conjoncturelle, c'est que nous allons avoir dans les prochains mois les prochaines années un sujet investissements dans les communes et dans les plus petites en raison de la situation financière dans laquelle elle se trouve en raison de l'inflation et je ne vais pas développer ça ici, et donc particulièrement dans la période si on veut, parce que la DETR, ça a quand même un impact sur le tissu économique et je dirais le tissu économique le plus, enfin, l'artisanat, et cetera dans nos territoires, voilà pourquoi il est important que les plus petites communes puissent en bénéficier sans seuil. Merci l'avis de la commission, monsieur le président. D'abord, madame la présidente, je voulais me féliciter que nos rapports si bien lu et si bien retraduit donc je ne pensais pas qu'on avait un tel succès et donc on avait indiqué effectivement qui avait en cours, un mouvement qui allait dans ce sens d'une fixation minimal par les préfets pour s'en inquiéter, on n'avait pas fait d'amendements parce qu'on considérait il fallait voir attendent de voir comment ça se mettait en place, mais de fait, c'est une réalité alors pas dans tout, dans toutes les préfectures mais dans quelques-unes, on comprend bien qu'il y a une question, une volonté d'économie de gestion si je puis dire, au sein des préfectures, on comprend qu'on prend l'objet si je puis dire, bon, on a été maire tous c'est commencer essayer de gérer au mieux, sang, maître des d'effectifs supplémentaires, mais en même temps c'est contraire à l'esprit à l'esprit de la DETR c'est contraire au fait que on est effectivement notre propre enveloppe qui parlementaire qui a été mise à la DETR et qui était pour l'essentiel consacré à des tout petits projets et donc nous sommes favorables à ce que on indique clairement que, on ne peut pas mettre de critère minimale dans les critères de DETR il y a des critères qui sont fixées par la loi, on en reste là, et on essaie de faire en sorte que les préfets soient ouvert à tous les projets que ce ne soit pas une barrière. Donc favorable, Monsieur le Président merci l'avis du gouvernement, Madame la ministre. Merci madame la présidente, je vous rappelle que la fixation des catégories prioritaires, ainsi que des taux minimaux et maximaux de subventions sont du ressort de la commission départementale des élus et non des préfets si cette pratique est reprise dans les circulaires de certaines préfectures, c'est qu'elles ont été décidées et validé par ces commissions, subvention inférieur à 5000 euros 5570 projets ayant bénéficié d'une subvention inférieur à 5000 euros, il semble donc que cet amendement. Introduirait des rigidités au niveau local sans véritables besoins avérés des projets de montant limité reste donc bien soutenu, grâce à la DETR, la gestion des dotations d'investissement aux collectivités volontairement déconcentrer, cela répond à une demande locale mais aussi un nécessaire pragmatique. Il me semble vraiment nécessaire de conserver ses principes, l'avis du gouvernement et le retrait sinon défavorable merci. Merci monsieur Richard. merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ma mamie, je sais pas qui a fixé ça toujours est-il que ce un chiffre existe et et clairement il n'est pas possible de subventionner au titre de la DETR des petits projets c'est c'est je crois qu'il faut d'autant plus changer ça, Madame la Ministre que en terme en terme dimanche c'est juste catastrophique pour les mères qui reçoivent un courrier qui reçoivent un courrier qui leur dit le sous-préfet, leur dit : écoutez, votre projet n'a pas pu être retenue parce que, tenez-vous bien les le, la motivation est expliqué le le montant qui qui est demandé par votre commune est trop faible, trop fait pour bénéficier alors quand vous savez que ce sont les tout petits projets et ça a été dit tout à l'heure, ça va empirer compte tenu du

par des communes, auxquelles on a donné ce type de réponse c'est désastreux désastre donc une commune qui peut pas faire d'autres projets que ce petit projet comprend pas

Oui, madame à la ministre, franchement, je pense qu'il faudrait que vous reveniez sur votre décision tout simplement parce que c'est même pas des projets à sept mille euros je crois que vous ne connaissez pas les communes rurales, des fois, ce sont des projets de de mille euros pour eux, c'est beaucoup de surface, ce sont des projets des gros projets pour eux donc je crois que vous connaissez pas les communes rurales et franchement, ça me ferait bien plaisir vous reveniez sur une telle décision, je vous remercie. Merci alors ah pardon, madame la présidente de. Juste Juste pour rebondir sur les propos de Madame la Ministre quand elle dit que la commission à la main, mais la commission ne voit que les projets au-dessus de 100 mille donc, de toute manière, ces sommes-là, nous ne les voyons pas, c'est-à-dire qu'elles ont déjà été éliminés, et nous ne voyons pas ses projets les critères, moi j'ai une commission DETR le 5 décembre je vais demander dans les critères par exemple que les communes qui ont subi des incendies puisse avoir des compensations dans la DETR, je sais déjà qu'elle va être la question, on va me dire : mais non c'est pas possible, ça a pas été visés par le PLF et cetera, donc moi je crois qu'on n'a pas vraiment beaucoup de marge de manoeuvre en tant qu'en tout cas, il est vrai que si on a ce débat dans l'hémicycle, c'est vrai qu'on souhaiterait que des consignes redescende auprès des préfets, on a déjà essayé mais là effectivement, Madame la Ministre, ce qu'on souhaite vous dire, c'est qu'il faut vraiment que vous fassiez redescende ses consignes là dans au auprès des des préfets parce que dans les commissions n'a pas vraiment la main pour changer les critères, ça se passe pas vraiment comme ça. Merci, alors je mets aux voix donc ces cinq amendements identiques : avis favorable de la commission avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, ils sont donc adopté amendement 80 Madame Noël. Merci madame la présidente, madame la Ministre, le premier amendement vise à fixer un délai de réponse maximale de 3 mois de l'administration pour répondre aux demandes de subventions et le second vise à fixer un délai minimum de 6 mois à compter du lancement des appels à projets département pour déposer leur dossier.

Alors cet amendement prévoit de fixer un délai minimum de six mois pour solliciter une subvention de on peut comprendre l'objectif le principe car les délais pour déposer une demande serait effectivement très court, entre un et 2 mois à la suite de la publication de la madame je retrouve Madame Noël de la circulaire, cependant, cependant, les élus anticipe souvent leur projet et de fait et l'élaboration de leur dossier avant même la publication de la circulaire annuelle par ailleurs l'article du code général des collectivités territoriales prévoit que ces subventions doivent être notifiés en totalité, c'est ça qui est le point important, finalement doivent être notifiée en totalité au cours du 1er trimestre de l'année civile en fixant un délai minimum donc de 6 mois pour déposer une demande, monter des des dossiers bah la notification au cours du 1er trimestre deviendrait impossible, or les élus s'ils ont besoin de temps, on le comprend, pour monter leurs dossiers ont également besoin de temps, de temps court pour recevoir les crédits le plus rapidement possible afin d'engager des investissements, donc on est entre deux deux intérêt finalement mais comme finalement le code général nous impose la notification à 23 moi je vous propose le le retrait de cet amendement

alors quand la réponse est positive, ce délai est respectée, puisque l'article L 23 trente-quatre trente-six du CGCT prévoit déjà que les subventions doivent être notifiée en totalité au cours du 1er trimestre comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure par défaut et, en creux, les collectivités qui n'ont pas reçu de notification peuvent en déduire condition qui connaissent la règle évidemment que leur projet n'a pas été retenu, donc cette absence de notification pour les projets rejetés peut cependant effectivement poser certaines difficultés et d'ailleurs notre amendement visant à fournir la liste à la Commission de terre de tous les projets recevable mais non retenu répond à cette difficulté de manière à ce que, ensuite, quand vous êtes membre de la commission puissiez revenir rapidement vers les communes, avant même qu'elles reçoivent une lettre de refus de la préfecture pour déjà leur indiquer que leur projet n'a pas été retenu donc demande de retrait également. Merci l'avis du gouvernement, Madame la Ministre, sur ces deux amendements 80 et 81 avis défavorable pour les de de la part du gouvernement pour les raisons évoquées merci

cet amendement vise à déployer, à titre expérimental une évaluation environnementale des projets territoriaux qui pourraient être financées par la dotation de l'équipement des territoires ruraux, la DETR ou la dotation de soutien à l'investissement local à voilà ce que je vous propose, c'est-à-dire un vrai critère et non pas celui d'écologie, comme nous avions tout à l'heure qui était floue, mais un quelque chose d'expérimental, une évaluation ex qui serait réalisé pour chaque projet et d'abord sollicité par une métropole et aidés par la mission régionale d'autorité environnementale aussi au soutien d'un de ses de fonds l'expérimentation ne concerne dans un 1er temps que les projets des métropoles dans la mesure où elles ont les capacités d'ingénierie pour réaliser de telles évaluations dans un second temps, et une fois la méthodologie poser ses une étude pourrait être généralisé à toutes les collectivités porteuses de projets améliorer le pilotage et financement public dédié aux collectivités doit aujourd'hui être une nécessité un tel mécanisme permet de répondre entre autres au référé de la Cour des comptes du 23 juillet dernier critiquant vertement le pilotage par l'état de ses concours financiers à l'investissement public local au travers des 2 principales dotations que sont la ici la DETR, et notamment je mentionne dans ce rapport de la Cour des comptes, le ciblage géographique et sectorielle problématique la soutenabilité incertaine et la gestion fragile ou encore une démarche de performance inabouti par cet amendement on cela permettrait à l'État d'avoir les outils et aux collectivités Turriers territoriale de suivre et d'évaluer l'efficacité et des impacts des différents investissements vis-à-vis de l'urgence climatique, l'analyse de l'exemplarité des projets portés réalisées par les territoires devra se faire au regard de critères précis, défini en lien avec les l'estrade. l'amendement 465 Monsieur Bénard Roche. Je comptais dire défendu mais du coup je termine la phrase en disant que les critères précis et définis le sang en lien avec les PC a été mais aussi l'estrade tu et les projets de territoire a fait s'assurer du réel bénéfice pour l'environnement. Ainsi beaucoup l'avis de la commission, monsieur le président. Alors on a, on a un petit problème d'écriture de l'article, puisque cet article finalement parle des évaluations environnementales par les métropoles et les projets financés par la DETR et la déciles or par principe les métropoles sont par principe exclus du bénéfice de donc ce n'est pas le cas évidemment des communes de certaines communes membres de la métropole, mais telle que rédigée l'amendement il précise bien qu'il ne concerne que les projets des métropoles elles-mêmes et donc c'est inopérant et donc demande de retrait.

alors je mets aux voix donc ces deux amendements identiques 406 465 donc avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient ne sont pas adoptés, alors

OK, tout le monde est d'accord, ça va bien, bon, ça marche, alors le 629 monsieur Marie. Merci madame la présidente, cet amendement qui est proposé par notre groupe vise à donner aux préfets de département, le rôle d'attribuer des subventions au titre de la dotation de soutien à l'investissement local comme il le fait pour les crédits de la DETR en lieu et place du préfet de région, par ailleurs, cet amendement crée une commission départementale des investissements locaux chargés de contrôler la répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux et de la part départementale de la déciles, cette commission est modelé sur l'actuelle commission DETR mais ses compétences sont renforcés, elle serait ainsi signataires de la liste des demandes de subventions aux préfets de département et appelé à formuler un avis sur la liste complète des subventions projeté cela ramasse l'ensemble des demandes que nous formulons chaque année. Si l'amendement 153 qui le défend.

et un pouvoir très faible de la commission des élus afin de remédier à cette situation, le présent amendement propose de rendre obligatoire la communication à la Commission de l'ensemble des dossiers déposés d'abaisser à 80000 euros contre 100000 euros actuellement, le seuil du montant de subventions au-delà duquel l'avis de la commission et requis contraindre le préfet à respecter les catégories prioritaires d'opération à financer, fixé par la Commission prévoir que le préfet rendent compte à la commission de ses choix et des critères retenus pour sélectionner ou rejeter les demandes de subventions, enfin, des critères excluant une commune du bénéfice de la DETR autre que ceux fixés par la loi ne doivent pas pouvoir être prévu dans le cadre du règlement départemental certains départements mettent déjà en oeuvre, à l'initiative du préfet, une partie des dispositions en matière de transparence prévus par le présent amendement toutefois les bonnes pratiques restent trop rare, c'est pourquoi il convient de les généraliser par la loi, je vous remercie. Merci, moi je vais vous demander quand c'est pas votre amendement de faire soit défendu ou franchement très, très court, parce que sinon on n'y arrivera pas à 20 heures 15 merci beaucoup madame, je pense que c'est Madame Estrosi Sassone pour le 378. Oui, alors se présente cet amendement au nom de notre collègue Jean Marc Boyer et d'un certain nombre de nos collègues qui ont été signataire l'amendement permet aux parlementaires de demander l'attribution d'une dotation d'action parlementaire et que 20 % de l'enveloppe DETR soit affectée à cette dotation parlementaire cet amendement prévoit également que l'ensemble des parlementaires et quelles que soit leur nombres dans un département soit tous membres de la commission DETR et enfin, il précise que les parlementaires ne vote pas, lorsque la commission DETR se réunit sur les projets qui serait présenté par ceux-ci, en effet, cela reviendrait à leur demander de se prononcer sur des projets qu'il propose et il pourrait être à l'origine de sources de conflit d'intérêts

en faisant en sorte qu'on soit en en transmettre avant la fin du 1er trimestre chaque année la liste complète de l'ensemble des opérations éligibles est recevable et non plus simplement, c'est la subventionner. Si le 451 monsieur Sautarel. madame la présidente, la ministre cet amendement déposé par notre collègue Jean-Baptiste Leblanc et signé par nombre d'entre nous, vise à ce que le préfet expose les raisons des refus aux communes qui n'aurait, dans les dossiers n'aurait pas été retenu au titre de la DETR, merci.

qui, lui, vise à élargir les pouvoirs de la commission DETR dans chaque département afin qu'elle puisse non seulement donner un avis sur les projets importants mais décisionnaires sur les demandes de subventions au titre de l'ensemble des dossiers de la DETR. Si le 390 Madame Goulet. Alors, mais un président de la la Ministre c'est un amendement qui a déjà reçu plusieurs vote favorable du Sénat, il s'agit de la motivation des refus DETR donc, ce qui semble une logique quand même pour que les maires sache pourquoi on le refuse, la DETR, donc il s'agit d'une demande de motivation que le Sénat déjà voté plusieurs fois. Merci, 2 amendements identiques le 32 madame. Défendu.

Oui merci madame la présidente, il s'agit de de créer pour pour la déciles une commission à l'image de celle qui existe pour la DETR, donc au niveau régional, qui intégrerait aussi un certain nombre d'élus. Merci beaucoup, l'avis de la commission sur ces amendements, monsieur le président. donc tous les amendements ont pour objectif d'augmenter les pouvoirs de la déco de la commission DETR et ou d'améliorer son information, il nous semble indispensable de garder le meilleur équilibre possible entre l'association des élus et les prérogatives du préfet pour

s'agissant de la décide cette amélioration pourrait passer par une saisine pour avis, non contraignant du président du conseil départemental sur les projets subventionnés au titre de la décide des améliorations sont également prévues en matière d'information des commissions DETR en 1er lieu nous proposons une communication à la commission DETR de l'ensemble des demandes de subventions dès lors que le dossier est bien éligible, afin de mieux cerner les critères de sélection appliquée par les services de l'État et vérifier le respect des priorités fixées par les commissions, en second lieu, nous proposons d'inscrire dans la loi l'obligation d'une communication annuel du préfet des départements à la commission DETR sur l'emploi de la décide, dans le département, comme c'est déjà le cas pour la cette information permettrait ainsi de trouver un juste équilibre entre l'association des élus et les prérogatives du préfet pour l'octroi de crédits d'investissement en provenance de l'État et permettrait également aux membres de la commission d'avoir une vision exhaustive de l'emploi de subventions d'investissement dans leur département, ils nous paraissent tous ces amendements de nature, présenté par la Commission de nature à répondre aux préoccupations dont les élus locaux nous ont fait part à l'occasion des travaux de contrôle que nous avons menées sur le sujet sans alourdir démesurément les procédures, je tiens d'ailleurs à souligner que la commission des lois a déposé des amendements identiques aux nôtres, ce qui, depuis que je suis rapporteur spécial est une innovation que je salue nous vous invitons nous vous invitons donc à vous rallier opposition clairement exprimée par nos 2 commissions et par conséquent à retirer vos amendements avec lesquels ils sont incompatibles,

on vous propose de la sagesse sur la 378 c'est celui. La réinstallation de la réserve parlementaire même sur le proposait pas osé qui serait votée, donc si vous voulez, on préfère être populaire, comme disait l'autre, on on en a pris suffisamment sur la cafetière, toute la journée, donc on termine oh les embouté et et la demande de retrait, donc sur tous les autres, merci. Merci madame la ministre, l'avis du gouvernement aussi rapidement, on serait parfait.

Mais je n'ai pas de 22. Ah, il est après non, donc il n'est pas défendu là, celui là, pour l'instant, hein, ah oui oui. Bon,

Bon alors je je vais mettre aux voix, donc les les amendements alors 629 avis défavorable de la commission et du Gouvernement retrait le 153

Trois donc 292 et 410 qui sont identiques de la Commission, avec un avis défavorable du gouvernement qui est. Pour un contre qui s'abstient et donc son donc adopté le 451 Monsieur Sautarel retirer le 160 et retirés merci 390 Madame Goulet il est pas retiré, donc je le mets aux voix donc défavorable commission gouvernement qui est pour. Ah oui, qui est contre. Qui s'abstient donc adopté. Amendement 32 McGuinness retirer vous le maintenez donc défavorable commission du gouvernement qui est pour.

Alors je vais reposer une question est-ce que vous pensez qu'en un quart d'heure on fini complètement le texte.

madame la présidente, je crois que c'est, c'est très simple et il faut faire une présentation en 3 secondes, voir sur défendu, écoutez la réponse de la ministre voilà. Donc fait ça, si on fait ça, je vous rappelle que samedi, il y a grève des trains, donc plus personne ne va pas revenir, Alors qu'il n'est pas d'accord sur ces amendements, juste des 10 défendu qui n'est pas d'accord, OK, on y va

avis de la commission. La commission, monsieur le président. Demande de retrait, Madame la Ministre,

Qui est contre qui s'abstient donc adopté je mets aux voix, l'article 45 et pour contre qui s'abstient adopté

Donc je mets aux voix cet amendement, donc avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre.

Qui est contre. Je mets aux voix l'article quoi 45 quater, qui est pour, contre qui s'abstient adopté Mandement 444

Il est défendu et je veux attirer l'attention sur le fait que on a prévu les crédits pour cet amendement, pas pour le précédent. Alors Monsieur Delcros. Pas entendu c'est bon, bon voilà 226 n'pas défendu, bon il y a personne, le 397 madame De Lattre défendu et le sous-amendement 987, monsieur le président Gontard défendu. Il est défendu oui. Merci donc avis de la commission. Sur le 447. Bien plus globalement sur tous ces amendements, on est favorable sur le 50 de monsieur Delcros de toute façon, que ce soit clair et de de cette manière mais bien entendu c'est il serait intéressant que les autres se retire, notamment le 447 le sous-amendement on est défavorable. Défavorable au sous-amendement OK, hé à du gouvernement, Madame la Ministre, sagesse et sinon même avis. Sagesse sur le cinquante et sur le sous-amendement. Comme la commission. Merci donc le 447 Monsieur soutar elle vous retirer. le cinquante ans oui le sous-amendement, donc avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre.

favorable, favorable, favorable. OK, donc je mets aux voix là cet amendement 151 vie favorable qui est pour.

défendu avec du de la commission défavorable merci avis du gouvernement, Madame la Ministre, favorable, favorable, donc je mets aux voix donc le 152 avis défavorable de la commission favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Bon, on refait avis défavorable de la commission assez favorable.

D'accord, donc je mets aux voix défavorables, Commission et gouvernements qui est pour. Contre qui s'abstient mais donc pas adoptée selon procéder au vote, nous allons procéder donc au vote des crédits du compte spécial avances aux collectivités territoriales figurant à l'état des, je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite je vous rappelle que la commission des finances, est favorable à l'adoption des crédits du compte spécial, je me vois les crédits du compte ce spécial qui est pour. Qui est contre qui ça devient ils sont bons, accord. monsieur le président Gontard. C'est un rappel au règlement, oui. Oui merci madame la présidente, non, juste un un rappel au règlement par rapport,

et que ça pose quand même la question de l'organisation générale de la et de la manière dont on dont il n'étudie ce ce budget et que je pense que voilà, on ne peut pas se satisfaire, en tout cas de cette manière de de fonctionner, je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 21 heures 40 pour l'examen de la mission Agriculture alimentation forêt et affaires rurales, la séance est suspendue.